Collègues, la séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023. Dans la discussion des articles. Nous sommes parvenus au sein des amendements de suppression de l'article 1er bis à la présentation de l'amendement numéro. 1320. Donc je donne immédiatement la parole. À Madame 13 villes. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. La retraite à points c'est encore à un ancien 1er Ministre qui en parlent le mieux. François Filon Fillon pardon dans un moment de vérité, de sincérité. S'adressant en 2016 à des dirigeants d'entreprise, je le cite, le système de retraite par points. En réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue de les, de baisser chaque année la valeur des points et donc de diminuer le niveau des pensions, voilà qui est dit. À bon entendeur. À travers cette demande de rapport, c'est le spectre d'une nouvelle réforme qui pointe son nez. Et à très court terme. Avez-vous seulement mesurer comment les Français vont vivre cette nouvelle remise en question du système social français. Vous voulez malmener tout bonnement en les plongeant dans l'incertitude. L'inquiétude et pour tout dire la peur du lendemain et de l'avenir cela confine à un projet pyromanes devant l'inflammabilité de la situation actuelle. Cette demande de rapport questionne ce qui nous constitue la solidarité va être tout simplement balayée et c'est le chacun pour tous ce qui prévaudra dans notre devise notre triptyque républicain Liberté Égalité Fraternité. C'est la fraternité qui lient la liberté et l'égalité, et qui ont et qui pour lui donner toute sa valeur humaniste. N'oublions pas ceci, la solidarité, la fraternité doigte. Et doit être là des dans la déclinaison de nos de tous nos projets de loi. Et parce que nous devons l'incarner commerciaux. Merci, cher collègue, la parole est maintenant à Madame Monnier. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à supprimer l'article 1er qui prévoit la remise d'un rapport sur la possibilité et les conditions et le calendrier de mise en oeuvre. D'un régime universel c'est-à-dire régime de retraite à points. Maintenir cet article conduit à nourrir encore davantage la confusion de nos concitoyens et concitoyennes entretenu par les aller retour du président de la République sur le sujet. En témoigne, cela dit. La ration du 25 avril 2019 à l'occasion, à l'occasion d'une conférence de presse dans le cadre du grand débat national. On laisse 62 ans comme âge légal pour faire une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus profonde qui est de créer ce nouveau système par points. Qui va permettre la confiance. La forte mobilisation sociale avait à l'époque contraint le gouvernement à renoncer à la mise en place d'un régime universel à points. Il sait aujourd'hui fixé hein. Un nouveau. Un nouveau cap semble-t-il loin peut être de cet horizon 1er celui d'une réforme paramétrique avant tout dictés par des objectifs financiers. Dans un contexte où les Françaises et les Français s'interrogent à raison sur la réalité de ce que prévoit cette réforme au regard des incertitudes et contre-vérités qui se confirme de jour en jour. Cette a encore un nouveau signal contre-indiqué. Bonsoir à rebours qui est envoyé l'inquiétude ne cesse de grandir avec cet article et ce que l'on a eu déjà comme débat précédemment on entrevoit l'ouverture de la porte vers le régime de retraite à points.

L'introduction d'un tel rapport sur l'affût sur une future mise en oeuvre d'un système universel de retraite. Intégrant qui plus est, les paramètres de la réforme prévue par la présente loi me paraît tout bonnement anachronique nos compatriotes ont déjà exprimé leur refus massif en 2019 et 2020 souvient du chaos provoqué par le déclenchement du 49.3. À la veille du grand confinement. Vous ne pouvez pas refaire le match par le truchement le truchement de ce texte. Ainsi, tant sur la question de la méthode que sur le fond mon amendement demande la suppression de cet article 1 bis. Merci. Merci Monsieur prison un amendement de suppression de donc de cet article. D'abord parce que je me demande ce que viennent faire un rapport sur un nouveau système de retraite dans un une projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale et je me demande effectivement s'il n'y a pas un risque d'inclus, constitutionnalité. À ce sujet il main. Les Français ont rejeté en 2019 la réforme du système universel de façon massive et je ne rappellerai pas ici les grèves dures qui ont marqué cette lutte. Seule la crise Covid a permis de sauver du gouvernement, il avait une autre urgence est réelle celle-là. Et voilà que vous remettez l'ouvrage sur le métier et que vous voulez nous imposer très rapidement avec un rapport de un an seulement votre retraite universel vous êtes vous, vous dites très attaché au système par répartition. Mais vous faites tout pour le faire disparaître. Nous ne sommes pas d'accord oui. Nous défendrons notre système de solidarité et qui était historique bien puisque créée par le CNR et nous ferons connaître nos intentions de vos intentions de réforme caché à l'ensemble de nos concitoyens. Merci madame Meunier n'est pas là. Madame bonne foi non plus. La parole à Monsieur le comte. Oui, merci Monsieur. Le président Monsieur Miss mes chers collègues d'abord comme l'a indiqué, notre collègue Alain Millon. Je m'interroge sur le sens finalement de laisser dans un texte, un amendement dont nous savons déjà qu'il sera retoquée par le Conseil constitutionnel puisque non conforme à la loi organique relative à aux lois de financement de la Sécurité sociale. Deuxièmement, je me demande comment nous pouvons avoir confiance finalement dans le Parlement et d'une manière générale dans l'action politique, si nous votons des à un rapport qui acte le fait que la réforme qui est discuté, ne sera pas satisfaisante. Bon en tout cas pour ceux qui l'ont proposé et pour ceux qui vont la voter. Nous ne pensons pas qu'elle est satisfaisante et nous pensons qu'il y a d'autres choses à faire. Enfin. Puisque c'est une réforme ce rapport demande de revenir. À à la retraite à points. La retraite à points quand même de grosses difficultés, d'abord elle. Elle n'a plus aucun caractère redistributif puisque les pensions sont strictement fonction du nombre de points accumulés et donc pas de carte. Pas de caractère redistributif et aucune capacité de prendre en compte les accidents de la vie, donc cette retraite à points posent des problèmes fondamentaux. toutefois il est clair qu'aujourd'hui nous avons une réelle difficulté avec un système de, des systèmes de retraite qui sont. L'ombre. Et finalement des carrières qui sont beaucoup moins linéaire qu'il y a 50 ans avec plus de la moitié des Français qui sont des polypensionnés et je ne parle pas de ceux qui font une partie de leur carrière à l'international et par conséquent s'il devait y avoir une priorité aujourd'hui c'est pas de tout casser pour reconstruire quelque chose qui a, qui aurait des des des des des défauts fondamentaux mais c'est de créer des passerelles entre les différents systèmes pour que en particulier par rapport au régime général et le calcul du taux et le calcul du de des des meilleurs compatibles avec l'intérêt des polypensionnés et des personnes qui ont une partie de leur carrière à l'international, ce qui n'est pas le cas de la situation actuelle et ce sera encore pire, après la réforme puisque elle posera des conditions de cotisations et d'âge qui ont clos la situation encore plus difficile, je vous remercie. Merci. Monsieur Todeschini n'est pas là Monsieur Jomier non plus le président Kader merci. Si Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Finalement cet article 1er biche c'est pas, c'est un article anodin incolore, inodore exotique. Non. C'est un article terriblement politique et. Je ne connais pas sur les arguments de fond concernant la retraite par points mais. On dit que c'est l'amendement de monsieur Ferracci. Grand. Député. De renaissance proche de du président de la République. Excusez-moi, je crois que c'est pas l'amendement Ferracci un amendement Macron. Clairement, faut appeler un chat un chat. C'est un amendement du président de la République parce que ce n'était pas dans le texte initial. Ça a été rappelé à plusieurs reprises et on se le retrouve là dans la navette. Alors que rien n'obligeait le gouvernement à pouvoir le, le reprend donc. Prennent République dans ce dossier, c'est le pompier pyromane l'apprenti sorcier, les deux en même temps vous choisirez. Mais la question. Que je voudrais poser au ministre et j'espère qu'il pourra me répondre tout à l'heure c'est mais pourquoi cet article. Qui a une connotation manifestement systémique. Dans un projet de loi qui se veut paramétrique. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas.

J'ai l'impression que concernant, concernant. La retraite par répartition, c'est un corbillard peut en cacher un autre. Et nous on est contre les corbillards concernant la retraite par répartition. Donc, nous voterons contre cet article 1er bis. Merci monsieur Joly n'est pas là la présidente Rossignol. Merci, merci Monsieur le Président, je vais être relativement rapide parce que j'étais déjà intervenue sur cet article premier bis et que notre but n'est pas de ralentir les travaux du Sénat pour ralentir les travaux du Sénat. Je ne savais pas comment faire pour vous faire plaisir en ce début d'dimanche après-midi et dimanche on est tous ensemble, dès qu'elle petit signe pour-je envoyer. À, à nos collègues. Et donc je n'aurai qu'une seule question pourquoi parmi tous les amendements qui ont été qui ont été adoptées à l'Assemblée nationale et que le gouvernement n'a pas choisi de retenir sort différent a bénéficié d'un sort différent des autres. Pourquoi vous avez absolument voulu le garder et j'imagine pas un instant que ce soit pour des raisons d'amitié que qui que ce soit et voulu faire préside plaisir au président de la République en conservant un amendement d'un de ses amis. Ce serait vraiment indigne de la République et jamais dans et jamais dans votre façon de présider le pays. Merci cher collègue. Et donc le 2027 monsieur Dufour. monsieur le plaisir, merci. Si le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement a pourvu de la suppression de l'article Miss car il prévoit effectivement la convergence des du régime après le an de la promulgation de la loi effectivement cela priverait des régimes autonomes de leur capacité et c'est la raison pour laquelle le régime des des avocats. Bon et, et particulièrement. À à ce texte d'ailleurs cet élément a été retenu publiquement par la Première ministre donc suppression de cet article, merci. Merci, monsieur Jean Sanitas n'est pas là. L'amendement de des rapporteurs chez madame Jouanno. Merci monsieur le président, chers collègues. 59 amendements de suppression. Je pense que je n'ai pas grand chose à dire parce que je pourrais être soupçonné d'être de l'anti-monnaie d'un petit poney. Donc je m'arrête là et je dirais que tout a été défendu. Merci Madame Espagnac. Défendu défendu. Ensuite le. Madame Guy dès.

La présidente Gruny excusez-moi. Merci monsieur le président. Ben moi je vais juste simplement vous dire que. La confiance qu'on qu'on peut obtenir en fait. De l'ensemble des Français, c'est de ne pas changer de ligne tous les quatre matins Cette étude, je suppose qu'elle avait déjà été fait sur le système. Le régime universel par points elle revient là au détour de cette loi, je vous assure que ça ne peut pas donner confiance et moi je voudrais juste attirer votre attention sur la situation des artistes, auteurs que si jamais vous recommencez une étude de bien vouloir ne pas oublier leur spécificité. Merci. Ensuite Madame Poncet Monge. Merci monsieur le président, alors. Moi je crois qu'effectivement. Ça sa place ici parce que c'est la prochaine étape et cette cette attaque là elle est pas prête depuis. 2019 allait prête depuis 2017 en fait de quoi il s'agit vous l'avez voté raboter tous les régimes qui sont plus. Auteur hein. Nous allons aggraver presque tous les paramètres, on l'a bien vu. Contre ça effectivement pour faire passer la brutalité de la réforme on donne on rendra 3 milliards sur les 18 qu'on a cagnottée. Mais surtout, surtout, cette réforme bloque le paramètre de l'augmentation des cotisations et c'est pas du tout un hasard parce qu'il faut. Il faut bleuté. Ce paramètre parce que désormais, et vous le savez il faudra augmenter les ressources et en partie il faudra augmenter les cotisations. Mais vous voulez pas que ça aille dans le 1er et le 2ème étage de la fusée. Vous voulez que ça aille dans le. Et là pour dans le troisième il y a plus de problème de pouvoir d'achat, il y a plus de problème de compétitivité. Mais il faut que ces cotisations nécessaire qu'qui devrait être augmentée partent dans le 3ème étage. Ce que je veux dire ce que vous voulez faire exploser un principe qui là et de gauche, Monsieur le Ministre. Qui dit De chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins en fait. Là quand vous adhérez au principe un euro doit donner le même nombre de de 2 points. Tout ce que vous dites, c'est que c'est de chacun a selon ses moyens et à chacun selon ses moyens. Toujours selon les moyens et là aussi nous aurons quelques mesures d'atténuation vous donnerez de ci, de là des points gratuits c'est gentil mais un peu dans la même proportion du 3 18, c'est-à-dire d'un sixième. Donc il s'agit effectivement. C'est tout à fait cohérent que ça soit là on. Les cotisations et après on demande l'abondement de l'employeur. La défiscalisation et on demande aux salariés. Devant la baisse des pensions programmé par toutes vos efforts, il faut conclure. Je conclus vous de dites aux salariés. Il y a qu'une solution c'est le troisième étage et celui-là il est en capitalisation. Merci. Ensuite. 44 03. Madame Gréaume. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Notre système de retraite par répartition est un des fondements de notre système social, c'est un bien précieux et un symbole de notre nation, notre objectif est de le préserver ce sont les mots de la Première ministre Élisabeth Borne. Cet article abysses confirme au contraire nos craintes ce que vous poursuivez comme une chimère. C'est la destruction profonde de notre système de retraite et sa transformation en régime universel à points qui serait réévalué chaque année vous remettez sur le tapis un projet dont personne ne veut un projet qui va renforcer les inégalités que vous avez contribué à créer avec le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Un projet d'autant plus regrettable, qui procède à une réforme du Route du système de retraites inédite depuis 1945 les destinées à transformer pour les décennies à venir. Un système social qui constitue l'une des composantes majeures du contrat social, ce sont les. Selon les mots du Conseil d'État en 2019, un projet qui obligera à travailler plus longtemps avec une pension aléatoire en fonction d'une valeur de points fluctuante. C'est une gestion individualisée des retraites visant à opposer les professions entre elles. Nous n'en voulons port un jeu de points et cela a été largement démontré en 2019, où tous seront perdants, les femmes, la majorité des 20 millions de salariés du régime général, les professionnels libéraux. Les 400.000 agents des régimes spéciaux. Les quatre millions quatre de fonctionnaires, tous seront perdants. nous qui nous permettrait de bien vieilli au travail alors que nous voulons bien vieillir libéré du travail profiter de ce temps de la vie qui a pris un nom, celui de la retraite. Nous ne voulons pas de ce rapport, prémices d'une réforme qui au nom du marché. Remettre en cause le principe de solidarité qui fait la force de la protection sociale en France. Merci. Défendu. Et Madame Hustache Brugnaut pour le dernier amendement de suppression défendu. Donc nous en avons fini avec la présentation des. Amendements de suppression. Bon, la commission a donné son avis, puisqu'elle est partie prenante de ces amendements. Monsieur le Ministre. Merci beaucoup monsieur le président. Sachant compter voyant. Les signataires sur tous les bancs. Je je connais je pressens en tout cas à l'issue. En terme de d'espérance de vie pour cet article bis. Mais cette intervention permettra d'. Portée peut être de précision, d'abord pour dire à Madame la Présidente Rossignol. Le texte que le gouvernement a transmis au Sénat. Dans le cadre de l'application de l'article 47 syrien. Et le texte initial du gouvernement auquel nous avons ajouté la totalité. Ils étaient peu nombreux, la totalité des amendements adoptés par l'Assemblée nationale il y a eu aucun tri tous les amendements adoptés par la session de l'Assemblée nationale ont été ajoutées au texte que nous vous présentons. Vous dites pas suite. Suppression de l'article de mais l'article 45 tiens renvoie au projet initial du gouvernement accompagné les amendements adoptés par la Chambre qui l'a examiné et que le gouvernement souhaite conserver, nous avons conservé tous les amendements qui avait été adopté. La 2ème, précisons que que je voulais apporter avant de donner l'avis du gouvernement que vous présentez. C'est le fait que le système universel de retraite que nous avons présenté en 2019 n'était pas un système par capitalisation. Je tiens à le souligner. Je tiens aussi à souligner que le fait de faire un système à points n'implique pas automatiquement de mettre en place un système par capitalisation. Et j'ajoute d'ailleurs que dans les souvenirs que nous avons les uns et les autres du système universel de retraite proposé en 2019 une part considérable des cotisations acquérir à obtenir des points pour chacun des assurés, mais une part importante était consacrée au financement de mécanismes de solidarité qui se traduisait ensuite par l'octroi de points considéré comme gratuit mais qui n'avait rien de gratuit puisqu'il était financé par la par des cotisations consacrée aux mécanismes de solidarité et donc il n'y a pas d'antagonisme entre un système à points et un système par répartition et la loi de du projet de loi de 2019, malgré. Son devenir. Pouvez ainsi l'illustrer. Pour ce qui concerne les amendements de suppression. Je l'ai dit Monsieur le Président sachant compter, je vais faire court. Le gouvernement a donné un avis favorable à la demande de rapport qui avait été présenté par un certain nombre de députés de la majorité pour cette seule raison. Je ne peux donner un avis favorable à leur suppression mais voyant la liste des signataires je m'en remets au Sénat. Bien merci. Alors explications de vote, je signale que je suis saisi d'une demande de scrutin public. Par les groupes CRCE et les groupes socialistes. Donc nous allons. Passer aux explications de vote. Alors Madame Poncet. Mon jeu. Oui, merci Monsieur le Président, j'ai bien entendu me monsieur le 1er Ministre moi j'ai parlé de troisième étage qui sera un étage de capitalisation. J'ai jamais dit que les deux premiers ne pouvait pas l'Agirc, l'Arco, le montre bien, être dans un régime de pas de. de. Répartition oui. Alors. Moi je crois je voudrais revenir sur le fait effectivement que la grande différence quand même. Avec ses deux de de régime c'est que aujourd'hui dans toute la protection sociale. Nous avons alors souvent on dit c'est un salaire différé, moi je préfère dire que la protection sociale au nom du principe que je vous ai dit à chacun selon ses moyens et de et enfin de chacun et à chacun selon ses besoins, fait des prélèvements socialiser le prélèvement socialiser et le droit ça ouvre un droit qui est différée et dans toutes les branches, enfin pour ce qui est de la santé. Vomis. Pour ce qui est de la santé, vous voyez bien que on s'intéresse pas au rendement, on se dit pas. Ah j'ai cotisé autant, faudrait que je fasse un cancer pour. Pour avoir un retour sur investissement et c'est pareil pour tout hein. Et pour la retraite c'est pareil aujourd'hui nous payons pour les retraités. D'aujourd'hui et effectivement on ouvre un droit. Pour demain ce qui empêche pas de faire des réserves pour travailler à long terme, donc c'était un petit peu un petit peu ça que je je voulais pointer le fait que le 3ème étage lui qui sera effectivement très certainement. Par capitalisation futals collective puisqu'elle se verra comme supplément d'âme comme comme étage. Eh bien effectivement effectivement a besoin ma collègue a dit du premier étage qui lui quand même assure. Le respect de ce principe de socialisation. Dont j'ai parlé. Merci. La parole à Madame Lienemann. On a beaucoup débattu du système à points. Mais enfin, quelles que soient les formes qu'il prend. Le système à points des défauts structurels. Qui fragiliserait considérablement les Français. Effet redistributif quasi nul. Le point est incertain puisque son niveau peut changer et Madame prévu il a eu raison de rappeler ce que Monsieur Fillon. Dire ni vu ni connu, on change le point donc on baisse retraites. Et troisièmement, ça met tout le monde dans un système d'instabilité. Alors qu'on est déjà dans un système social ou tout ceux qui protègent garantit la sécurité permet de voir loin et totalement déstabilisé. Finalement déstabilisant l'ensemble du pacte républicain et de la société française. Mais je voudrais surtout insister. Sur l'incohérence. De la position gouvernementale. On nous dit dans un an. On va remettre sur le tapis. Les conditions n'a pas passage vers une retraite à points. Mais je ne demande pas simplement le retrait de de cet article. C'est bien le retrait de la réforme. Parce que si dans un an, il faut remettre tout sur le tapis. C'est pas la peine de continuer à mettre le pays à feu à 100. Réouvrir les négociations avec les organisations syndicales, prenez vos responsabilités pour qu'on ait enfin un débat politique avec les, les organisations syndicales de longue durée sur un système de retraite. Nous, nous avons nos propositions mais nous faites pas le coup de Jarnac. Dans un an. Pourquoi pas. Alors outre le fait que c'est incohérent. Ça ça donne cette ce sentiment dramatique d'instabilité chronique de nos systèmes de retraite qui le peuvent elles perdent toute confiance dans ce système et notre cohésion nationale. Alors non seulement retrait de cet article. Mais Monsieur le Ministre, soyez cohérent, retrait de la réforme. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, le gouvernement continue de nous tromper de tromper les Français. Après avoir fait le choix d'un véhicule législatif inadapté à l'examen d'une réforme aussi importante pour les Français un PLFR SS plutôt qu'un projet de loi en tant que telle. Le gouvernement sur le dire introduit par ce nouvel article la mise en oeuvre d'un système universel de retraite en proposant la remise d'un rapport système rejeté massivement par les Français. Rappelez-vous, alors oui il y a tromperie, quand vous nous dites qu'il faut cette réforme pour préserver notre système par répartition et insidieusement vous préparer le terrain pour demain. Alors Monsieur le Ministre, je vous le demande. Dites la vérité aux Français, ne les trompait pas nous les trompait pas en déclarant, c'est une réforme de gauche et en affirmant qu'il n'y aura pas de perdants. Dites, Monsieur le Ministre ce là ce qu'il en est et retirer cette réforme.

Qui est arrivée au Sénat. Et l'initiale du gouvernement parce qu'il n'a pas été au bout et vous l'avez dit, avec les articles ou amendements que nous souhaitions amendement que nous souhaitions conserver donc l'amendement de monsieur Ferracci adopté à l'Assemblée nationale. C'est bien un choix politique de le mettre parce que vous auriez pu ne pas le mettre et donc c'est un choix politique, il faut assumer. Monsieur le Ministre, de le conserver et que c'est ce texte avec cet amendement 1er bis que vous avez souhaité. Que nous échangeons entre nous et donc si c'est un choix politique assumé. Qui dit que d'ici un an. Il va falloir revenir vous souhaitez revenir devant le Parlement pour un nouveau débat des questions des retraites et là vous ouvrez l'amendement ouvre toutes les possibilités répartition comme aujourd'hui. Retraite par points. Vous avez raison. Qui est pas la même chose que capitalisation ou capitalisation individuelle ou collective, donc. Vous ouvrez toutes les possibilités y compris la capitalisation pour d'ici un an. Et donc là. Sincèrement, Monsieur le Ministre. Un projet de loi aussi mal fagoté dans les conditions dans lesquelles nous l'étudions et nous l'examinons. Avec une opposition féroce de l'ensemble des organisations syndicales et de la très grande majorité des Françaises et des Français. Franchement au point où nous en sommes. retrait de cette réforme, il n'y a que ça. Pour que nous puissions à nouveau. Avoir un débat serein que vous repreniez les négociations, comme l'a si bien dit ma collègue Marie-Noëlle Lienemann et que vous reveniez peut être avec une nouvelle proposition. La retraite par points qui était celle de 2019, donc on vous le redis il y a un agenda caché. vous ne voulez pas du système par répartition. Vous avez une autre ambition et cet amendement qui est retenue et en réalité votre véritable. Véritable ambition je vous remercie monsieur le président. Merci. Monsieur Jacques Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, vous n'avez vraiment pas convaincu par vos explications, j'interviens sur l'amendement de Madame Préville. Il y a véritablement un problème de cohérence et d'un DJ d'intelligibilité. Nous sommes dans un PLFSS avec un caractère d'urgence. Les Français ne peuvent rien y comprendre. un manque complet de cohérence quand vous revenez avec le régime de retraite à points du universelle qui a été rejetée massivement par les Français lors du premier quinquennat Macron. Et qui a obligé le président de la République et son gouvernement d'alors à abandonner son texte de surcroît le 10 janvier dernier. En présentant une nouvelle réforme des retraites. Cette fois-ci paramétrique, la Première ministre a signé le même l'arrêt de mort définitif de la retraite par points. Mais vous y revenez. Il y a donc pas lieu d'agiter le nouveau le spectre d'une future mise en oeuvre d'un système universel de retraite intégrant qui plus est, je cite les paramètres de la réforme prévue par la présente loi les Français ont clairement exprimé qu'ils ne veulent aucune des deux non seulement le gouvernement ne veut rien entendre et sans tête à ponctionner un impôt de 2 ans sur la vie des Français avec la retraite à 64 ans mais il leur dit en plus collier d'une réforme, ils vont en avoir deux. C'est de la provocation supprimons cet article. Supprimons la réforme est massif manifestons massivement ce mardi devant tant d'incohérences. Le rejet est considérable et la cohésion et l'adhésion seront dans la rue, je vous remercie. Merci Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en complément des éléments que j'ai déjà évoqué précédemment, je porte une explication de vote à l'. Demain 15, 47. Je souhaitais appuyé dans cette explication de vote l'impuissance du pouvoir politique qui traduirait que traduirait le maintien de cette demande de rapport il renvoie en effet à l'idée que cette réforme est inachevée incomplète et que le gouvernement doit une fois de plus revoir sa copie prochainement sur le sujet. Mais au vu de ce qu'a dit mes, mes collègues, je vois qu'on partage nombre cette inquiétude, ce constat, nous ne sommes pas en réalité seulement sur ces bancs le partager, puisque il me semble que le. C'est aussi le cas du Conseil d'État qui est très qui critique envers cette réforme mais ce n'est pas ainsi que vous communiquez depuis maintenant plusieurs mois sur ce projet de réforme mise en avant comme étant la bonne solution. D'une part pour sauvegarder le système de répartition. D'autre part pour renforcer son équité. Et voilà que l'on remettrait sur les rails la préparation d'un système universel de retraite se reposant sur les reculs sociaux déjà opéré par le présent texte puisqu'il est bien précisé que doivent être intégrées les paramètres de la réforme actuelle si vous souhaitiez réellement prendre davantage compte. En compte les spécificités inhérentes à chaque métier et à chaque parcours, alors il ne fallait pas supprimer les régimes spéciaux adaptés à la réalité des métiers qui les concerné. Il ne fallait pas encore pénaliser les femmes par cette réforme, il fallait rétablir les critères de pénibilité supprimés en 2017 par le gouvernement. Oui, la copie doit être revue. Mais alors allons jusqu'au bout de la cohérence et ne votons pas cette réforme. Merci monsieur le président. Je dois avouer que je suis très frustré parce que je ne peux pas demander l'avis du Conseil d'État. Sur cet amendement qui a été réintroduit par le gouvernement pour ce texte. Je voudrais. Re-insister sur un sujet parce qu'on en plaisante, on on passe du temps ensemble un dimanche après-midi. Mais ce texte. Qu'a-t-il à faire dans un projet de loi de finances rectificatif de la Sécurité sociale. n'a rien à y faire et donc on revient sans cesse. À chaque, outre le fait de l'autre l'incohérence de réouvrir ce débat qui monte qu'au fond vous-même savez que votre réforme n'est ni fait ni à faire, mais à chaque fois ça revient au fait que votre choix de ce projet de loi de finances rectificative de la Sécurité sociale est une ruse procédurière. Pour éviter d'avoir un débat de fond sur le travail et sur les retraites. Donc Monsieur le Ministre, je vous dis retirer la réforme évidemment nous ne voterons pas cet article 1er bis mais surtout retourner devant les partenaires sociaux parce qu'on ne peut pas imaginer une réforme des retraites sans que les partenaires sociaux y soient associés de façon réelle et continue, donc si vous voulez un an hé bien prenez cette année retirer la réforme et cette année de dialogue avec les partenaires sociaux, eux, ils sont toujours prêts à défendre les retraites des salariés. Merci. Madame Vogel. Merci monsieur le président. Pourquoi nous allons voté pour les amendements de suppression de de cet article. Il y a eu en 2019, la proposition d'une réforme des retraites pour instaurer un régime de retraites universel à cette époque, il y a eu la publication d'une étude d'impact. Sur un système de retraite universel. Cette réforme a été abandonnée. Nous avons maintenant quelque chose de tout à fait différent, qui est proposé dans la précipitation vient. Un véhicule législatif que nous considérons inopportun. Et on nous dit la majorité nous dit le gouvernement nous dit, dans cette même réforme que nous allons réfléchir à faire un rapport pour réfléchir à la réforme que nous avons abandonné il y a 2 ans. Alors il y a deux solutions. Soit vous avouer en réalité que le rapport que vous aviez eu l'étude d'impact. Que vous aviez lu j'espère. Publié en janvier 2020 était insincère. Incomplète. Hein. Satisfaisante et qu'elle permettait pas au fond de savoir si le système de retraite universel à points étaient bon ou pas ce que, à l'époque nous disions, soit vous reconnaissez que vous les avez ces informations j'imagine bien que si vous avez choisi cette réforme là c'était basés quand même sur des informations j'espère quand même que c'était basé sur. Des comparaisons entre les différents systèmes et à ce moment-là vous avouer qu'en réalité, le fait de cet article dans cette réforme, c'est bien pour nous préparer à l'étape suivante c'est bien pour nous dire que ceci n'est que la première étape à la mise en place d'un système qui a déjà été rejetée il y a quelques années. nous, nous pensons que si vous êtes toujours pas très clair ni avec vous même ni avec les Françaises et les Français. La solution la plus simple, puisqu'apparemment vous avez besoin d'un an pour savoir exactement ce que vous voulez faire ou en tout cas ce que vous voulez dire. Eh bien prenez cette année n'est pas pressé. Revenez l'année prochaine et puis nous verrons ce que nous ferons avec votre proposition finale.

il prévoit que dans un délai d'un an à compter de la promulgation de cette présente loi vous nous demandez de prévoir que le Gouvernement remette au Parlement un rapport sur un de les conditions trois le calendrier de mise en oeuvre d'un système universel de retraite faisant converger les différents régimes et intégrant les paramètres de réformes prévues par la paix présente loi alors le président de la République nous demande et demande aux Français de faire preuve de bon sens. Alors, le bon sens indique que si ce rapport est utile, il aurait dû être réalisé avant que vous nous présentiez les premiers éléments d'un nouveau système de retraite. Il est donc inutile. Retirer cette réforme est retiré. Donc cette demande de rapport. merci Monsieur le Président, chers chers collègues. Cet amendement est intéressant. En réalité, même si évidemment. Je vais m'y opposer avec, avec mes collègues. Il donne le sens.

et qui fait l'objet central de ce texte. Il y a la mise en oeuvre d'un régime à terme. Par capitalisation, ça j'en suis absolument certain et ce. À quoi je voudrais. ce que je voudrais aussi évoquer c'est c'est le climat dans lequel on est et dans lequel on est. Dans lequel sont les Français depuis 2019. Les Français, ça a été rappelé, on dit ce qu'il pensait de la de la réforme qu'qui leur qui leur été proposé en 2019, ils sont toujours sur la même ligne et là, avec cet amendement, en gros, on met le feu quoi on en rajoute, on en rajoute. Les les théoriciens du management de l'entreprise. Évoque un trotte technique le management par le chaos.

Je trouve qu'on est typiquement là dedans. Le management par le chaos. Voilà on prévoit que la population française et j'espère hein. Je suis un peu j'en suis certain. Elle saura nous dire mardi prochain et les jours à venir. Les semaines à venir les mois à venir qu'elle ne veut ni de la réforme qui nous est proposé en 1er lieu dans ce texte, ni de ce qui est annoncé par le biais de cet article à peu un rapport sur les régimes de capitalisation, même si on a tendance plutôt à les appeler les régimes. Systémique. Voilà donc je m'opposerai fermement à cet article qui en dit beaucoup sur l'état d'esprit. Au plus haut niveau de ce que. Notre président de la République veut faire de nos retraites et de la retraite des Français. Merci monsieur le comte.

même si nous ne comprenons pas pourquoi monsieur le Ministre. L'article 1 bis qui a été effectivement voté par l'Assemblée nationale reste dans votre projet présenté au Sénat alors que l'article 2 qui a été rejetée.

notre système et ça restera après la réforme et ce sera encore plus compliqué. Après la réforme, compte tenu des nouvelles exigences en terme de. De, de durée de cotisation et d'âge n'est pas adapté et de moins en moins adapté à des carrières hachées entre plusieurs dirigeants régimes de retraites différents. Je vous pose la question Monsieur le Ministre, êtes-vous prêt oui ou non à ouvrir des négociations avec les partenaires sociaux et avec les personnes concernées pour que les. Les les les les les personnes qui ont des carrières dans plusieurs régimes et qui sont aujourd'hui particulièrement en. Pénalisée par le calcul des des des des, du revenus des 2 des meilleures années de du revenu annuel moyen par l'imposition des 25 meilleures années. Qui bloque finalement le passage d'un système à l'autre et qui bloque les le calcul des retraites pour les personnes qui ont une carrière à l'international, est-ce que vous êtes prêt à bouger sur ce point. Merci monsieur Boyer. Merci monsieur le président. Je présume que dans cette assemblée. L'ensemble de nos collègues parlementaires, ont une culture politique. Très affirmée. Alors je cite. Allongement de la durée de cotisation. Sans réforme le système de retraites va droit dans le mur. Il faut demander aux Français de travailler plus longtemps et allonger la durée de cotisation. Qui a tenu ces propos. Je vous le répète parce que je crois qu'il n'avait pas très bien entendu. Allongement de la durée de cotisation. Sans réforme le système de retraites va droit dans le mur. Il faut travailler, il faut demander aux Français de travailler plus longtemps.

ans ça fait 10 ans que Madame Touraine a tenu ces propos. Et aujourd'hui apparemment à cette époque vous deviez trouver ses propos juste et responsable parce que il n'y a pas eu de mouvement de et donc. Aujourd'hui, on peut quand même dire que, à travers toutes les remarques, vous nous rabâché depuis 2 jours dans une démarche très politicienne est très démagogue. Je crois qu'il faut le dire, il y a un moment donné, il faut le dire lors cette proposition aujourd'hui qui est fait dans la loi que l'on discute. Elle prévoit d'accélérer. La mise en place de la réforme Touraine justement en 2027 plutôt qu'en 2035. Donc. Et et si on veut demain que pour nos enfants, nos petits-enfants. Nous puissions avoir un système de retraite ou il y aura certainement plus de retraités que d'actifs, il faut quand même que l'on ait des décisions à prendre. je voudrais aussi répété que dans. Et dire que dans cette assemblée, il n'y a pas les méchants sénateurs qui méprisent les Français ce que j'ai entendu ce matin et les bons sénateurs qui eux sont vertueux et qui ont le monopole du coeur, pour reprendre une citation d'un homme politique célèbre Auvergnat. Donc je pense qu'aujourd'hui on ne doit pas s'empêcher de réfléchir, ça a été dit ce matin et gouverner, c'est prévoir et c'est aussi anticiper. merci Monsieur le le président. Je tombe à pic. Juste après cette belle intervention. Vous présenter d'ailleurs. Cette réforme. qui eux qui allait qui va sauver notre régime de retraite. Ce qui est un peu inquiétant, c'est que logiquement si ça sauve le régime de retraite. Il aura pas besoin d'autre sinon c'est que ça ne sauve pas vraiment donc. Si on regarde vos stratégies en plus vous n'utilisez toujours qu'un seul paramètre de manière assez idéologique qui vous amène a reculé. Dans le futur finalement sans cesse l'âge légal de départ à la retraite là c'est 64 dans deux ans vous nous proposerez 66 après 68 70 et on n'arrêtera plus puisque vous souhaitez agir que sur le paramètre en plus le plus injuste, alors qu'il y en a plein d'autres. Ça fait deux jours qu'on vous les expose. Mais vous voulez rien entendre d'ailleurs ce qui est d'autant plus inquiétant et qui renforce cette impression c'est que vous prenez toujours par exemple tous ceux qui ont poussé le plus l'âge légal de départ à la retraite, c'est votre modèle vous dites regarder dans les autres pays font de 67. Mais avez-vous regardée dans ces pays, le taux de pauvreté chez les retraités pas, vous l'avez pas regardé. D'ailleurs il y a un bon exemple dans notre propre pays. Quand on est passé de 60 à 62 ans, ça a augmenté les allocataires au RSA. Parmi les personnes les plus âgées. Ça a augmenté le nombre de chômeurs et de chômeuses qui plus est avec la réforme que vous avez fait monsieur Dussopt, vous allez encore plus les précariser parce que leur droit au chômage va être rogné. Donc en fait si c'est ça votre modèle ben oui nous c'est pas le modèle que nous défendons. C'est pour ça que nous vous demandons à nouveau de retirer cette réforme injuste et brutale. Merci. Monsieur. Merci Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment de souffler un peu trop sur les braises. À un moment donné après les régimes spéciaux, qu'on a traité hier qui ont déjà mis la population en effervescence, elle ne l'était déjà pas beaucoup avec ce cavalier législatif, on peut dire que vous allez avoir un résultat immédiat. Ce que vous allez doubler voire tripler le nombre de manifestants. Pour la journée du mardi 7 mars qui joueront sans doute les prolongations sur le neuf et le 10 mars. Nous ne comprenons pas l'intérêt de cet article, dont vous connaissez maintenant. Le la destination et votre obstination à vouloir ne ne soutenir puisque. Nous sommes déjà. Dans une confusion totale sur ce que vous voulez véritablement en terme de régimes de retraite mais nous identifions de plus en plus la cible qui est la votre. Et c'est vrai que, à terme, la volonté de plus en plus explicite, c'est d'arriver à un régime de retraite par capitalisation. Et je vous dis de, d'ores et déjà. Telle que nous l'avons affirmé mais c'est sans doute une une image de façade. Nous sommes pour la retraite à répartition. Il n'est pas question de s'orienter vers de la retraite à capitalisation nous vous demandons instamment. De retirer cet article mais plus que cela de retirer votre réforme puisque elle n'est pas abouti. Elle n'est pas réfléchi et donc elle nécessite encore beaucoup beaucoup de temps de travail. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le gouvernement et les députés la République en marche, tente de faire revenir la réforme avortée de 2019 par une porte dérobée. Nous ne sommes pas dupes. Le régime de retraite à points dit universel a été massivement rejeté par les Français. Ils n'en veulent pas. Tout comme ils ne veulent pas du projet antisocial que vous présentez aujourd'hui dans cet hémicycle. Avec la présentation du texte que nous examinons. Madame, la Première ministre a pourtant signé l'arrêt de mort définitif de la retraite à points pourquoi dès lors, revenir à la charge avec cette demande de rapport. Pourquoi nier l'opposition des Français à ce qui est un texte inique. Votre mépris à l'égard de nos concitoyens vont jusqu'à envisager l'idée de l'Europe de leur imposer de réforme. Qu'ils ne veulent pas vous comptez Monsieur le Ministre, sur la lassitude le renoncement des Français empêchés par l'inflation, la perte de pouvoir d'achat. De se mobiliser les grèves et les manifestations historiques depuis le 19 janvier montre pourtant le contraire. Il n'oublie pas les Français, que vous avez refusé d'augmenter le SMIC. Il n'oublie pas que vous avez fragiliser l'assurance chômage. Ils savent que vous ne dites pas la vérité sur les retraites. Monsieur le Ministre. Écoutez la grande majorité d'actifs qui vous demandent le retrait de ce texte. Resté sourd leur mobilisation démocratique serait nourrir des lendemains de colère et de ressentiment. Ils ne se lasseront pas jusqu'à l'abandon de cette réforme, une réforme qui est rejeté. Et vous le savez par toutes les organisations syndicales. Merci. Merci monsieur le président. L'ancien président de la commission des affaires sociales du Sénat, homme d'expertise dans ce domaine a qualifié explicitement cet article de cavalier social. Monsieur le Ministre, la nostalgie vous accapare auprès de qualifier à votre tour votre proposition de loi de gauche alors que comme vous l'avez constaté la gauche de cet hémicycle refuse avec énergie et arguments fondés et précis qu'elle ne veut pas du texte. Et ne veut pas non plus de rapports, ni même de cet article. Monsieur le Ministre, écoutez les partenaires sociaux et sur tous les Français que nous représentons ici. Écoutez, ceux qui sont dans la rue et qui seront encore dans la rue le et surtout à ce qu'il faut veulent condamner Madame Touraine elle au moins elle n'a pas mis le pays à la rue en occultant les partenaires sociaux. Je vous remercie. Alors moi je vais refaire un petit peu d'histoire récente. Je l'ai déjà fait hier, mais c'est pour répondre. C'est pour répondre à mon collègue. La réforme Touraine à l'époque pas si lointaine, c'était 30 milliards d'euros de déficit annoncé à courte échéance la réforme Touraine. Elle a maintenu, François Hollande avait mis la retraite anticipée à 60 ans, quelques mois avant et la réforme Touraine elle a maintenu les 62 ans et les 62 ans pas nous qui les avions mis elle a maintenu les 62 ans alors d'aucun me disent oui mais ça sert à rien puisqu'il faut cotiser 43 ans et donc je répète que tout le monde ne fait pas des études supérieures, qu'il y a des gens qui commencent à travailler jeune. Et dans ce pays et qu'il y en aura toujours et que ces gens ont le droit de partir à la retraite à 60 ou à 62 ans, donc la réforme Touraine et ça n'était absolument pas la même chose, moi j'assume ce que je suis, j'assume ce que j'ai à un moment soutenu, je ne veux pas laisser dire n'importe quoi et en l'occurrence, vous avez dit n'importe quoi.

et pas très respectueux du Parlement sur le ministre dont vous avez parlé de la sagesse du Sénat. Moi je vous appelle la sagesse retirez retirez cet article et et c'est fini. Pourquoi. On ne va pas vous donner un an de plus et y compris sous l'impulsion de votre collègue quand même c'est monsieur Ferrat était rapporteur de la loi sur l'assurance chômage. C'est-à-dire qu'on discute de faire travailler les travailleurs et travailleuses 2 années de plus. Et on prend un article qui vient d'un député qui a rapporté sur la loi assurance-chômage qu'à moduler les conditions de l'accès de l'indemnisation quand on n'a pas de travail. Donc la question de cet amendement. C'est quoi. C'est les retraites mais c'est aussi le travail. D'une nouvelle précarité d'une nouvelle flexibilité d'une nouvelle chasse à des gens qui sont privés d'emploi. Donc franchement on va pas vous donner un an de plus pour ça et je vous le dis, il y a il y a une question de respect. Moi je pense, je vous le dis là sur tous les bancs, quelles que soient nos divergences et mais quand il y a l'unanimité ici pour retirer l'article la sagesse peut aussi être du côté du gouvernement, pas d'opération politicienne. Pas d'opération politicienne donc retirer cet article c'est pas il y a pas de honte à le faire. Voilà il fait l'unanimité contre donc retirer le et là on débat dans des bonnes conditions mon débat pas avec quasiment un fusil dans le dos en nous disant ça va être 64 ans ça va être 2 années de plus. Ça va des annuités en plus et. Attendez, d'ici un an, on va encore aggraver sur les mêmes conditions la réforme retirer le Monsieur le Ministre, ce sera votre honneur et celui de votre gouvernement. Madame briquet. C'est un prise de parole en soutien aux amendements de suppression de cet article, puisque le gouvernement souhaite. Passer par un rapport pour annoncer sa vraie réforme. un système universel, après une première tentative en 2019 alors que nous sommes censés discuter d'une réforme de la retraite par répartition, il pose les jalons pour le coup d'après et ce sans aucune garantie de concertations, de négociations de dialogue social avec les partenaires sociaux. Bien curieuse méthode que de dire aux Français que la réforme dont nous discutons aujourd'hui et qui conduit les Français dans la rue pour crier leur opposition. Hé bien. Que cette réforme n'est pas celle que l'on veut vraiment faire c'est vrai le pire n'est jamais certain. Et si le sort de cet article semble heureusement scellé. Monsieur le Ministre, vous pouvez faire mieux en retirant purement et simplement cette réforme injuste et inutile. Merci. Le président rénale. Merci. Monsieur le président. Ma. Je voudrais voir où on en est qu'on fasse un petit point de synthèse là. Dimanche là en début d'après-midi pour essayer de comprendre où en année. Et si on essaie. Faudra-t-il 40. Vous inquiétez pas je m'en occupe. Cette. Cette réforme des retraites nous avait été présenté où nous a été présenté, on s'en souvient avec. Combien de qualité sous le terme de la mère de toutes les réformes. pas, c'est pas rien. La mère de toutes les réformes. Elle devait elle avait cet objectif essentiel de rassurer nos jeunes sur le devenir. De la retraite par répartition. Alors après cette. Demi-journée, aujourd'hui on en est où. Hé bien on en est à avoir eu finalement de propositions. Complètement contraire à cet esprit. La première c'est de dire. Bon écoutez, on a fait ça mais ce qui est important c'est demain d'introduire je reprends vos Et là à l'instant, nous sommes sûrs. Plutôt revenir au projet de retraite à points. Alors moi je vous pose la question.

Et qui font que finalement ce que vous appelez tous la mère de toutes les réformes. Ce n'est jamais. Que le plus petit commun dénominateur entre les forces de droite de notre hémicycle. Oui, merci Monsieur le Président. Je. En écoutant l'ensemble de nos collègues, je me pose de questions. Je devais être un petit peu naïf probablement et je me demande pourquoi quand on présente un amendement. On a besoin ensuite de revenir pour se convaincre que cet amendement est bon et demandé à ses collègues de le voter. Première question. 2ème question. C'est c'est c'est une aurez le droit. J'espère bien, j'espère bien. 2ème question si c'est pas ça. La réponse à ma question c'est que vous considérez que les adversaires, enfin ceux qui sont en face de vous et qui pense pour une fois la même chose que vous n'ont pas compris ce que vous nous disiez et c'est extrêmement désobligeants pour nous. Voilà c'est ce que je voulais dire Monsieur le Président. Donc maintenant j'aimerais qu'on passe au vote parce que je pense qu'il y a urgence.

sur ces amendements de. De suppression. Je vous rappelle que je suis saisi d'une demande de scrutin public par les groupes CRCE. Et socialiste avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du gouvernement il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin. Est ouvert.

Le scrutin est clos. Oui. On votants 343 exprimés, 293 pour 292 contre 1, le Sénat a adopté les amendements de suppression.

Il nous reste un amendement après l'article 1er bis. C'est monsieur mouillé qui le présente. L'amendement 31 08. Attends Monsieur le président, Monsieur le Ministre c'était moment et tu aurais été une demande de rapport mais il a surtout vocation à donner le de donner l'occasion au ministre de réagir sur une situation anormale. En effet la l'article 14 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique prévoit la prise en compte des allocations d'enseignement dans la Constitution et la liquidation du droit à la pension de retraite des enseignants. Ces allocations ne sont toutefois à l'heure actuelle pas comptabilisées pour les droits assez retraites alors que les parce que les décrets d'application prévus ne sont jamais non jamais Or l'obligation de prendre une rayure réglementaires d'application de la loi est une compétence du gouvernement et l'administration est tenue de prendre dans un délai raisonnable, on dit bien raisonnable. Les dispositions réglementaires, étant donné le débat et étant donné la situation que nous évoquons aujourd'hui nous souhaitons entendre Monsieur sur ce point important et donc l'occasion de porter cet amendement sur le rapport vous donnera ses ministres à l'occasion de nous donner votre position. Merci madame la rapporteure. Oui, la commission demande l'avis du gouvernement pour régler cette vieille affaire. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur. Monsieur le Sénateur, pardonnez-moi mais pour. À dire vrai. J'ai découvert une partie de cette problématique. Il y a, il n'y a pas si longtemps, comme vous pouvez le constater au que j'ai à la main et et c'est ce qui fait un peu de confusion dans mon esprit. Non plus sérieusement, vous, votre amendement renvoie un engagement politique des années 80, époque où il y avait un déficit d'attractivité du métier d'enseignant ce qui. Démontre qu'il est bien souvent. Notre tâche est un peu celle de Sisyphe. Il s'est traduit par la création par décret d'allocation d'enseignement à destination des candidats se décidant concours d'enseignement notamment préparant ses concours suivant la première année de formation à l'IUFM et cet engagement a été prolongé par la loi en matière de droits à pension avec l'article 14 de la loi du 26 juillet 91 que vous mentionnez et qui prévoit que ces périodes de perception à l'occasion d'enseignement créé par le décret de 89 ainsi que la première année passée en IUFM en qualité d'allocataires seraient prises en compte dans des conditions fixées par décret pour la constitution la liquidation des pensions. Cet engagement des années 80. 80, c'est en réalité dilué au fil des ans cela aboutit un cadre juridique incomplet, puisque le décret prévu par la loi de 91 n'a tout simplement jamais été prise en compte et jamais été publié. Je vous rejoins sur le fait que ça n'est pas satisfaisant. Je vous invite plutôt au retrait d'amendements pour une raison en particulier, c'est que la loi de 1991 est toujours en vigueur. Et votre amendement propose de supprimer la mention fixé par décret. Si nous suivions votre raisonnement. Le gouvernement ne pourrait plus prendre de décret et ne pourrait pas apporter de corrections la correction que nous pouvons apporter passe par un décret. Mais ce décret soeur tu as une difficulté très matérielles très concrètes qui fait que. Les étudiants inscrits. En préparation mon première année d'IUFM pendant la période couverte par la loi de 1991 sont en réalité des enseignants qui aujourd'hui pour la plupart d'entre eux sont soit en retraite soit dans une situation, il demande à liquider leurs droits à la retraite, donc il faut qu'on trouve quelque chose et et un moyen pour le le valoriser. Je ne sais pas le dire à l'instant où je vous parle ce c'est un chantier que nous avons découvert avec la réforme pour dire la la réalité des choses que nous devons ouvrir mais pour l'ouvrir. Il nous faut un véhicule législatif permettant de prendre le décret d'où la demande de retrait.

Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En effet depuis 1991 certains agents titulaires de l'Éducation nationale sont pénalisés lors de la. Leur dossier de retraite par l'absence de de publication de ce décret et certains d'entre eux découvrent. Que leur première année à l'IUFM en tant qu'allocataire ne peut être validé pour la liquidation de leur droit à pension. Alors Monsieur le Ministre, vous indiquez que vous Découvrez ce problème à l'occasion de cette réforme.

Question écrite à laquelle il avait répondu en 2021 vous voyez 2017 2021. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'un examen interministériel du dispositif avec le ministère chargé des Comptes publics, de la fonction publique et le secrétariat d'État chargé des retraites était engagée afin d'identifier les évolutions à apporter de la tête de, de nature législative ou réglementaire pour répondre à cette situation donc visiblement quand même le dossier s'est perdu puisque le gouvernement le connaissais depuis. Plusieurs années suite à la saisine de parlementaires et je m'étonne que rien n'a été fait. Rien ne s'est passé. Donc c'est pour cela que nous soutenons cet amendement pour réparer cette injustice. Oui, monsieur le président, j'aurais dû intervenir plus tôt m'été je vais retirer l'amendement regarde la présentation du du ministre en sachant que. Nous au souhaitons être associée en tous les cas à la recherche de solutions. Le message est entendu. C'était une demande de rapport hein simplement. Et donc je retire l'amendement.

Donc l'amendement et et repris par Madame bla Trix compta. Madame Monnier, vous demandez la parole. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Oui, c'est un beau geste de Madame Florence Béatrix compta. Nous avions avec elle et Jacques Bernard Magner demander des rapports respectivement sous trois et six mois sur les modalités pour faire. Aboutir cette 10. Pour l'État Madame Monnier, nous allons l'écouter dans le calme et la sérénité. Allez-y. Merci. Dans ce que nous avions déposé comme amendement avec Jacques Bernard Magner Florence que ça avait été jugée recevable. Donc je trouve très bien qu'on puisse en débattre. C'est un sujet important, j'espère qu'on trouvera malgré tout, malgré ce qui vient d'être dit. Les explications données par Monsieur le ministre, il faut que nous trouvions un consensus sur ce sujet parce que c'est vraiment une aberration. Il est plus que temps de le corriger en droit d'ailleurs s'interroger plus globalement sur le temps de publication de. Décrit quand il ne tombe pas tout bonnement aux oubliettes par ailleurs. Imaginez le signal de bienvenue que ce sera qui sera envoyé à l'ensemble des enseignantes et des enseignants concernant cette disposition. J'espère qu'il ne sera pas le seul même si bien sûr il serait encore préférable de ne pas les obliger à partir à la retraite plus tardivement.

Madame Rossignol au moment madame ce on a a dit qu'elle reprenait l'amendement que je vois que le ministre qui n'a jamais été sénateur mais qui connaît certainement mieux règlement de l'Assemblée nationale que celui du Sénat, est aussi un peu perplexe. C'était un hommage aux députés qu'il a été franchement pour une fois que j'essaie d'être gentil, vous pourriez être soutenant.

après que sa discussion à commencer peut être immédiatement repris par un sénateur qui ne n'était pas signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue donc madame Béatrice compta reprend l'amendement en vertu de cet article du règlement du Sénat. Actuellement. Donc je donne la parole à Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président, mais Madame Madame Rossignol je je ne connais pas le règlement du Sénat comme vous mais je n'ai aucun doute sur le droit des parlementaires à reprendre un amendement pour avoir siégé à l'Assemblée depuis 2007. Il m'est arrivé d'en reprendre. Ce qui me surprend. C'est que j'entends des expressions de votre groupe que vous souhaitez comme les auteurs de l'amendement qu'une solution soit trouvée pour permettre la valorisation des trimestres passés à l'IUFM par les enseignants. Or. Si l'objectif de madame la sénatrice de l'Afrique à et que cet amendement soit adopté. Et si cet amant et si cet amendement est adopté. Je vous indique à en lire le corps de l'amendement qui dit qu'il s'agit d'insérer un article additionnel. l'article 14 de la loi de 1991. Sont supprimés les mots et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, ce qui signifie, madame la sénatrice, que si le Sénat vous suit dans la reprise de l'amendement et adopte cet amendement vous priver le gouvernement de toute possibilité de prendre de décret et donc d'apporter une solution. Madame. Contrat. Monsieur le Ministre, je souhaitais que la discussion soit poursuivi parce que vous avez été alertés par les parlementaires. monsieur Blanquer avait répondu après 4 ans après, la question de la parlementaire que quelque chose se fait vous nous indiquait que vous Découvrez le problème. Il y a quand même une vraie question. Donc j'espère que cela vaut pour engagement d'avancer sur ce sujet que votre parole vos engagements d'avancer sur le sujet, je le retire, je vous remercie. vous plaît. Nous allons franchir une étape significative puisque nous entamons la discussion de l'article de. Alors je vais tout de suite donner la parole. Au rapporteur. Monsieur Savary qui veut prendre la parole d'emblée toute de suite. Vous souhaitez maintenant ou à ou à ou après la discussion de la motion.

avant la motion comme vous le souhaitez, monsieur le président. C'est vous qui êtes maître. Ce que vous m'avez indiqué que vous souhaitiez la prendre avant. Mais si cet après on fait tout de suite la motion de renvoi et ensuite je vous donne la parole. Pas de problème. Alors on fait d'abord la motion de renvoi. D'accord. Madame Émilienne pou Myrhol et les membres du groupe socialiste, écologiste et républicain ont déposé une motion tendant au renvoi à la Commission de l'article de cette motion porte le numéro 47 40. La parole est donc à Madame Émilienne rôle. Pour la motion. Monsieur le Ministre, chers collègues. plus de 12 ans, de 55 ans, cet article introduit un indicateur, relatif à l'emploi des salariés âgés, pour les entreprises de plus de 300 salariés, l'index senior. Cette réforme des retraites voulue par le gouvernement et donc bien non seulement une réforme budgétaire, mais bien aussi une réforme du marché du travail qui ne dit pas sur le nom, la création d'un index seniors en est un exemple. Et si nous obtenions. La fameuse note du Conseil d'État dont nous parlons depuis deux jours, peut être il dit rien ne nous évoqué le risque d'inconstitutionnalité de cet article de. L'index senior n'a en effet aucune incidence financière et n'a donc rien à faire dans un Plfss SS rectificatif. Alors oui. La situation des seniors sur le marché du travail en France n'est pas bonne. Cela veille d'ailleurs été pointé dans un rapport de nos collègues René-Paul Savary et Monique Lubin en 2019. Selon la Darès 56% seulement des seniors dans l'emploi contre 65 pour 160,5%. Anne Europe et les chiffres du ministère du Travail parle de 53 8 %. Contre 70% en Allemagne ou en Suède. Par ailleurs, nous savons que le recul de l'âge de départ de 60 à 62 ans de la réforme. Woerth en 2010 a provoqué 100.000 chômeurs de plus combien. Pour le passage de 62 à 64 ans, 90.000 selon la Darès 300.000 selon l'OFCE et l'Unédic. Dans un rapport récent du 1er mars 2023. Viennent de confirmer que l'approche de l'âge de légal de la retraite entraînent un pic de rupture conventionnelle. Monsieur le Ministre, avez-vous évalué le coût de ces données supplémentaires par ailleurs nos collègues LR ont déposé des propositions sur l'emploi des seniors et donc nous avons besoin d'étudier en profondeur ce dossier en commission. On ne peut pas régler par un simple article rectificatif du PLFSS, sans qu'il y ait un débat de fond au sein de la Haute Assemblée. Le président de temps donc cette motion de renvoi en commission que nous vous demandons d'adopter.

Elle ne s'est pas réuni sur cette motion spécifique qui vient de tomber, mais on a donné déjà 2 fois des avis défavorables sur des renvoi en commission d'abord, il y a eu une motion d'irrecevabilité que nous avons rejeté. On est un peu dans la même veine et dans le même esprit. Donc voilà pourquoi je donne un avis contre et puis je voulais aussi préciser que. Le renvoi en commission. Moi je veux bien, mais lorsqu'on a fait la commission mardi dernier, on a passé 2h en commission. et il y a eu très peu de prise de parole, mais ce que je ne vous reproche pas nous disant on se réserve pour le débat. Alors si on se réserve pour le débat et on a vu en effet que vous réserviez pour le départ, ça c'est indéniable, on l'a bien remarqué, je ne vois pas l'intérêt d'un renvoi en commission. C'est donc un avis défavorable. Merci monsieur le ministre. Même avis. Même avis pour le gouvernement, donc il y a la possibilité d'une explication de vote par groupe à ce que certains souhaitent. Madame Poncet Monge. Allez-y. Oui, merci Monsieur le Président. Donc pour mon groupe. Moi je vais, je vais soutenir cette demande de renvoi et pour une raison bien précise Parce que je souhaite qu'on rediscute des amendements que la commission a jugé irrecevable sur l'index des seniors. Alors qu'on est en plein paradoxe parce que le gouvernement laisse l'index là tout en 2, tenant compte, lui qui a pris connaissance de la vie, je dis bien de l'avis du Conseil d'État qui risquent d'être supprimés donc il le maintient. C'est normal parce que. C'est censé atténuer non pas atténué mais là. Avoir une obligation de petite demande une petite contrainte envers les employeurs alors il aimerait bien. Laisser cette illusion qui demande quelque chose aux employeurs. Pourquoi pas, mais moi ce que je, je vois c'est que beaucoup d'amendements ayant trait à l'index, ont été non pas refuser ce c'est, c'était des demandes de rapport sous prétexte que c'était l'article 40 tout ça mais quand même indirectement parce que il semblerait que c'est pas de lien Direct ou indirect. J'ai bien compris. Avec la réforme. Donc il faut savoir si l'index est maintenu pour donner se semblant. De demander quelque chose aux employeurs. Et on en reparlera ou s'il n'a pas lieu d'être là et que des on va le discuter. Alors que le conseil constitutionnel risque de le le retirer. Dans ce cas-là, il faut peut-être revisité. Le la décision sur plusieurs amendements. Demandant des rapports la décision donc de les juger irrecevables comme étant, paraît-il, sans lien immédiat Direct ou indirect, avec la réforme. Merci madame Lubin. Rien de surprenant à ce que je vous dise, et qu'effectivement nous soutenons cette demande de renvoi en commission, puisque c'est la nôtre. Mais parce que nous estimons. Bon alors on aura l'occasion, on a beaucoup de choses à dire hein sur cet index des seniors et sur la forme et sur le fond, mais nous estimons effectivement que cette. Réforme des retraites ne prend absolument pas en compte la situation des seniors, qu'elle n'a. Que nous n'avons aucune étude chiffrée qui nous permet, à part quelques approximations de temps en temps qui nous permet de savoir quelle sera la situation des seniors après ces ces 2 années supplémentaires. De de de travail du chômage pour certains. Enfin bref. Donc nous, nous considérons que même si nous avons eu une réunion de commission effectivement mais à la limite ça n'est, ça n'est presque pas ça que nous remettons en question, c'est les éléments dans la commission aurait pu bénéficier pour travailler. Nous estimons que nous que nous en avait n'en avons pas eu suffisamment dans ce projet de réforme des retraites et puis bon même en arrêtant de gamberger sur cette fameuse note. Dont nous aimerions en avoir connaissance. Il nous en a été parler à l'Assemblée nationale. Nous savons à peu près ce qu'il y a dedans. Et nous savons que ce cet article de va certainement être. Effectivement, était un cavalier législatif et donc nous allons-y passer beaucoup de temps dessus. Pourquoi au final et peut être juste pour le vote d'un projet de loi qui abîmeras considérablement la situation des seniors. Merci monsieur Savoldelli.

Le gouvernement met en place un index pour les entreprises de plus de 300 salariés, avec pour seule obligation. J'irai dire l'unique obligation c'est la publication de ce dernier. Et une sanction pouvant aller jusqu'à 1% de la masse salariale, le cas échéant. Il faut savoir que cette rédaction là je l'ai retrouvé texto. Dans les affirmations et les volontés, ça va étonner personne du hop des grandes entreprises et pour pas le nommer, c'est le MEDEF. Donc sans contrainte cet index n'aura aucun pouvoir de contrainte, alors que les trajectoires entre l'emploi et la retraite ne sont pas linéaires tout le monde le sait ici. En effet, nous ne pouvons ignorer qu'à 60 ans près d'une personne sur 3 n'est ni en emploi, ni en retraite. Et que la majorité d'entre elles sont en situation. Des fois malheureusement d'invalidité. De RSA ou le chômage les tous dans une grande précarité, ainsi nous dénonçons cet allongement du ce qu'on peut appeler le sas de précarité des seniors qui aura des conséquences désastreuses pour trop de personnes et puis je voudrais faire aussi hein. Un petit. Revenir un petit peu en arrière, j'espère que ça nous rassemblera unanimement ici. Parce que l'expérience, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. C'est qu'à l'instar il y a eu un index égalité. Hommes-Femmes, rappelez-vous il a été créé en 2018. Et ben cet index, il n'a pas favorisé l'application de la loi sur l'égalité salariale. Donc on a aussi l'expérience pour nous. Et si on pouvait l'avoir communément. Ça serait bien d'avoir cette expérience pour nous un index. Ne fait pas les changements que la société doit opérer donc ça a été vrai pour l'égalité salariale hommes-femmes. Il faut que ça soit pareil pour les seniors. C'est pour ça tout le bon sens de cette de cette renvoie en en bleu. La motion en commission, et puis tout le travail d'amendement de l'ensemble des parlementaires que nous sommes. Merci. Merci. Il n'y a pas d'autres groupes qui ont demandé la parole. Donc nous allons passer au vote sur cette motion de renvoi. Donc qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Elle n'est pas adopté. Donc nous allons attaquer la la discussion et les paroles sur article à propos de l'article de et. Donc je vais d'abord donner la parole à monsieur le rapporteur.

En plus. Et tant mieux fait que nous vivons plus longtemps, il nous faut revoir sur le plan sociétal. La prise en compte des seniors et. On a une tranche de vie, une tranche de vie intermédiaire sur laquelle jusqu'à présent nous n'avons pas légiférer entre la fin d'une carrière active et le début d'une sédentarité et cette sédentarité dure de plus en plus longtemps, donc il faut la préparer. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours dit qu'il manquait un un volet de prise en compte. De l'employabilité des seniors et qu'il ait été plus judicieux de prendre en compte. Cette tranche de vie avant de passer à un projet définitif de retraite, c'est ce qui nous a animés. À travers nos réflexions pour vous faire des propositions d'ailleurs ça a déjà été pris en compte par des gouvernements précédents puisque nous sommes face à une augmentation de la durée nécessaire de cotisations, 43 ans, qui a été votée il y a quelques années sous le gouvernement Hollande et qui fait que on est amené effectivement à travailler beaucoup plus longtemps, donc il faut prendre en compte ce qu'ils peuvent être usés à travers cette longévité que l'on admet bien volontiers. Dans l'emploi. C'est la raison pour laquelle il nous a semblé important de bâtir des à présent bien que ce soit une loi retraites une politique vis-à-vis de l'emploi des seniors qu'on pourrait appeler Monsieur le Ministre. Un senior, une solution. Il y avait le plan un jeune, une solution qui a a manqué marquer une ambition justement de faire en sorte qu'il y ait une une dimension collective pour la prise en compte des emplois des jeunes, et bien là. Nous souhaitons une dimension collective pour la prise en compte des seniors 3 volé il y a les seniors qui sont au chômage, les seniors qui sont en emploi et puis ceux qui voudraient hein un peu une période de transition transitoire en ce qui concerne les seniors au chômage. Nous proposons un nouveau CDI, le CDI seniors, nous aurons l'occasion d'un article à un article suivant d'en parler. En ce qui concerne les seniors en emploi. Nous proposons des dispositifs qui permettent à la fois d'être plus généreux sur les pensions notamment pour ses des mères de famille dont vous nous avez dit toutes les difficultés rencontrées autour de leur carrière. C'est la raison pour laquelle nous proposons une surcote et nous proposons aussi d'autres dispositifs. La retraite progressive des 60 ans et puis également que le temps partiel dans le cadre du c'est de paix qui donne cette possibilité nous le réserve pour la fin de carrière de façon à aménager, prendre en compte les difficultés des seniors du côté des employeurs, il y a aussi une certaine attractivité, hé bien nous avons. Développé les positions de mutualisation de la prise en compte sur les cotisations. AT-MP pour que ce soit pas le dernier employeur qui paye la note pour l'usure de notre salarié qui aurait que connu différentes. Différents emplois et d'autre part nous avons pensé qu'il fallait dissuader cette rupture. Conventionnelle de deux 3 ans avant le départ à la retraite est un consensus social où tout le monde s'y retrouve ma foi le salarié, on lui dis vois. Peut y avoir. Une fin de carrière en en passant par la case chômage avant la retraite et puis. L'employeur qui y voit effectivement quelques indemnités sans qu'il y ait une taxation suffisante, donc nous avons souhaité augmenter la taxation 30% de la rupture conventionnelle ça une réflexion d'ailleurs qui qui venait de l'Assemblée nationale qui nous a. Qui nous a paru pertinentes. Voilà un petit peu le dispositif qui va être décliné lors des différents articles. En ce qui concerne l'index aussi Niort.

à un certain moment. Ça veut dire que. Une entreprise qui a beaucoup de seniors, c'est pas pour autant qu'elle aime les seniors c'est parce que, au fil du temps il en état si elle a des seniors, elle aura un très bon index puis quand il s'agira de remplacer ces personnes on va embaucher des jeunes, l'index va se dégrader à contrario, une entreprise qui a beaucoup de jeunes parce que c'est une entreprise de technologie de biotechnologie, madame la présidente, hé bien ces entreprises là elles ont que des jeunes pourquoi parce que les compétences. Ne sont pas retrouvé forcément à travers des seniors sont plus volontiers des compétences. Plus récente et qu'il n'y a que des jeunes qui les possèdent donc elle va avoir un mauvais index seniors néanmoins, néanmoins, nous avons convenu que il fallait effectivement lancé ce plan senior et convaincre les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de reprendre ce des dispositifs. Index senior mais en le mettant à 300 salariés et non pas des 50 salariés. Pourquoi, parce que 300 salariés. C'est le seuil où il y a ces discussions au niveau de l'entreprise pour la gestion prévisionnelle des emplois et c'est là que l'on peut définir une politique des seniors et faire en sorte qu'elle soit clairement. Décliné pour être éventuellement. Dans le quatre des index, voilà ce qui nous a animé dans notre réflexion et que je souhaitais vous présenter. le reste des amendements sur cet article de donc les paroles sur article et je passe tout de suite la parole à Madame. Cathy ah pour. Merci monsieur le président. Nous n'avons pas proposé de supprimer cet article bien évidemment que l'index des seniors telle qui nous est proposé est à l'heure c'est une facétie du gouvernement pour faire croire que vous parlez du travail et du ciel des seniors. Nous aurions voté plutôt contre 2 fois qu'une. Mais voyez-vous, nous avions l'espoir d'en faire un outil réellement contraignant au service de l'emploi des seniors. Nous proposions une réécriture intégrale de cet article. Cet amendement est irrecevable. Écoutez le motif c'est assez drôle. Cet amendement qui concerne le droit du travail et l'emploi des seniors et ne prévoit pas d'affectation de la pénibilité à la sécurité sociale n'a pas d'effet sur les recettes des régimes obligatoires de base de la sécurité pour 2023. Il est donc irrecevable en application de l'article L O 111 tirer 3 tirer 12 du code de la sécurité sociale. Donc nous crayons. une pénible une pénalité financière de 10% des rémunérations et gain pour les entreprises de plus de 5000 salariés qui ne respectent pas les critères de l'index que nous fixons.

dont l'impact budgétaire. Je veux vous dire que c'était autre chose que la maigre sanctions facultative si enfin peut être les entreprises ne daigne même pas publié le fameux index senior et ça aurait été une incidence financière si ces mêmes entreprises ne le respecte pas c'est le régime 0 sanction. Il est impératif d'en faire un outil au service des entreprises incitatif. Nous reviendrons sur le dévoiement du sens de ce terme dans le débat public. Pardonnez-moi, mais le Conseil d'État. Non. Dont nous attendons toujours la note qui vous a été transmise Monsieur Savary et que vous allez vous faire un plaisir de nous remettre disait l'index senior était un cavalier social quand car sans incidence budgétaire. Merci madame pour. La parole est à notre collègue Monique Lubin. l'd'un index d'emploi des seniors. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet. Il faut parler de la forme, mais il faut parler du fond. Sur la forme. Sur la forme. Le gouvernement sait pertinemment que dans une loi de finances de la Sécurité sociale rectificative. On ne peut pas parler d'autre chose que de mesures budgétaires et donc on ne peut pas. Valablement discuter de la situation des seniors et surtout mettre en place de véritables mesures en faveur des seniors.

Sur le fond, le gouvernement ignore-t-il la situation des 10 seniors. Alors on va en discuter, on aura le temps hein. Seniors, c'est à quel âge, 50 ans, 55 ans pour certaines entreprises c'est même 45 ans mais allez on va dire que la situation est critique. À partir de 55 ans. Est très tendue à partir de 50 ans, le gouvernement ignore-t-il cela. Le gouvernement s'est-il que de très nombreux Bruce senior après 55 ans ne retrouve pas d'emploi et se retrouve après une vie de labeur dans la spirale du chômage des fins des fins de droits des minima sociaux et attends la retraite avec impatience pour pouvoir enfin avoir une. En. Revenu qui leur assure un minimum de dignité et ça n'est certainement pas à travers de ce projet de loi que les choses vont s'améliorer. Alors nous, nous proposerons la suppression non pas je vais terminer Monsieur le Président que nous n'ayons pas confiance au rapporteur parce que je le dis, je connais la volonté du rapporteur de traiter ces sujets-là et son attachement à ce sujet-là mais nous ne pouvons pas cautionner ce que le gouvernement nous propose. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Pour ma part je considère que l'index et aussi utile qu'un numéro Vert pour lutter contre la canicule l'été dernier. C'est-à-dire nulle et non avenue. D'ailleurs. Cet index. Il l'a redit, mon collègue Pascal Savoldelli il sera pas contraignant. On ne sait pas ce qu'il y aura parce qu'il y aura par décret seulement peut être le nombre de seniors dans l'entreprise et sur les questions de formation même l'index. D'égalité salariale femmes-hommes qui est déjà pas assez contraignant. Il. Propose. Qui est quand même une sanction si des mesures correctives ne sont pas faits là, vous allez même pas vers la. Seules les entreprises. Qui ne l'auront pas publié se verront. Infliger une amende qui sera évidemment extrêmement faible. Moi je pense qu'on devrait se poser de questions,

et les entreprises au-delà de 55 ans les pousse dehors donc quelles mesures concrètes, vous nous proposez pour conserver des seniors. Au travail, il va falloir bien qu'on débatte de ça parce que c'est pas l'index qui poussera les entreprises à les conserver, puis la 2ème, c'est un chiffre, c'est l'adresse qui nous le donne. 1,4 millions de personnes. Âgées de 53 69 ans ne perçoivent ni pension de retraite ni revenus d'activité. Oui c'est dans L'Humanité spécial. Retraites. Très bon numéro d'ailleurs si vous l'avez pas, vous pouvez le prendre. La. Et là, le recul de 62 à 64 ans. N'agira pas sur ces 1,4 millions ces personnes-là continueront à être sans ressources et sans emploi. Donc qu'est-ce que, concrètement, vous allez faire sur ces questions là, je vous remercie. Merci monsieur. La parole à la présidente, Éliane Assassi. Oui, merci monsieur le président, mes chers collègues. Monsieur lors de la discussion générale vous avez affirmé que cette réforme allez mécaniquement augmenter le taux d'emploi des personnes en fin de carrière. Alors pourtant France Stratégie et j'ai les les documents ici France Stratégie nous rappelle que je cite l'effet des règles du système de retraites, sur l'emploi des seniors est loin d'être mécanique même des règles coercitives telles que le relèvement de l'âge d'ouverture des droits sur se heurte à l'hétérogénéité des situations de fin de carrière, L'index senior ne permettra pas et nous le savons tous de remédier aux représentations négatives qui sont liées à l'âge, l'âge constitue. Je dirais. Avec le sexe avec les. Origines des individus parmi les premiers motifs déclaré. Des expériences de discrimination Les au travail. L'autre fait que vous veniez c'est quand même assez important, c'est l'état de santé. Toujours selon France Stratégie. Plus de la moitié des personnes prématurément sorties de la, de l'emploi on impute leur décision à des problèmes de santé. Un chiffre à prendre je crois très au sérieux, dans un contexte de quasi-stagnation de l'espérance de vie sans incapacité à 50 ans depuis le début des années 2000. Concrètement, la taxe seniors ne remettra pas en cause des pratiques délétères par exemple ce qu'on appelle le harcèlement moral démissionnaire qui consiste à dégrader les conditions de travail d'un salarié pour provoquer son départ à moindre coût. La mise au placard dans les entreprises, concernerait 200.000 salariés coûterait, écoutez-moi bien, 10 milliards d'euros par an. Bref, vous avez la prétention je vous aussi de poser les bases d'une nouvelle société du travail. y a 2 mois mais je crois que c'est surtout une société du travail qui ressemblent plus à un grand retour en arrière, plus qu'à une véritable nouveauté. Merci. Notre collègue maintenant Laurence Cohen. Oui, merci Monsieur le Président, confirmant largement les éléments qui sont fournis par le démographe Hervé Lebras avec la survenue de la période Covid. L'espérance de vie dans notre pays aurait tendance à stagner, voire à décliner. C'est ce que nous indique le bilan démographique 2023 récemment publié par les services de l'Insee en 2022, 667.000 personnes sont décédées en France soit 5000 de plus qu'en 2021. Ce nombre élevé de décès dus au vieillissement de la population mais aussi à leurs conditions de vie et de travail. Le changement climatique. Il est aussi pour quelque chose avec des périodes de canicule qui comme chacun et chacune le sait ont une incidence et des conséquences sur les corps des travailleurs âgés. Seule une retraite anticipée pour toutes et tous, serait une solution. On est en 2023, mes chers collègues, on pourrait s'appuyer sur les formidables progrès technologiques, informatiques et donc travailler beaucoup moins longtemps. D'où l'absurdité de votre réforme allonger la vie active, sans prendre en compte les conditions effectives de l'emploi est source de beaucoup beaucoup de souffrance et de peu d'efficacité économique puisque vous faites primer l'équilibre comptable et financier est fallacieux pour justifier votre réforme, et non le bien-être de chacune et chacun. Vous faites fausse route. La Cour des comptes souligne une croissance notable des dépenses pour le risque maladie dans les années qui ont suivi le passage de 60 à 62 ans, le coût des indemnités journalières liées à l'absence pour maladie a augmenté en moyenne chaque année de 4,2. Enjeux financiers pour les organismes publics, mais aussi pour les entreprises qui doivent pallier les absences plus fréquentes de salariés. Alors évidemment pour faire passer la pilule, si j'ose m'exprimer de manière familière vous sortez cet index et comme mes collègues l'ont dit avant moi, c'est un index qui en vérité un écran de fumée parce qu'il n'y a aucune contrainte. La seule contrainte qui est demandé aux entreprises, c'est la publication, on voit bien que vous êtes extrêmement loin des enjeux et que c'est un recul terrible que votre réforme pour la plupart des salariés. Si cher collègue et la parole est maintenant à notre collègue Raymonde Poncet mange. Merci monsieur président alors. Là dis donc. Nous allons discuter ici et le 1er d'une maigre série d'atténuation de la brutalité de cette réforme. Je rappelle que ça concerne 3 milliards seulement sur 18 milliards de gains. Enfin, ou plutôt ici une prétendue contreparties demandées aux employeurs. Voilà. Contrepartie sans. Sans contrainte bien sûr car il n'est pas question de sanctionner le comportement des employeurs qui est pourtant à l'origine et le principal responsable de l'effondrement du taux d'emploi des 60 ans à travers cet index le gouvernement en fait fait le lien effectivement avec les effets délétères de son projet de loi pour tous les seniors. Et notamment du sas de précarité et de pauvreté qui va s'allonger. Je rappelle qu'à 61 ans, plus d'un tiers des femmes ne sont ni en emploi, ni en retraite. Plus d'un tiers c'est elles sont sur-représentés par rapport aux hommes. Effectivement, c'est une loi contre les femmes. Nous y reviendrons. Le 8 mars prochain. Donc ces personnes ne vont pas retrouver un emploi, on le sait, entre 61 et 64 et ils iront grossir justement les les rangs ni emploi ni honte ni en cet index s'appuie par ailleurs sur des prémisses non documenté celui que le taux d'emploi des seniors. Ce serait faible comparativement à d'autres pays européens mais c'est normal, nous avons nous partons à la retraite à 62 ans, je le rappelle, nous nous souhaiterions 60 chez les écologistes. Donc du coup c'est pas étonnant que les statistiques d'Eurostat. En s'appuyant sur la tranche d'âge des 55 64 ans trouve que sur la tranche, soit à partir de 60, nous n'avons pas hein. Un bon top. Comparatif.

Donc c'est l'effet essentiellement du comportement des employeurs à partir de 60 ans d'ailleurs sous l'effet des ruptures conventionnelles que vous avez. Cher collègue qui est dû effectivement souvent à des mises en placard. Merci. La parole à Marie-Noëlle Lienemann. D'abord. Indice des seniors ou pas. La réalité. Il y a pas besoin d'attendre l'indice des seniors. C'est que ce l'allongement pourra pouvoir partir en retraite à 64 ans. Va augmenter considérablement la précarité des seniors. Et le nom le grand nombre d'entre eux, qu'on appelle en zone grise, c'est-à-dire qui sont ni en emploi, ni en retraite. Premièrement. Il faut se rappeler que le départ réel en retraite. Aujourd'hui déjà, et deux ans. Avant la date légale de départ en retraite. Et par ailleurs. Il faut savoir que dès à présent. La zone grise des salariés seniors qui sont ni en emploi, ni retraite est considérable. 16,7% des personnes de 62 ans. En 2021 étaient dans cette zone. 3% étaient au chômage. 13 7 en actes. Une une activité ou au RSA. Si la réforme de 2010, c'est ce que nous dit en allongeant la durée de pour pouvoir passer légalement en retraite ça va inciter ça va allonger et améliorer l'emploi des seniors. Alors on a déjà le bilan de la réforme 2010. La réforme 2010 qui a fixé à 62 ans, le départ n'a fait gagner que 20 points d'activité pour les seniors. 20 points. Et par contre a augmenté considérablement la fameuse zone grise des salariés en question. Ça n'a pas été une amélioration de l'emploi des seniors. Ça a été une détérioration de la situation massive des seniors qui sont dans cette zone grise. Évidemment c'est très inégalitaire. C'est très inégalitaire. Parce que le nombre d'ouvriers en zone grise. Pendant ce temps, lui, augmenté de 16%. Et en 2019 à 61 ans. Il y a plus de seniors qui sont dans la zone grise que de seniors qui sont en emploi. C'est donc on voit bien qu'on est en train de changer structurellement. Les dernières années de la vie des seniors avant qu'on d'avoir droit à la retraite. Alors on aura le temps de poursuivre l'argumentaire mais lundi senior à côté tout ça c'est évidemment

dans la majorité sénatoriale sur ce véhicule ne soit pas plus nombreuses. Nous allons donc discuter d'un indice d'un index senior dont l'avis du Conseil d'État que nous n'avons pas dit qu'il est manifestement inconstitutionnel. Moi je fais une totale confiance au rapporteur Savary. Qui sur ce sujet à un désir de travailler et d'amélioration de la situation. Je suis surpris parfois par les propos puisqu'il dit, nous avons accepté cet indice comme si au fond, la loi avait été dit les et déjà négociés avant de venir dans l'hémicycle mais je suis certain que c'est exactement le genre de sujet qui mérite un débat dans notre assemblée et qui méritent de trouver des solutions parce que garder l'expertise des seniors dans l'entreprise est un enjeu pour notre pays et parce que garder des conditions de rémunération d'emplois de qualité de travail et de santé au travail est un enjeu pour tous les salariés concernés. Donc voilà un beau sujet. Manque de chance, nous sommes dans un projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale et donc ce débat qui mériterait d'être mené. Nous allons le mener à partir de cet article de. Mais vous avez évacué les amendements que ah a très bien présenté Khattiya pour chaud notre collègue et qui traitait justement de cette question des seniors au travail avec une vision alternative. C'est dire à quel point le détournement de procédure auquel vous vous livrez malmène la possibilité d'un véritable débat sur le fond du travail et je le redis, ça n'est pas acceptable. Enfin puisqu'il ne reste plus que 23 secondes et je ne veux pas dépasser. Je vais vous dire que cette indique Senior, ça a été dit par d'autres il y a déjà un indice de l'égalité femmes hommes qui fait qu'aujourd'hui il y a 8% d'écart de rémunération entre les femmes et les sommes, mais cet indice senior. Moi je vais vous le dire, pour moi c'est l'index 9 3 quarts d'Harry Potter à King Cross, il suffit de traverser le mur, vous arrivez et puis d'un seul coup ça va aller mieux. Non il y a beaucoup d'illusions. Je pense qu'il faut travailler avec les partenaires sociaux pour améliorer le travail des seniors. Merci, cher collègue, la parole à Jean-Yves Leconte. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord je voudrais remercier notre. Rapporteur pour les explications et l'importance qu'il a donné. Au sujet même si. Je souhaiterais d'abord lui poser la question de savoir si, selon l'expression de notre collègue Alain Mion cet article n'est pas un cavalier social compte tenu de ce qui a pu être dit sur. Finalement. la pénalité. Qui. Ne semble pas aller au financement de la Sécurité sociale. Donc j'aimerais une précision sur ce sujet. Il est vrai que le taux d'emploi des seniors, plus que toute autre chose est l'outil le plus puissant pour essayer essayer de rééquilibrer. Ou de mieux financer le système de retraites et que lorsqu'on constate le faible taux d'emploi des 60 des 55 64 ans hein qui est bien plus faible en France que dans le reste de l'OCDE. On voit qu'il y a des marges de progression importante toutefois. Il est vrai et il est particulièrement inquiétant de constater qu'en repoussant de 62 à 64 ans l'âge légal la zone grise comme l'indiquait Marie-Noëlle Lienemann va conduire. Plus longtemps et plus de personnes dans une situation de précarité. Le nombre de personnes au RSA. Le nombre de, le le le chômage les maladies. Et les allocations d'invalidité tout cela certaines estimations les monte à près de 5 milliards d'euros, donc plus du quart des économies entre guillemets envisagée par la réforme, alors Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous donner une estimation sérieuse de la situation à taux d'emploi des seniors constant du coup de ce report de 62 à 64 ans pour l'ensemble des autres prestations sociales enfin bien entendu cette. Publication c'est juste une publication c'est-à-dire que finalement cet article ne prévoit rien pour répondre au problème simplement une obligation d'information qui. Finalement ne changera rien s'il n'y a pas d'autre politique qui sont développées et c'est la raison pour laquelle je voulais saluer les. L'intervention préalable de notre rapporteur. Merci. La parole à Corinne Féret. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en matière d'emploi des seniors, les statistiques nationales officielles sont là pour en attester. Le taux d'emploi des 60 64 ans et seulement de 35,5%. en repoussant de 2 ans l'âge légal de départ en retraite. On va augmenter d'autant la durée de chômage d'une grande partie des travailleurs âgés qui sont à la recherche d'emploi tout en réduisant encore davantage leurs droits à retraite quand ils seront en âge d'y prétendent. Le gouvernement se garde bien aussi d'évoquer les coûts cachés de sa réforme paramétrique. Une étude de l'Unédic qui était publié cette semaine, portant sur les Liens entre assurance chômage et système de retraite. Depuis la réforme de 2010, confirme un pic de rupture conventionnelle, 3 ans avant l'âge légal de départ à la retraite. Ce faisant, les dépenses d'indemnisation chômage des plus de 55 ans ont augmenté de 38% depuis 2010 et sont passés de quatre de 8 milliards d'euros au moment de la réforme à 6,7 milliards en 2022.

dans ce contexte, on voit mal comment créer un index seniors pour valoriser je cite les bonnes pratiques en matière d'emploi des seniors. Comment donc cet index seniors pourraient avoir le moindre impact sans sanction cet index n'aura aucun aucun pouvoir de contrainte sur pour les entreprises. Au final, les seniors sans emploi non encore à la retraite n'auront pas d'autre choix que de journées de se tourner vers d'autres filets de sécurité. Revenu de Solidarité Active, l'allocation chômage ou invalidité. Merci. La parole à Marie-Arlette Carlotti. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le gouvernement jure qu'il veut prendre à bras le corps le problème du chômage des seniors. Mais nous constatons une fois de plus que vous nous faites encore de fausses promesses. Monsieur le Ministre, la moitié des salariés ont déjà perdu leur emploi lorsqu'ils prennent leur retraite sans salaire, sans retraite les conséquences sont désastreuses pour beaucoup. Certains sont pris en charge par d'autres filets de sécurité. RSA, allocations chômage ou invalidité mais pour tous, absolument tous et la précarité. ce ce là votre réponse est extrêmement décevante. Vous proposez de créer un index seniors fin de carrière pour valoriser les bonnes pratiques. Une mesure qui se limite pour les entreprises à publier des indicateurs sans prévoir de sanctions. Mais vous pensez vraiment, Monsieur le Ministre, que les chefs d'entreprises vont être sensibles à tout ce qui touche à leur bonne réputation. Nous le savons, vous avez reculé sous la pression du MEDEF encore par en revanche vous restez sourd par rapport aux manifestants qui tous les mois vous disent et le sept encore ça va être le cas que de votre retraite. Ils n'en veulent pas. En fait, vous faites un pari. Le pari qu'un recul de l'âge de départ à la retraite va augmenter automatiquement l'emploi des seniors. Mais vous le savez, il y a un vrai risque que le prolongement de l'âge légal provoque justement un pic de rupture de contrat. Aucune de vos mesurettes ne nous donne satisfaction. et de là je parle encore que des seniors actifs, ceux qui sont encore sur le marché de l'emploi mais que fait-on des plus éloignés de l'emploi, il serait à 1,4 millions d'hommes et de femmes surtout de femmes d'ailleurs de 53 65 ans à ne pas avoir suffisamment cotisé pour pouvoir partir à la retraite et que si ils survivent comme ils peuvent. En attendant, le taux de pauvreté des seniors n'ayant ni emploi ni retraite atteint le chiffre de 32% mais c'est énorme, c'est 5 fois plus que pour les seniors en emploi ou à la retraite, et monsieur le ministre, il y a fort à penser

pour 2 raisons, la première, ça a été dit à de nombreuses reprises. Ce que l'on sait dans la presse, de l'avis du Conseil d'État, c'est qu'il est probablement anticonstitutionnelle et pourquoi parce que dans un projet de loi rectificatif de la Sécurité sociale doit de finances. Pour être constitutionnelle. Il faut que les mesures est un impact financier Direct sur les finances de la Sécurité sociale sur l'année en cours. Or, apparemment, il est fort probable que ça ne soit pas le cas, ce qui veut dire que ça ne sert à rien puisque si ça servait à quelque chose, on aurait un meilleur emploi des seniors, plus de cotisations sociales et donc ça aurait un impact si ça n'en a pas. C'est bien que cette mesure ne sert strictement à rien. La 2ème raison c'est que l'article a été rejeté par l'Assemblée nationale. Alors, le gouvernement s'est beaucoup plaint de l'attitude de l'opposition de l'obstruction, qu'on n'avait pas pu pu voter discuter de tous les articles. Et quand il y a un article qui est voté qu'il ait rejeté. Ça vous intéresse pas. Moi je comprends pas. La 2ème, chose que je voulais dire, c'est sûr. Sur le fond, qu'est-ce que c'est cet index, au fond, on a déjà l'exemple avec l'index sur les les inégalités salariales et le résultat c'est quoi, c'est que ça ne sert absolument à rien hein parce qu'il y a pas de sanction de parce que c'est tellement mal fait que même les indicateurs sont faux, on a en France des entreprises où il y a des inégalités salariales énorme et qui ont des notre magnifique. 100 pour 190% et cetera donc c'est comme essayer de soigner la fièvre avec un thermomètre ça ne sert absolument à rien, si vous voulez vraiment améliorer l'emploi des seniors, fait des choses qui améliorent la voix des seniors et il y ait des sanctions, investissez dans la reconversion des seniors qui sont dans les dans les entreprises des activités polluantes qui vont disparaître et qui s'y sont pas formés à se reconvertir ne trouveront pas de boulot après avoir été licencié là en l'occurrence, qu'on a ne sert absolument à rien absolument à rien et je ne comprends pas qu'on soit même en train d'en discuter. Y et je passe la parole à Jacques Fernique. Oui, merci Monsieur le Président. L'examen de de ce cavalier social l'examen de cet article sur l'index senior ça ça nous apporte une une illustration assez claire de la façon dont le gouvernement considère la démocratie parlementaire. Ce fameux Index a été son nom l'y prédestinait mise à l'index puisque cet article a été rejeté. Ça vient d'être dit par les députés et il sera peut-être sans doute probablement censurée par le Conseil constitutionnel. Mais le gouvernement renvoie cet article devant le Sénat sans doute pour espérer atténuer si c'était possible l'impopularité lourde de cette réforme brutale en Alsace les adeptes du vélo ont ont une expression pour appeler ça, ils appellent ça pédaler dans la choucroute, passez-moi l'expression. Alors que que l'Unédic estime que le report de l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans a entraîné entre 2010 et 22, une hausse de 100.000 bénéficiaires de l'assurance chômage de plus de 60 ans, le gouvernement s'obstine à vouloir détériorer encore un peu plus le taux d'emploi des seniors en France et ne pouvant plus donc nier que leur réforme aura logiquement un impact négatif sur l'emploi des seniors. Le gouvernement est prêt à à toutes les manoeuvres pour tenter de de de cacher les conséquences. Catastrophiques de cette réforme et pour laisser penser qu'ils oeuvrent en faveur de l'emploi des seniors, cependant. Personne n'est dupe. Cet index obligeant seulement les entreprises à publier chaque année des indicateurs de suivi relatifs à l'emploi des seniors dans l'entreprise n'est qu'un écran de fumée qui n'améliorera en rien l'emploi des seniors, puisqu'il n'oblige pas les entreprises à présenté des résultats satisfaisants. Alors c'est ça a été dit inspiré de l'index d'égalité professionnelle alors que même que celui-ci n'a pas montré d'impact particulier dans la lutte contre les inégalités. Hommes-femmes. Comment le gouvernement hostile exiger des Français qui travaillent jusqu'à l'âge de 64 ans alors même que nous savons qu'en 2021, seulement 56% des plus de 55 ans occupé un emploi. Merci. La parole à monsieur Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre. On a lu ce matin que cette réforme était une réforme de gauche. On répond que c'est une réforme qui résulte d'une initiative du PLFSS de la majorité sénatoriale pour partie d'autres pourraient être tentés de dire que c'est le en même temps finalement, peu importe ce qu'on cherche c'est l'intérêt commun et le bien général. Et je pense que cet index seniors il y participent. Et nous sommes au groupe UC favorable à cet un index seniors sur la question de la forme et du droit. Le Conseil d'État rend un avis mais enfin, le Conseil constitutionnel. On verra bien ce qui le rendra comme comme avis lui-même il, il sera bien toujours temps de de voir si c'est un cavalier et donc il est intéressant d'aborder cette question parce que l'emploi des des seniors. Est indispensable si on veut équilibrer cette. Réforme et plus largement le système de répartition et là il y a du travail, disons-le, il y a du travail, 57% des des 55 64 ans sont en emploi dans notre pays, contre 75% en Allemagne que le seuil de 300 et raisonnable. Pourquoi, parce que c'est à partir de ce seuil que nous abordons que les entreprises à bord des questions comme le bilan social mais il y a une différence. Mes chers collègues. Avec ce que vous venez de dire, nous on désespère pas du tout de l'emploi des seniors. Nous pensons que les seniors peuvent être très utiles dans les, dans les années à venir dans l'entreprise on nous pensons aussi que cet index seniors et cette question de l'emploi des seniors. C'est une question qui concerne le paritarisme. Qui demande du grain à moudre s'du grain à moudre Alim. À l'image de ce qui se passe dans le modèle rhénan et enfin on désespère pas non plus à la différence de ce qu'on entend de la responsabilité sociale des entreprises, sociale et sociétale des entreprises et des entrepreneurs et c'est tout le sens de cet index seniors, je vous remercie. Merci la parole est maintenant à nos. Merci bien. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ce matin j'ai évoqué le rêve ou plutôt le cauchemar que j'avais fait d'une flopée de livreurs à vélo de plus de 65 ans qui paie d'aller trop doucement et qui vous livrer des repas froids déclenchant votre courroux. J'ai évoqué cela hein parce que je souhaitais parler de la sous-déclaration massive de leurs revenus. Un article précédent, je souhaite poursuivre lors de cet article De vous décrire une réalité contemporaine d'une catégorie de travailleurs pauvres soumis à une forte pénible une pénibilité et qui gagne très peu. Vous conviendrez qu'ils ne sont pas des fainéants. J'insiste lourdement. Selon la sociologue. Laëtitia da blanc, spécialiste de la question. Ils gagnent en moyenne beaucoup moins que le seuil de pauvreté, aux alentours de 590 euros par mois, le revenu pas le seuil de pauvreté, seuil de pauvreté est presque au double. Par ailleurs, la proportion de travailleurs irréguliers est en forte croissance sans que vous ne mettiez Monsieur le Ministre, les moyens de contrôle nécessaires pour y fixer des des limites. J'ai eu lors de la défaite de la Saint-Nicolas, à Nancy un échange avec un groupe de travailleurs pauvres pauvres livreurs à vélo dans un français tout à fait approximatif en même temps qu'il part, qu'ils parlent de leur situation extrêmement pénible et ils nous demandent. de les laisser travailler parce qu'ils n'ont véritablement rien donc quand on parle de faire travailler au-delà d'un certain âge dans certains métiers, sans prendre en compte véritablement la pénibilité ça n'est absolument pas acceptable. Je vous remercie. Merci monsieur dessus. Merci Monsieur le Président. Alors ça, beaucoup de choses ont été dites, mais on attaque vraiment la partie la plus gadget de ce projet de loi avec ce, ce, cet article 2 sur la création d'un index seniors la publication pour certaines entreprises un certain nombre d'indicateurs relatifs à l'emploi des salariés les plus âgés. Mais alors au-delà de la fragilité législative de la présence de cet article dans ce PLFR de la sécurité sociale cet article il existe. Parce que vous êtes bien conscient que c'est de votre réforme arrive dans un contexte extrêmement dur. Concernant l'emploi des seniors et vous allez agraver évidemment tout ça en reculant l'âge de 62 à 64 ans vous allez voler aux Français. 2 ans de vie pour beaucoup les meilleures années de la retraite, vont être transformés dans les pires années de travail pour ceux qui travaillent parce qu'en fait vous feignez d'ignorer les informations relatives vous on demande aux entreprises. Mais les données, on les connaît. Ça a été dit, je suis se plonger dans les rapports de la Darès ou l'adresse, 35% des 60 64 ans occupe un emploi la Darès comptabilise 1,4 millions de chômeurs de plus de 50 ans au dernier trimestre Will 22 dont 865.000 depuis plus d'un an 20% des ruptures conventionnelles individuelles ont concerné les plus de 50 ans en 2020 un tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent en dessous du seuil de pauvreté. Alors votre il va rien corrigé, il va jusqu'. C'est ce qu'ont constaté ce que l'on sait déjà et sans contrepartie ou contraintes liées à la plus publication des données de la son impact dans les finances, pardon de la sécurité sociale. Donc vous avez déclaré que vous allez peut-être mettre des dispositifs concernant l'employabilité des seniors dans un futur projet de loi sur le travail. C'est pas anodin comme annonce puisque vous êtes bien conscients de la brutalité de cette réforme même et de la faiblesse de vos mesures d'atténuation de cette brutalité dont vous annoncer d'hypothétiques mesures à venir. Mais alors, n'attendez pas de nous un chèque en blanc. Nous combattrons en bloc votre projet de. Report de l'âge de départ à la retraite et votre gadget. Monsieur Chantrel. Merci monsieur le président. On a effectivement un un souci quand même avec cet article puisque comme ça l'a été très bien rappelé avec par mes collègues. C'est quand même un article qui a été rejetée par par l'Assemblée nationale que vous avez décidé de représenter devant le Sénat. Ça montre quelques pas, le peu de fait que vous faites, vous faites du Parlement. En nous proposant un nouveau c'est un irrespect par rapport à à l'autre assemblée mais passons. Je vais en 2019 Emmanuel Macron. Faisait lui-. Même constat que les gens avaient du mal à rester en emploi après l'âge de 55 ans, il déclarait à l'heure, je cite, on doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens mais bons amis aller travailler plus longtemps. Voilà des propos frappée au coin du bon sens. Le taux d'emploi des 60 64 ans en France est inférieur à la moyenne européenne de senior sur trois sont au chômage en invalidité ou bénéficiaires du RSA en plus d'être socialement insupportable cette, cette situation est la première cause du déséquilibre de notre système de retraite et au lieu d'améliorer la situation. Votre mesure d'âge va aggraver la précarité des seniors plutôt que découper les arguments à la limite de la schizophrénie de ceux qui veulent se débarrasser des plus de 55 ans, tout en demandant le report de l'âge de légal de départ en retraite. Écoutons l'Emmanuel Macron de 2019. Écoutons aussi Hervé Lorenzi, titulaire de la chaire Transition démographique transition économique de la fondation du risque. Il explique qu'une hausse de 10 points du taux d'emploi des seniors permettrait au système retraite d'être à l'équilibre il faudra évidemment plus que cet index seniors qui est plutôt un cache-sexe seniors. car sans contrainte significative l'effet sur la réputation de l'entreprise ne suffira pas à lui faire changer bien évidemment son approche de l'emploi des seniors, surtout s'il ne s'adresse qu'aux entreprises de plus de 300 salariés. Vous citez souvent l'index de l'égalité professionnelle alors que justement cela n'a aucun effet en tout cas sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci la parole à Madame Gréaume. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Vous l'avez bien compris, je suis je suis pas d'accord avec cet index seniors et cela vous vous en doutez, car en plus de tout ce qui a été dit, cela va occasionner de nombreux emplois précaires. Mais j'aurai besoin de connaître à partir de quand on est senior parce que selon les la définition de l'Insee on est senior à partir de ça sur le site du gouvernement ces CDD seniors à partir de ça qu'on ne s'étend sur 4 Cadremploi on est senior à partir de 45 à 50 ans et selon certaines entreprises on est senior à 49,6. Or donc je voudrais bien connaître, vous comprenez, Monsieur le Ministre, c'est important pour la bonne raison c'est que plus qu'on est âgé, plus qu'on a des accidents, notamment ça va avoir un effet sur l'assurance maladie. Vous comprenez bien, et je suis sûr que demain il y aura encore des exonérations qu'on va donner aux employeurs pour prendre ces seniors donc en asséchant la sécurité sociale. Comment on va pouvoir payer ses arrêts maladie et notamment. Aussi. Une répercussion sur toutes les les aides sociales parce que si on a des personnes qui sont en invalidité. Il faudra aussi. Forcément les rémunérer et avec la réforme chômage ces personnes âgées vont aussi arriver à un moment ou un autre sur le RSA. Donc je me pose sincèrement toutes ces questions là et en plus de celle-là les des nombreux critères qu'on n'a pas abordé comme les critères de salaire les tours 9h qui risque d'arriver dans les entreprises parce que j'ai du mal à avoir un senior qui va travailler à la chaîne chez Renault par exemple les taux de mobilité professionnelle en interne et la part des seniors dans la barre chez la formation, donc j'espère que j'aurai réponse à toutes ces questions et notamment comment on va régler ses problèmes financiers. Merci. Merci madame Le Houerou. Merci monsieur le président. Alors vous avez l'ambition d'améliorer l'emploi des seniors pour cela vous rendez obligatoire pour les entreprises la publication d'indicateurs. La publication d'un index et une faible sanction associée puisque les entreprises seront pénalisés uniquement en cas de non-publication. Pourquoi les projets de sanctions ont été abandonnés, alors qu'il semble que ces sanctions étaient initialement envisagée, celle-ci aurait pu avoir un impact sur les comptes de la Sécurité sociale et aurait peut être justifié la place de cet index à l'article 2 du PLFSS rectifie mais cet index n'est pas un totem. À 61 ans, déjà 61,3 pour % des personnes ne sont plus en activité à 62 ans 73 6% ne sont plus en activité. Le constat, nous le faisons déjà, pas besoin d'un index, ce que nous voulons, c'est une véritable politique de valorisation du travail des seniors et dans laquelle les seniors auraient toute leur place dans l'entreprise et ne que ces personnes d'un certain âge donc à 50 ans à 5 55 ans à 60 ans à 62 ans ne soient pas poussés hors de l'entreprise. En attendant l'âge de départ que vous repoussé à 64 ans avec l'obligation, mais je dirais surtout parfois l'humiliation de terminer leur vie professionnelle au RSA. On sait que l'index égalité femmes-hommes ne fonctionne pas et n'est pas à la hauteur de Lambic de l'ambition pour aboutir à faire changer les choses à faire que les salaires des femmes soit à l'égal de ceux des hommes et qu'elles puissent accéder aux postes de responsabilité, la situation des seniors sur le marché du travail en France est très mauvaise, donc quelle politique d'emploi des seniors, prévoyez-vous. La parole. À David Assouline. Merci monsieur le président. Je. Je réfléchissais, je me disais-je chercher un mot pour qualifier cet article là. Et puis j'ai j'ai trouvé cette citation. Mars 2019. 2019. Franchement ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal de départ en retraite. Quand on est soi-même en difficulté. Il faut du courage pour arriver à 62 ans. Emmanuel Macron, donc lui il dit hypocrite, c'est l'article hypocrite dans l'hypocrisie de cette loi, parce que vous le savez l'Unédic vient de donner une étude au 1er mars de cette année. Qui se penche sur le moment où on est passé de 60 à 62 ans. Et. Son évaluation c'est que il y a eu 100.000. Demandes. Bénéficiaires des allocations d'indemnisation du chômage en plus 100.000 mécaniquement. Et si on regarde la période 2010 a aujourd'hui. L'augmentation du chômage des plus de 55 ans a été de 38%. Donc ça c'est. La réalité, et vous le savez très bien et le président de la République quand il disait ça en 2019, savait très bien que, mécaniquement. Dans un pays où le chômage des seniors et massif. Augmenter de deux ans s'est prolongé ce chômage et. Bien sûr l'accroître. Et et et crée une situation de fragilité parce que là c'est les bénéficiaires de l'indemnisation chômage. Mais tous ceux qui sortent des circuits d'indemnisation. À ce À ce moment-là il y en a beaucoup et ils sont dans une situation de précarité, bien plus grave bien plus difficile et donc. Très franchement, venir nous dire parce que vous avez conscience de ça. Donc le seul sujet, je le répète de cette loi c'est de faire de 62 à 64 ans, le reste c'est de l'habillage c'est de l'hypocrisie totale. Et je pense que là-dessus dessus on le démontrera à travers les nombreuses discussions qu'il aura encore sur cet article. Merci de vos encouragements. Merci monsieur Assouline. Donc nous en avons terminé avec les prises de parole sur article et je vais donner la parole à monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Quelques mots à mon tour sur. La question de l'index senior et hausse de la sur la question de l'emploi des seniors. Quelle est l'intention du gouvernement et quelle est la démarche dans laquelle nous sommes. L'intention du gouvernement, c'est le ce que porter le projet de loi, telle qu'initialement proposé devant l'Assemblée nationale et créent un outil de mesure de l'implication des entreprises pour l'emploi des seniors. De faire en sorte que cet outil s'applique aux entreprises de plus de 300 salariés. Et de la sortir finalement. De, de conditions de 2 outils de contrainte ou d'encouragement. Premier routiers l'obligation de publicité de l'index de l'emploi des seniors, pour les entreprises de plus de 300 salariés. Dès 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Et j'insiste sur le fait que ces de 2023 pour les entreprises de plus de 1000 salariés puisque dans la mesure où nous avons prévu et que nous proposons au Parlement d'adopter ces dispositions que les pénalités versées par les entreprises qui se soustraire à cette obligation de publicité soit versée directement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est ce mécanisme, qui a un effet Direct sur les comptes sociaux de l'année 2023 puisque

Nous avons un deuxième outil que nous avons prévu. Qui est de réintégrer la question de l'emploi des seniors dans les items de négociation obligatoire tous les 3 ans pour les entreprises de plus de 300 salariés au type de la gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels. C'est ce que monsieur le rapporteur. Savary a mentionné, il y a un instant, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avions prévu dans le texte initial que cette obligation de publicité s'applique aux entreprises de plus de 300 salariés puisque l'obligation de négociation triennale en matière de gestion des des emplois et des parcours professionnels pour tous les autres items auquel nous ajoutons l'thème de l'emploi des seniors concerne les entreprises de plus de 300. Plus Pour toutes ces raisons, j'aurai l'occasion mais je reviendrai tout à l'heure si les amendements de suppression ne sont pas adoptés. Mais à l'occasion de le l'examen des autres amendements de donner un avis de sagesse à l'amendement de la commission qui propose de ramener le seuil d'application de de 50 à 300. La 2ème, chose que je voulais souligner concernant l'index. C'est que la la majorité présidentielle. À l'Assemblée nationale, proposé un amendement qui prévoyait d'ajouter un 3ème outil d'encouragement ou de contrainte selon le point de vue que l'on a. Cet outil consistait à dire que après. Avoir rempli l'index après que les résultats étaient publiés et au bout de la première période d'observation, parce que dans tous les index. Il y a une période d'observation. Il y a un durcissement des conditions pour faire en sorte que les entreprises qui ayant respecté l'obligation de publicité. Ayant. De droit et et parfois de manière formelle mais ayant été. Contrainte à cette obligation de négociation triennale sur l'emploi des seniors

Cet amendement qui visait finalement à durcir et à rendre effectif. Les résultats de de l'index senior pour les entreprises ne jouant pas le jeu a été repoussée dans la mesure où ces et ce qui est présentant une position à l'occasion de cette discussion de l'article et ce qui nous ont reproché de ne pas avoir un outil assez incitatif. Sont sur les bancs de la gauche. Il faut souligner que l'intégralité des des députés de gauche ont repoussé cet amendement qui prévoyait de durcir les conditions de mise en oeuvre et donc de rendre l'index plus efficace. La 2ème, chose que je voulais dire. Et et de nature plus technique mais certains d'entre vous au travers de leurs interrogations sur la recevabilité. Ont interrogé le gouvernement directement ou indirectement. Sur les effets financiers je l'ai dit. L'absence de publicité, le refus de cette obligation de publicité sera durable par une sanction dès 2023 affecter directement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et et pour plus de précisions. Vous me permettrez de renvoyer à l'annexe II dans ces pages 22 et 23, qui précise justement les effets attendus en en la matière. Je voudrais profiter de cette occasion du du renvoi à l'annexe pour dire que oui, nous sommes aussi inspiré de de l'index en matière d'égalité professionnelle. Que cet index en matière d'égalité professionnelle dont les résultats pour la dernière période d'observation sera rendu public dans la semaine qui vient. Présente des particularités et les premiers résultats dont je dispose. Font que ces particularités sont intéressantes. D'abord parce que la note moyenne et la note est déterminé par des critères qui n'ont pas évolué, et donc on peut garantir la stabilité de la méthodologie. La dette moyenne des entreprises, ceux qui sont assujettis à l'obligation de publication ne fait que croître et c'est tant mieux. Et par ailleurs nous sommes entrés depuis l'année dernière dans la période de mise en oeuvre des pénalités pour les entreprises qui. Voient leur mode se dégrader ou rester substantiellement inférieur. À la moyenne de leur secteur, ce sont plusieurs dizaines d'entreprises de plus de 1000 salariés qui sont assujettis à fonction depuis 2022 et 2023. Bah a priori mais j'attends les résultats consolidés marqué le même mouvement. Vous avez certainement vu ou lu que la première ministre souhaite aussi que nous puissions regarder si le maintien durable avec une note inférieure à 75 points, ce qui est véritablement le bas du classement ne pourrait pas être ne pourrait pas être pardon une condition ou. À motif pour écarter ses entreprises d'un certain nombre d'appels publics mais c'est un sujet qui est à en cours d'instruction. Sur et pour revenir. La question de l'index et de l'emploi des seniors peut-être pour élargir le sujet, au-delà du seul index si je me présentais devant le Sénat en en indiquant que la politique en matière d'emploi des seniors du gouvernement se réduit se réduit à l'index, ça serait évidemment très insuffisant. C'est une première Pierre et nous voulons aller vite. La raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que dès fin 2023, il y a cette possibilité de sanctionner les entreprises qui se soustrairait. À cette obligation de publicité. Pourquoi fin 2023 et pas plus tôt si nous sommes dans l'hypothèse où la loi. Est adoptée par le le Parlement tel que nous le proposons. Parce que nous devons avoir un peu de temps pour permettre aux différentes branches de négocier sur cet index négocier de choses, la première concerne les. Critères les indicateurs que nous voulons soumettre à une négociation une une concertation pardon interprofessionnel au titre de l'article L-1 du code du travail. chose que nous devons laisser pour laquelle nous devons laisser un peu de temps. Discussion. C'est que nous avons indiqué notre volonté que les branches professionnelles puissent procéder à quelques adaptations, si elles le souhaitent aux critères de l'index parce que nous savons que d'une branche à l'autre le nombre de seniors, la possibilité d'employer les seniors peu varier et il nous paraît utile de confier aux branches le soin de négocier quelques adaptations. Mais au-delà, il faut évidemment aller plus loin, aller plus loin avec des dispositions qui sont dans ce texte, notamment le fait de faciliter la l'accès à la retraite progressive pour les salariés affiliés au régime général et de l'ouvrir pour les agents de la fonction publique le fait mais cela renvoie à une disposition que nous prendrons par voie réglementaire. Si les les critères d'assouplissement du du contre du compte professionnel de prévention sont adoptés, le fait que nous facilitons l'accès au temps partiel pour les salariés titulaires d'un. Actuellement, pour bénéficier de 3 mois de temps partiel avant le départ à la retraite. Il faut disposer de 10 points. Nous souhaitons qu'avec 10 points. La période de temps partiel soit portée de 3 mois à quatre mois et donc ainsi permettre pour des salariés titulaires d'un c'est de paix d'avoir accès à plus de temps partiel pour le même nombre de points, c'est une des pistes de renforcement nous poursuivons et puis enfin mais cela été évoqué à plusieurs reprises, je, je ne le cite que pour mémoire le fait de maintenir la plupart de des âges de départ anticipé telle que nous l'avons prévu pour les questions liées au handicap pour les questions liées à l'amiante permet aussi d'accompagner et cela a un coût en termes de perte de rendement. Mais c'est un coup utile permet d'accompagner la mise en place de cette politique, je sais. Monsieur le rapporteur. Parce que vous l'avez dit que votre commission est plutôt favorable si j'ai bien entendu cela. Ah à de dispositions adoptées par l'Assemblée nationale. La première concerne la mutualisation du taux AT-MP pour les salariés de plus de 55 ans puisque nous savons que ça peut être un frein à l'emploi que de recrues qui souhaite recruter un salarié de plus de 55 ans en matière de maladies professionnelles. Les maladies professionnelles généralement se déclenche après une période d'Exposition. Et si un chef d'entreprise aujourd'hui recrutent un senior de plus de 55 ans, en l'occurrence. Et que ce seigneur déclenche une maladie professionnelle, c'est la dernière entreprise qui a recruté qui connaît la majoration du taux AT-MP. Le fait de mutualiser ce taux permet de réduire le risque si on peut dire liées à l'embauche d'un senior exposées précédemment à à des critères pouvant déclencher une maladie professionnelle. La 2ème disposition qui me semble de recueillir votre approbation et celle qui permet d'aligner le régime fiscal et social des ruptures conventionnelles pour celles qui sont passés avant ou après l'âge d'ouverture des droits. Jusqu'à présent. Une rupture conventionnelle décidé avant l'âge d'ouverture des droits à vers un régime fiscal et social à 20% alors qu'une rupture conventionnelle décidée après l'âge d'ouverture des droits et dans l'hypothèse où le salarié continue notamment pour atteindre la durée d'affiliation requise au régime de retraite et avait un taux de 1 To fiscales et sociales, mettent tout le monde à 30% c'est cassé cet effet d'aubaine et c'est éviter d'encourager à des ruptures conventionnelles avant le d'ouverture des droits. Je crois que ça va dans le bon sens. En plus de générer quelques recettes pour nous permettre de tenir notre objectif partagé d'équilibre. Je sais que vous avez enfin travailler et j'en terminerai par ces deux points, sur la question d'un d'un CDI réservé aux seniors dans des conditions particulières et vous savez monsieur le rapporteur. Notre volonté de continuer à avancer, discuter avec vous pour faire en sorte que. Les effets d'aubaine soient les plus minimes possible, nous le savons et que ce soit le le plus efficace possible aussi. Je terminerai par un dernier point pour dire que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale n'est qu'une étape et nous aurons effectivement un projet de loi sur le travail, l'emploi, l'insertion dans dans les prochaines semaines et qui sera présenté à votre assemblée au cours de l'année 2023, je l'espère, avant l'été 2023. Ce projet de loi permettra de porter d'autres dispositions en matière de formation pour les seniors. C'est un enjeu aujourd'hui les salariés plus de 50 ans ont un accès à la formation continue, moitié inférieur aux salariés de moins de 50 ans soit parce que eux-mêmes considèrent que l'investissement en temps en énergie et moins utile, soit parce que leur employeur considère que cet investissement est moins utile. Nous travaillerons aussi sur. Des questions relatives à l'articulation entre les règles d'assurance chômage et la reprise d'emploi. Nous, nous savons par définition. Que reprendre un emploi lorsqu'on est. Ah. Locataire d'un minima social et est toujours une, une opération gagnante si je puis dire. Par contre, nous savons aussi qu'il y a quelques semaines, quelques mois quand on passe d'un système à l'autre canton. Je, là je ne parle pas des seniors mais c'est un exemple, quand on a sur soi-même la garde de ses enfants mais que la reprise d'activité, un poste de trouver un site, un, cette expression les les aides à la garde d'enfant peut créer quelques décalages et empêcher la reprise d'activité. C'est un phénomène qu'on retrouve aussi chez les seniors. Parce que souvent des seniors qui ont perdu un emploi. lorsqu'il perd 7 emploi une rémunération qui tient fond quant à la fois de leurs compétences mais aussi de leur ancienneté dans l'entreprise et lorsqu'il trouve une entreprise qui acceptent de les réemployer. Le chef d'entreprise accepte évidemment payer les compétences mais pas nécessairement de reprendre à son compte l'ancienneté qui n'était pas dans son entreprise et donc il faut qu'on voie comment trouver des systèmes d'incitation pour les seniors à la reprise d'emploi tout en tenant compte de ces différences de revenus et enfin mais vous l'avez compris, je je souligne à plusieurs reprises la complexité de ce que nous faisons. Madame Gréaume a posé la question de, de l'âge à partir duquel on est senior. C'est une des raisons parmi. Celles que j'ai évoquées qui nous amène à privilégier la concertation et notamment le renvoi de branche parce qu'effectivement, et vous l'avez dit Madame dans votre intervention l'âge à partir duquel on est senior. Est assez variable.

et donc nous préférons renvoyé à cet âge-là parce qu'en réalité, dire à partir de quel âge on on est senior. C'est quelque chose qui est finalement assez différent d'un secteur à l'autre et parfois même d'une personne à l'autre raison pour laquelle vous ne trouverez à aucun moment dans le texte sur l'index des seniors en tout cas dans ce qui en fait des dispositions législatives un renvoi explicite à l'âge pour ne pas gêner et ne pas figer le le débat que nous attendons des branches professionnelles. Voilà. Monsieur le Président, je dirais un peu plus vite. Je vous en je je vous en Les explications de position du gouvernement. Pardonnez-moi sur les différents amendements mais je pense utile de rappeler, c'est, c'est l'état d'esprit qui est le nôtre pour cette question de l'emploi des seniors. Monsieur le Ministre. Donc nous allons commencer à examiner les amendements et commencer par 49 amendements. De suppression. Et le premier de ces amendements et présenté par Monsieur Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, chers collègues, après les interventions sur articles des différents collègues de gauche mais aussi après l'intervention du ministre à l'instant. Finalement. Assez longue et assez précises sur cette question de l'emploi des seniors. Je vous propose le premier amendement de suppression de l'article et y compris l'intervention du ministre me renforce dans la conviction qu'il faut le supprimer. Non pas parce que nous n'aimons pas les gadgets après tout cet article pourrait ne servir pas rien mais à pas grand chose et ce n'est pas grave. Sauf qu'on ne résout pas un problème aussi grave que celui des chômage c'est du chômage des seniors dans notre pays par un gadget et peut être que le seul caractère financier de cet article enfin. Si ce qu'on sait de la note du Conseil d'État est exact. Eh bien peut-être que son seul caractère financier c'est que cet article soit pour solde de tout compte en matière d'emploi des seniors. Or, c'est un sujet absolument dramatique dans notre pays et la réforme des retraites que vous proposez va bien plus l'aggraver, que vous ne vous vous ne le dites dans les différents éléments ces dernières semaines qui se sont révélés et qui montre les approximations, les contre-vérités les erreurs aussi du gouvernement dans la présentation de sa réforme, hé bien il y a l'étude de l'Unédic qui indique que votre réforme pourrait augmenter de 100.000 personnes le nombre de seniors au chômage dans notre pays pour quel coût pour les finances publiques dans leur ensemble, d'ailleurs nous ne le savons pas et pour combien de difficultés sociales accrues. Aggraver là nous ne le savons pas non plus et nous aurions évidemment besoin de le savoir. Alors nous proposons cet amendement de suppression de l'article pour que. Vous ne puissiez pas maître comme ça la charrue avant les boeufs. Vous proposez beaucoup de concertations et beaucoup de report à la fin 2023 pour travailler sur l'emploi des seniors, commencer par faire de même avec votre réforme des retraites. Merci. Monsieur plat n'est pas là donc je passe la parole pour la mention Madame Bricq. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Amendement de suppression de cet article là aussi puisque avec cet article le le gouvernement donc mis en place un index seniors fin de carrière pour valoriser les bonnes pratiques dans les entreprises. Pour ce faire il rend obligatoire pour les entreprises la publication d'indicateurs. Cet index seniors aurait du sens à la limite s'ils s'inscrivaient dans une véritable Blois en faveur de l'emploi des des salariés âgés. J'ai bien entendu Monsieur le Ministre, vous opposition tout à l'heure nous attendrons, bien entendu. Cette ces dispositions en faveur de de l'emploi des seniors avec impatience dans le cas d'une vraie loi travail. En l'espèce un index sans objectif ni sanction du non respect de l'objectif. N'aura aucun effet sur les entreprises qui ont plutôt tendance à pousser les plus âgés vers la sortie. Nous le savons les 2 tiers des licenciements et des plans sociaux sont en effet subies par ses salariés. La situation des des seniors sur le marché du travail en France n'est pas bonne et ce n'est pas un index seniors qui va y changer quoi que ce soit. À ce titre, les chiffres de la Dares parlent d'eux-mêmes en 2021, le taux d'emploi des seniors en France est nettement inférieur à celui de l'Union européenne. Par ailleurs, la part de temps partiel, augmente considérablement avec l'âge, pour ceux qui sont en emploi. Car pour les autres la réforme des retraites du gouvernement conjugué à la réforme de l'assurance chômage va faire basculer dans la précarité. Les demandeurs d'emploi proche de l'âge légal de départ à la retraite aujourd'hui fixé à 62 ans. Ceux-ci vont voir leur durée d'indemnisation chômage amputé de six mois la seule perspective sera alors le RSA lui-même conditionné à 15h d'activité par semaine. Il est sûr qu'à la fin d'une vie de labeur. Ça fait rêver, Merci cher collègue. Et la parole est maintenant à entre collègues Corinne Ferré. indiqué j'ouvre les guillemets, qu'il n'existe aucun dispositif miracle ni incitatif ni punitifs qui puisse régler à lui seul à lui seul le problème de l'emploi des seniors. Ainsi, avec cet index seniors le gouvernement fixe une obligation de publication d'indicateurs aux entreprises et non une obligation de résultat. La nuance et là elle est importante cet index seniors risque donc d'être inefficace dans l'amélioration de l'emploi des seniors. Pourtant, l'emploi des seniors est un paramètre clé du système de retraites sans même toucher à l'âge de départ, une augmentation du taux d'emploi des 55 64 ans, de 10 équilibreraient, le système des retraites d'ici à 2032, en tenant compte de 30 milliards d'euros de surcoûts. Compensé par l'État employeur notamment pour les fonctionnaires et les régimes spéciaux des entreprises publiques. À l'inverse, l'adresse a ainsi estimé qu'un report de 2 ans de l'âge légal de départ à la retraite engendrerait un surcoût pour l'ensemble des prestations sur mon assurance chômage de l'ordre de 3,6 milliards d'euros, soit 35% des économies recherchées d'ici 2027 par la réforme du gouvernement. D'autres mesures aurait été plus efficace pour améliorer l'emploi des seniors mais démonstration est faite que cette proposition de mettre en place une un index n'apporte rien de plus. Merci, maintenant l'amendement 456, monsieur. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est c'est une, un drôle de, de raisonnement. C'est-à-dire qu'on dit ben voilà on va reporter le départ. De l'âge à la retraite à 64 ans, donc on met deux ans de plus de travail aux seniors en question et puis on dit aux entreprises, ben vous allez nous à travers un index nous donner des indications sur le niveau d'emploi des des seniors c'est-à-dire que on va leur donner une charge administrative en plus alors qu'elle se plaignent déjà d'en avoir beaucoup pour donner des informations qui somme toute ne serviront à rien. Les seniors. Qui sont du coup mis à l'index ne sont pas des fainéants. C'est pas des gens qui ne veulent pas aller travailler. C'est des gens qui malheureusement pour une grande majorité passer entends se retrouvent soit au chômage, je suis en arrêt longue maladie. suis à la recherche de travail, il leur faut des dispositifs d'accompagnement qui font de la formation professionnelle mais aussi des offres d'emploi qui chante a adapté à leur situation d'hommes ou de femmes de 60 ans, si je prends un exemple qui me touche de près. L'industrie agroalimentaire en Bretagne. On sait aujourd'hui qu'une personne qui a travaillé pendant 25 30 ans à la chaîne et totalement épuisé a souvent fait l'objet d'ailleurs d'interventions chirurgicales pour des troubles. Ce que l'eau musculo-squelettiques et donc cette personne-là. Est en difficulté pour retrouver un travail. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des mesures d'accompagnement. Il faut lui trouver des postes adaptés et croyez-moi, elles seront vraiment très heureuse de pouvoir s'épanouir dans de nouveau dans des nouveau boulot donc ne change de cet amendement. Ça veut dire que l'index n'est pas signifiant et donc on demande le retrait de l'article, je vous remercie.

Il suffit de consulter les études de la Darès et de l'adresse pour mesurer l'ampleur de l'enjeu. Seuls 35% des 60 64 ans occupe un emploi. Et 20% des 427.000 ruptures conventionnelles individuelles concernés les plus de 50 ans en 2020. Selon l'adresse 4 millions de personnes âgées entre 53 et 69 ans ne perçoivent ni revenus d'activité ni pension de retraite prolongé de de gens. L'âge du départ légal de la retraite sans avoir obtenu au préalable des résultats tangibles en matière d'emploi des seniors n'est pas responsable. Compte tenu des conséquences d'une d'une telle mesure. Cela se traduira par une aggravation de la précarité des seniors après avoir épuisé leur droit au chômage que vous avez déjà rogné réduit par votre précédente réforme, ils seront poussés vers les minima sociaux et devront recourir à d'autres filets de sécurité en attendant d'accéder à leur pension de retraite maladie incapacité préjugés négatifs des employeurs manque d'accès à la formation. Telles sont les principales raisons qui expliquent le faible taux d'emploi des seniors. Ce n'est donc pas un index aux aux modalités inconnu qui permettra d'y remédier. Mais l'instauration d'un véritable plan pour les seniors passant par l'amélioration des conditions de travail et l'investissement dans la formation. Vous avez déclaré que des dispositifs consacrée à l'employabilité des seniors sera annoncé dans un futur projet de loi sur le travail. N'attendez pas de nous un chèque en blanc. Des mesures hypothétiques et longue à se concrétiser contre la présente. Réforme des retraites qui aura un impact immédiat sur les individus, fragilisant davantage une tranche d'âge en grande difficulté d'accès à l'emploi.

je défends donc comme mes collègues un amendement de de suppression et je voudrais simplement dire au gouvernement et et et à la majorité sénatoriale que ici, le problème est pris à l'envers parce que ça été rappelé tout à l'heure une étude montre que 10% d'augmentation de du taux d'emploi des seniors permettrait de résoudre le problème financier qui était évoqué par le gouvernement présenté d'abord un projet de loi sur la réforme du travail des seniors avant de faire cette réforme des retraites. Le 2ème point. C'est pour répondre au au répondre commenté en tout cas une L'intervention du du ministre-tout à l'heure. Qui a détaillé de manière très précise. L'ensemble du dispositif et qui a évoqué le fait que la sanction financière hypothétique mais néanmoins prévue par le texte serait reversés à la caisse et on voit peut-être poindre là une forme d'habileté, habileté parce que de ce fait peut être le gouvernement. Imagine pouvoir contourner la difficulté de la recevabilité constitutionnels de ce dispositif dans un projet de loi de financement de la Sécurité sociale et à ceux-là je dis au ministre et à ce qui pourrait être convaincu éventuellement par cet argument, qui n'en est rien. Pourquoi, parce que les sanctions n'arriverait qu'après l'échéance d'un an qui constateraient l'éventuel non-, respect de la publication du 10. ensuite du 10 indicateurs ensuite rappelé Michaël Zemmour qui a fait une célébrité depuis qu'il a débusqué la la la la tartufferie de la pension à 1200 euros on peut estimer que la réforme des retraites augmentera le nombre d'allocataires des minima sociaux. RSA et l'ASS de 60.000 le nombre de personnes au chômage indemnisé de 84.000 et que de ce fait on aura environ 150.000 à 200.000 personnes dans le sas de précarité entre l'emploi et la retraite, que nous n'en voulons pas et nous aurons l'occasion de dire pourquoi est-ce que ce qui est proposé par la droite du Sénat est encore pire que ce qui est proposé dans cet article. Merci monsieur renonce Arazi n'est pas là, donc le 673, madame Le Houerou. Par cet amendement. Donc 673, je demande la suppression de l'article de. Oui c'est ça hein. Sans contrainte pour les entreprises. Ce dispositif n'aura aucun impact concret sur l'emploi des seniors. Je rappelle à 60 ans près d'une personne sur 3 n'est ni en emploi, ni à la retraite. La majorité d'entre elles en situation d'invalidité de RSA ou de chômage et donc dans une grande précarité. Et insécurité en fin de carrière. Selon le ministère du travail en 2020, le taux d'emploi des 55 64 ans était de 53,8% sous la moyenne européenne bien sûr et très loin de la Suède et de l'Allemagne qui dépasse les 70 102 tiers des licenciements et des plans sociaux sont subies par ses salariés seniors. Alors plutôt que de repousser l'âge légal de départ à la retraite, permettant aux seniors, une meilleure insertion dans l'emploi déjà jusqu'à l'âge légal aujourd'hui fixé à 62 ans pour dissuader les politiques anticipent anti-. Senior de certaines entreprises travaillant sur la pénibilité au travail sur l'amélioration des conditions de travail. Or les quatre critères de pénibilité qui vous ont que vous avez supprimé en 2018, explique la difficulté d'emploi des seniors qui sont cassés. À 50 ans et même avant. Elle souffre de troubles musculaires ou musculo-squelettiques, c'est-à-dire de douleurs intenses pour avoir travaillé dans le dans le froid dans des postures pénibles avec David vibrations mécaniques ou exposés à des risques chimiques empêchent le travail proposé par certaines de nos entreprises. Employeuses de main-d'oeuvre et notamment je pense aux industries agroalimentaires qui se trouve dans cette situation dans ma région et donc en l'absence de demande de contrepartie aux entreprises pour améliorer les conditions de travail. Je crains qu'à l'image de l'index, femmes hommes égalité femmes-hommes ce dispositif ne soit ni utile n'inefficace.

obligerait à travailler plus longtemps alors même que les seniors connaissent des difficultés à trouver un emploi, notamment à en particulier dans les grandes entreprises donc cet index seniors. Vise à valoriser les bonnes pratiques. n'imposant dès 2023 cet index senior aux entreprises de plus de 1000 salariés, puis ensuite de 300 salariés en recul par rapport à ce qui avait été proposé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire jusqu'à 50 salariés et la seule obligation, finalement c'est de publier indicateur avec une sanction quand même relativement faible en cas de non-publication et l'objectif de l'index pourrait trouver un intérêt à condition que les entreprises subissent les conséquences d'un index dégradé et donc à condition qu'il y a une obligation de résultat, mais nous n'y sommes pas et en réalité, le gouvernement a reculé face au MEDEF. En refusant d'associer l'index énorme senior à des sanctions initialement. Donc sans sans sanction cet index n'aura aucun pouvoir de contrainte et aucune efficacité. Mes collègues. L'ont évoqué, hein. Les chiffres sont parlants, à 60% il y a le tiers. Des seniors qui sont déjà sans emploi et au delà, ça se dégrade très rapidement très rapidement chaque année supplémentaire donc cette réforme ne fera qu'allonger le sas de précarité, aura des conséquences désastreuses pour de nombreuses personnes qui seront au chômage puis au RSA et cet index ne va pas vraiment améliorer la situation de l'emploi. monsieur Mickael valait n'est pas là donc je passe la parole à Monsieur Jacquin pour le 815. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre. Il s'agit de supprimer cet article. En effet, l'article 2 instaurant un index seniors constituent un véritable cavalier social il ne relève pas du financement de la Sécurité sociale, mais d'une loi travail en faveur de l'emploi des salariés âgés. Le gouvernement confirme ainsi que cette réforme des retraites n'aurait jamais dû passer par un PLFSSR ce n'est que de la petite manoeuvre politique. De surcroît, par une procédure d'urgence dont la constitutionnalité interroge. l'intérêt de disposer des éléments du fameux rapport du Conseil d'État en outre un index de jeu. Sans objectif ni sanction du non respect de l'objectif n'aura aucun effet sur la culture des entreprises. Qui considèrent les salariés de plus de 55 ans, voire de plus de 50 ans qui ont une variable d'ajustement les 2 tiers des licenciements et des plans sociaux sont en effet subies par ses salariés, c'est pourquoi cet amendement entend de nouveau supprimer cet article de et confirmer ainsi le vote de l'Assemblée nationale il y a quelques jours, le fait que le gouvernement, par le truchement de la procédure de l'article 47 1 de la Constitution présente cet article devant le Sénat est une nouvelle preuve du peu de considération qu'il donne à la représentation nationale alors retiré cet article et cette réforme et au-delà de cet hémicycle soyeux. Soyons nombreux mardi Merci. Monsieur Lozach n'est pas là Monsieur dur hein non plus. Monsieur Lurel non plus Madame Artigalas s'. En plus monsieur Cardon, donc je passe la parole au président rénale. Oui, mes collègues déjà bien défendu cet amendement de suppression. Mais tout de même. Tout de même, on peut s'interroger toujours ce, ce qu'on fait

À la question que les questions comme souvent d'ailleurs malheureusement, sont traités dans le mauvais ordre mais ça je crois que tout le monde dans cet hémicycle finalement l'a dit. On aurait dû travailler évidemment d'abord sur la question du travail sur la question évidemment de comment faire en sorte que le, le taux de senior au travail augmente. C'est d'ailleurs ce que disent tous les économistes on peut régler un peu régler assez facilement la question du financement de la retraite si on améliore sensiblement le taux de travailleurs âgés. Bon voilà. Eh bien nous n'y arrivons pas, nous n'arrivons pas à faire les choses dans le bon ordre. Et si je voulais faire un parallèle, c'est exactement la même chose que la suppression de la CVAE. Quand on supprime la c'est même on a tous été d'accord ici pour dire qu'il aurait fallu d'abord expliquer comment les collectivités finalement seraient traités. Et quelles seraient les mesures de remplacement de la CVAE. Pour les collectivités. C'était un des sujets, nous l'avons demandé et là pour le coup sur tous les bancs pour avoir cela avant de supprimer la CVAE dont certains ont dit, on supprime. C'était mon cas, d'autres ont dit en report d'un an mais c'était la même idée, hé bien là on est dans le même sujet, c'est-à-dire qu'on prend toujours les choses à l'envers et c'est terrible de prendre les choses à l'envers sur une mesure et et sur une loi, un texte de loi sur laquelle on travaille ans on a on a on aurait bien eu le temps de travailler sur la question des seniors au travail hé bien on ne l'a pas fait, et aujourd'hui on nous propose un index seniors qui répond, pas du tout à la question, mais mes collègues l'ont fait et puis tout à l'heure. Eh bien la majorité ou demain la majorité sénatoriale nous proposera elle aussi des mesures qui aurait bien mieux trouver leur place dans les années précédentes. Merci. Monsieur temps de viande n'est pas là je passe la parole à Gisèle Jourda pour le 1034. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je suis toujours surprise. Qu'on aborde la question du recul de l'âge légal de départ à la retraite sans prendre des mesures d'envergure pour résoudre le résoudre la question de l'emploi des seniors.

ce devrait être pourtant la clé de voûte d'une réforme ambitieuse des retraites parce qu'elle répond à l'urgence sociale du travail et de l'emploi mais qu'elle répond également aux enjeux budgétaires qui vous inquiète tant chers collègues une réforme ambitieuse passe par des mesures d'envergure des mesures d'envergure pour mettre un terme à ce chiffre cruel à 60 61 ans, une personne sur 4 est inactive ou au chômage. Des mesures d'envergure pour mettre un terme à cette injustice car dans ces données. Les femmes sont particulièrement surreprésentés. Des mesures d'envergure, pas à la création d'un index, comment pouvez-vous croire une seule seconde que la solution passera simplement par la responsabilisation des entreprises, pas d'obligations. Pas de sanctions rien mais regardez les études et les chiffres de l'Unédic, Monsieur le Ministre déjà votre pari du retour mécanique à l'emploi, il concerne le plus souvent les seniors les mieux mieux insérés tels que les cadres ou les professions intermédiaires ensuite les répercussions de la réforme de 2010 qui décaler l'âge de départ à la retraite de 60 à 62 ans sont terribles. Ce sont 100.000 allocataires supplémentaires âgé de 60 ans et plus, entre 2010 et 2022. Alors conséquences pour l'assurance chômage. Au total, les dépenses d'indemnisation des plus de 55 ans ont augmenté de 38% depuis 2010 et comme la réforme de l'assurance chômage est venu modifier les règles d'indemnisation des seniors, des seniors, pardon. La seule chose finalement que vous avez à leur offrir ce n'est pas le le maintiennent à l'emploi, c'est la précarité, avec pour seul filet de sécurité le le RSA et ce serait là une réforme de gauche telle que vous l'infirmier ce matin votre argumentation de la Chine. Merci. D'une réforme des retraites ne tient plus. Mais c'est peut-être là votre objectif. C'est terminé donc. Mais ça va bien se passer, ne vous énervez pas alors.

Mes chers collègues. L'article 2 instaurant un index dits seniors constituent bien sûr un cavalier social il ne relève pas du financement de la Sécurité sociale, mais d'une loi travail en faveur de l'emploi des salariés âgés. L'affectation. Des pénalités relative à la non production. Tu dis index senior. Affectation au financement de l'équilibre de la branche vieillesse de la Sécurité sociale. Outre qu'il soit extrêmement choquant. Que plus la loi est respectée, moi on dispose de moyens pour équilibrer une branche essentielle de notre système de sécurité sociale, c'est quand même un paradoxe, vous en conviendrez. Mais surtout, mais surtout en droit. Il contrevient gravement. Au principe d'universalité budgétaire qui est l'un des 5 grands principes budgétaires des finances publiques en France le principe d'annualité principe d'unité budgétaire principe de spécialité budgétaire principe de sincérité budgétaire et donc principe d'universalité. Il s'agit d'une règle fondamentale du droit budgétaire. Universalité implique le rassemblement dans un document unique en une seule masse de l'ensemble des recettes brutes sur laquelle doit s'imputer l'ensemble des dépenses brutes. C'est donc un motif. Juridique totalement suffisant pour refuser cet article de et c'est la raison pour laquelle je vous invite à voter la suppression de cet article. Merci madame Lubin. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, j'ai entendu. Votre intervention tout à l'heure. Et à la fin j'ai entendu que nous allions débattre prochainement d'une loi travail. J'ai entendu que vous lanciez quelques pistes qui peuvent être intéressantes. Et notamment. Des des des choses qui ont existé hein, moi je ne me souviens nous avons tous connu une époque où. Un senior pouvait reprendre un emploi avec un complément de d'allocation du pôle emploi. des choses intéressantes qui ont été. Et les préretraites progressives qui ont été abandonnées petit à petit, donc tout ça ça peut franchement être intéressant. bon moi j'attends cette cette loi travail en espérant qu'. Il y aura vraiment des choses. Que l'on pourra discuter. Mais la seule question que j'ai et qui m'amène effectivement à vouloir supprimer cet article c'est pourquoi n'avez-vous pas mis cette loi travail avant la loi de finances de la Sécurité sociale rectificative pour allonger. La durée de cotisation. Enfin ça paraît d'une logique. Absolue. Et nous sommes quand même un petit peu inquiet, toujours beaucoup d'espoir hein. Dans la parole publique et donc je compte sur le gouvernement pour que cette loi travailler du contenu mais quand je vois ce qui s'est fait sur. L'assurance chômage et le fait que vous avez trouvé le moyen de réduire l'indemnisation des chômeurs de longue durée âgés de plus de 57 ans je crois. Alors qu'on sait très bien qu'à cet âge-là, la possibilité de retrouver un emploi de manière pérenne et quasiment nul Hervé il faut se, faut se dire les choses. Alors aujourd'hui ça se passe un peu mieux parce que les entreprises manquent de personnel. Bref, voilà, nous avons quand même quelques doutes sur la sincérité. N'est pas Houdini qui veut. Alors vous disiez pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est le magicien le plus célèbres de l'histoire. C'était un grand illusionniste. Et la création de cet indice seniors et finalement un tour de passe-passe un écran de fumée dans le seul but est de donner l'illusion que vous vous souciez hein t'soit peu du devenir et de la situation des salariés seniors qui vont pâtir du report de l'âge de départ à la retraite car c'est un fait votre réforme Osec aux objectifs purement comptable ne prend pas en compte une triste réalité, on l'a déjà dit à 60 trains, près d'une personne sur 3 n'est ni en emploi, ni à la retraite. La majorité d'entre elles sont en situation d'invalidité allocataires du RSA ou du chômage souvent elles vivent dans la précarité et avec l'âge. Rien ne s'avance, à 62 ans, c'est plus de 73% des salariés qui n'existe ce qui n'exerce plus d'activité. Cette réforme constitue donc un sas de précarité, inacceptable, face à cela, votre sur votre solution un index seniors qui rend obligatoire pour les entreprises d'une certaine taille. La publication d'indicateurs tels que le recrutement ou le maintien d'emplois. Une véritable révolution quand on sait que la non-publication n'entraînera pas ou peu de sanctions en d'autres termes, cette situation ne changera rien car les entreprises ne seront pas contraints d'embaucher davantage de seniors cette mesurette est une preuve de plus que cette réforme ménages et les entreprises au détriment des salariés vous cédez en effet à la loi des marchés vous succomber à la fascination d'un capitalisme financier qui broie les femmes et les hommes au service de l'intérêt des plus. Vous confondez leur travail et exploitation justice sociale et servilité face aux grands actionnaires à qui vous ne cessez de de donner des gages votre récit, elle n'est ni juste ni progressiste. Et maintenant le 1242 Madame Jasmin. Merci monsieur le président, c'est l'opacité. Monsieur le Ministre, c'est l'opacité l'index senior. C'est une forme de maltraitance maltraitance institutionnelle sur les personnes âgées. Moi, je demande de supprimer cet article parce que ce n'est pas normal que vous puissiez proposer de telles mesures. Au moment même où on a des absences d'analyse d'ergonomie dans les différentes entreprises. Des conditions de travail sont de plus en plus déplorable. Absence de contrôle des documents uniques et d'amélioration des conditions de travail. Absence du nombre d'inspecteurs du travail. Absence du nombre de médecins du travail. Défaut d'évaluation des différents risques dans les entreprises et concernant la la pénibilité bien vous en avez réduit, absence de transparence sur les revenus et les indicateurs de bien-. Être au travail. Alors à cet âge. Beaucoup de personnes ne sont pas en capacité de répondre à tout ce que vous voulez vous voulez leur proposer le nombre de congés de maladie dans cette tranche d'Assas été évoquée par d'autres collègues avant moi et particulièrement en outre-mer. Il est urgent de prendre des mesures mais pour les jeunes. Pour les jeunes parce que ce sont les jeunes qui sont au chômage, beaucoup de la personne de l'âge que vous souhaitez mettre au travail. Hé bien sont déjà cassés sont malades sont en longue maladie. Alors moi je veux vraiment qu'on passe du temps mais du temps pour les jeunes parce qu'ils ont besoin de travailler, il est nécessaire de supprimer cette Asics et de revoir l'ensemble de votre copie, merci. Merci monsieur Montaugé pour le 1285. Moi me questionne sur ses effets bénéfiques réel bon indéniablement. L'emploi des, des personnes de plus de 50 et 60 ans, est un véritable enjeu de société. Mais moi il me semble c'est partagé sur les bancs de mon groupe. Que cela devrait faire l'objet d'une loi ordinaire spécifique. Le taux d'emploi les réseaux. Le taux d'emploi des 60 65 ans, il est seulement de 56%, ce contre 80% pour les 25 49 selon les les chiffres du ministère du Travail. Alors tout ça d'abord du fait du chômage mais aussi parce que ces personnes sont souvent touchés par des une validité ou qu'elles sont devenues inactives et comme notre taux d'emploi des seniors est inférieur à celui de la moyenne européenne. De l'Union européenne à la question du maintien de l'emploi des seniors ne doit pas se poser sous l'angle simplement. De l'index me semble-t-il. De surcroît, l'index non contraignant et sans sanction ne peut porter d'objectifs concrets. Moi, je en suis convaincu. Cet index n'aura aucun effet sur les licenciements que subissent les salariés de plus de 55 ans qui sont souvent les premiers concernés par les plans sociaux le sait me fait cet index senior n'a rien à voir avec le financement rectificative du budget de la Sécurité sociale, c'est un cavalier législatif qui cache la nécessité d'une véritable loi travail. Sur l'emploi des salariés de plus de 55 ans. Ces personnes ne peut être considéré comme la simple variable d'ajustement de l'index leur emploi nécessite des mesures à la hauteur, surtout s'ils doivent travailler 2 ans de plus. Donc c'est un traitant d'abord de sujets comme celui-là, un sujet de de sociétés d'une certaine manière que vous auriez dû construire votre démarche au bénéfice de tous les les Français là aussi, comme sur l'énergie. On met la charrue avant les boeufs. Voilà on traite des mesures budgétaires avant de traiter les questions de fond politique qui intéresse le contrat social dans son ensemble, c'est tout à fait regrettable et inefficace. Merci Monsieur Montaugé pour le 1321. Madame Préville. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord sur la forme, l'article 2 instaurant un index dit senior ne relève pas du financement de la Sécurité sociale, mais d'une loi travail en faveur de l'emploi des salariés âgés. Ensuite, sur le fond dans cet article de la seule obligation c'est la publication de chiffres, soit le taux des salariés âgés dans une entreprise, et les seules sanctions concerneraient la non-publication de ces chiffres de ses taux. Autrement dit, il n'y a pas d'objectif réel ni de levier pour faire notablement évolué l'emploi des seniors. Cela s'apparente à ce qu'on appelle les engagements volontaires et on sait très bien le peu d'efficacité qu'on ses engagements volontaires. Je voulais attirer aussi votre attention sur une donnée les 2 tiers des licenciements sont subies par des salariés de plus de 55 ans. Voilà une réalité particulièrement cruel et rude 2 tiers. C'est colossal. Conséquence, 1,4 millions de personnes âgées de 53 69 ans ne perçoivent ni revenu ni pension de retraite. Certains d'ailleurs ne demanderont même pas le RSA par dignité, voyez-vous, tout simplement, est ce que, ce qui explique très certainement le non-recours aux droits. Résultat, une précarité grandissante, aggravée par les nouvelles dispositions de votre réforme récente de l'indemnisation chômage. Vous n'avez très clairement pas la bonne solution. Peut être faudrait-il commencer par valoriser toute la richesse d'expérience, de savoir du savoir-faire de savoir être des seniors. Oui, de remettre à l'honneur l'expérience tant de gâchis ont été faits dans la matière. Mais nous vivons dans un monde qui place l'innovation comme valeur cardinale mot magique qui écrase tout. Pour améliorer la situation des seniors, il faudrait penser différemment.

Merci Monsieur le Président aucune raison de figurer dans le PLFSS. Et que il relève bien entendu de la loi ordinaire. On sait aussi que le taux d'emploi en France des seniors est moins élevé que dans le reste. De l'Europe cette fait également. Avéré Vous avez dans cette loi, Monsieur le Ministre fait un objectif de publication avec cet indicateur est absolument pas un objectif de absolument Par ailleurs on sait également que le seuil qui est retenue n'est pas le bon parce qu'il ne concerne pas non plus assez de, de salariés. Je vous rappelle par ailleurs que la création d'un index sur l'égalité femmes-hommes au sein de l'entreprise par la loi de 2000 litres de 2019 sur l'avenir professionnel n'a eu aucun aucun impact sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes parce que. Justement, cet indicateur était lui aussi dépourvu d'obligation de résultat. Comment croire donc une mesure qui n'a pas fonctionné dans le passé pourrait désormais le faire par le simple fait de votre affirmation. Pourtant. Nous sommes au coeur de cette réforme, puisque on sait très bien que une augmentation du taux d'activité du taux d'emploi des 55 64 ans permettrait justement d'équilibrer l'ensemble du système. Mais ce n'est pas ce que vous recherchez. À vrai dire, vous êtes toujours dans la contrainte et non dans la proposition. D'autres mesures sont possibles. D'autres mesures sont pensable le déplafonnement du compte personnel de formation des travailleurs, la création d'un droit à un rendez-vous professionnel à 45 ans par exemple pour prévoir un conseil dans l'évolution professionnelle, un bilan de compétences, la formation continue. Autant de mesures que vous n'envisageait pas d'où cet amendement de suppression. Merci Martine Filleul n'est pas là donc je passe la parole à Joël Bigot pour le 197. Merci monsieur le président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet article 2 instaure une obligation de publication d'un index seniors pour les entreprises de plus de 50 salariés. Une nouvelle fois le gouvernement mise sur la bonne volonté des entreprises les codes de bonne conduite. Le nez mais chaîne sont désillusion auquel seul le gouvernement croate encore pour améliorer la situation des travailleurs seniors. En effet, cet article ne prévoit aucun moyen de contraindre les entreprises à un seuil minimum. D'emploi des seniors, pas même une contrepartie permettant d'inciter réellement les employeurs. Monsieur le Ministre, vous vous devez de proposer des mesures efficaces et non des mesures cosmétiques, alors que vous vous apprêtez à précariser encore un peu plus cette catégorie des de travailleurs déjà fragilisé. La question est fondamentale, une augmentation de 10 points du taux d'emploi des seniors augmenterait de près de 10 milliards les recettes. Cette question ne peut être abordé sur un coin de table sans concertation avec les syndicats. La réflexion de s'inscrire dans un projet dans un projet global sur le travail. Enfin cet article comme d'autres dans votre projet mérite mieux qu'une procédure accélérée mérite mieux qu'a raccourci démocratique en aucun cas, cette question ne touche au financement de la Sécurité sociale et justifie les les l'utilisation de la procédure du PLFSS. R comme cela a déjà été dit par mes collègues c'est l'avis du Conseil d'État que vous avez choisi d'ignorer ce sera sans doute l'avis du Conseil constitutionnel. Monsieur le Ministre, non content de de détourner une procédure de rééquilibrage du financement de la Sécurité sociale pour une réforme d'ampleur. Vous manifestez votre désintérêt pour la situation précaire des travailleurs seniors pour toutes ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, de supprimer cet index aussi in efficient qu'inefficace. Merci et maintenant pour le 1627 Madame Toumi rôle. Merci monsieur le président. L'index senior créée par cet article de n'a aucune valeur de contrainte aucune pénalité financière si l'on ne respecte pas ce fameux Index. L'emploi des seniors est certes insuffisant, 53% en France qu'on ne sont ni pour 100 en Allemagne ou en Suède. Et si on regarde de près les 60 64 ans, c'est à peine 36% des gens qui sont employés en reculant l'âge de départ de 60 à 62 ans par la réforme Woerth de 2010 on a créé 100.000 chômeurs de plus qu'en sera-t-il en la retardant à 64 ans. 90.010 la Darès et si on compte ce que Marine Lienemann appelle la zone grise, c'est-à-dire les seniors qui sont au chômage Anne ALD. En invalidité ou au RSA. Alors l'OFCE parle de 300.000 personnes. Quel sera le coût social, Monsieur le Ministre, dites-nous le et comment vivrons ces personnes ce qui est encore plus important. Le rapport de l'Unédic. Paris le 1er mars 2023 montre un pic de rupture. Conventionnelle quand on approche de l'âge légal de la retraite. L'arme de la rupture conventionnelle collective a été parfaitement comprise par les grandes entreprises qui en font un mode banal de gestion précarisant les salariés durcissant les conditions de travail et sacrifiant la santé et la sécurité des travailleurs. C'est donc un index inutile qui n'oblige à en rien les entreprises. Tout comme est inutile, l'index de l'égalité homme-femme qui n'a pas lui non plus de sanctions financières et qui n'a rien changé l'index senior ne changera rien non plus. Il faut donc supprimer cet article. Merci. Madame Meunier. N'est pas là madame. Moi non plus donc je passe maintenant la parole à monsieur le comte. Ou le 1698. Monsieur le président. Monsieur le Ministre, chers collègues. Un chiffre, un chiffre. Assez terribles. 55%. Des Français valident un trimestres de l'année de la liquidation de de leur retraite. Alors bien entendu, si. Ils ne peuvent la liquider que 2 ans après, la situation sera encore pire. Pourtant. Nous n'avons eu aucune réponse Monsieur le Ministre aux questions posées sur le coup. En matière. D'allocations chômage et de RSA que cette situation allait faire peser. Sur des personnes qui seront encore plus précarisés qu'aujourd'hui. Des estimations sont de 5 milliards d'euros. À quoi bon faire des prétendues économies si c'est pour précariser et engendrer de telles dépenses. Enfin, nous avons entendu les arguments de de de Vincent Eblé, j'aurais souhaité que notre rapporteur nous disent puisque finalement. Alloué. À la CNAV, le bénéfice des amendes. Liées à la non-. Publication de l'index senior relève. D'une, d'un détournement complet des lois relatives au au financement de la Sécurité sociale puisque c'est ce qui permet de prétendre aujourd'hui qu'on peut l'intégrer dans le. Alors parce que. Ce dispositif. N'est absolument pas efficace parce qu'il n'a pas sa place dans une loi, nous proposons de supprimer cet cet article qui n'a aucune aucune aucune efficacité par rapport au but poursuivi. Merci. Monsieur Todeschini Jomier ne sont pas là le président Kader. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Tout à l'heure j'ai évoqué l'article. 1 bis en l'appelant article E. Macron là c'est plutôt l'amendement ou l'article. En l'occurrence l'article Roux de Bézieux. Nous sommes. Finalement, face à une démarche.

Je vous cache pas que, en tant que ministre de la ville. Fin 2007 ou début 2017 je crois. J'avais porté cette idée avec ma collègue ministre du Travail de l'époque en disant mais. Il faut que, en matière de diversité sociale. Les entreprises qui ne jouent pas le jeu puisse être repéré. Et mise non pas à l'index, sans jeu de mot mais mise devant leurs responsabilités. Chers collègues, ça n'a pas marché. Je le dis, ça n'a pas marché parce que c'est pas comme ça que nous fonctionnons dans notre pays dans les pays anglo-saxons, ça peut marcher. Mais pas dans un pays comme la France. Moralité, j'ai regardé le, l'exposé des motifs. Monsieur le ministre et notamment la première phrase les crises motif issus du texte initial. Afin de faire de l'emploi des seniors, une priorité des entreprises le présent article prévoit la création d'un index senior qui a pour objectif d'objectiver la place des seniors en entreprise d'assurer la transparence en matière de gestion des âges et de valoriser les bonnes pratiques en la matière. Très honnêtement. C'est du violon quoi disons-le en entre nous. C'est de la bonne intention qui n'est pas à la hauteur de l'enjeu. L'emploi des seniors dans notre pays est très faible, trop faible et ce n'est pas votre index. Monsieur le Ministre, qui permettra de régler la situation. Merci la parole à monsieur Assouline pour le 1851. Oui. Quel dommage. Ça a été souligné par plusieurs de nos collègues. Quel dommage parce que c'est un vrai grand sujet qui ait jamais abordé à la hauteur de l'enjeu de l'enjeu, y compris de prospective parce que là il y a. Il y a du débat avoir. On est dans une société. Où effectivement. L'espérance de vie augmente. Et de l'autre côté. Le marché du travail, rétrécit en classe d'âge. Aujourd'hui les entreprises. À partir de 50 ans, considère qu'on est plus du tout assez productifs. Puisque c'est maintenant le seul étalon sur lesquels on fonctionne pour toujours faire plus de bénéfices, quelles que soient les vies qu'on broie ou. Les dégâts que l'on cause sur le plan social mais c'est un fait. C'est pas la peine je sais bien. La droite elle a ses atavismes mais ouvrez les yeux sur ce qui est une réalité. Or aujourd'hui nous dire qu'un index de ce type va faire quelque chose alors que s'il y a un domaine où nous avons essayé d'avancer parce que il y a des sanctions à la clé. L'emploi des personnes en situation de handicap. Seulement 30% des entreprises respectent les obligations de 6% de la masse salariale. C'est-à-dire que malgré. Le fait que on peut dire qu'il y a eu des avancées en terme de conviction de l'opinion en termes. De sanctions. Malgré cela, même pas un tiers des entreprises respect et là on nous ferait croire que parce que il y aurait une publicité. Qui ne sert qu'à justifier effectivement. Le le fait de de d'éviter qu'on dise que c'est un cavalier mais c'est un cavalier et je veux redire ici que Monsieur le Ministre on vous lâchera pas car il n'y a aucune raison pour la transparence de nos débats, de ne pas nous fournir la note du Conseil d'État qui dit que c'est un cavalier.

Je suis pas une spécialiste de l'emploi des seniors mais. Je en ce qui concerne l'emploi des femmes. Je j'ai la modestie de penser que ça fait quelques années que que je m'y penche et que je travaille dessus, et je sais que les index. C'est ce qui permet d'objectiver. Des réalités souvent invisibles dissimulés ou. Masqué par des arguties, des explications relativiste les données objectives, donc je suis plutôt a priori favorable à ce qu'on mette des index partout à chaque fois qu'on peut mesurer ce qui doit être mesurée, parce que ce n'est pas suffisamment visible. Pour autant, je ne considère pas que les index sont un outil de politique publique les index sont ce sur quoi on va pouvoir fonder. Des politiques publiques des politiques de l'emploi des sanctions ou éventuellement des incitations,

La l'index sur l'emploi des seniors. C'est pas tu fais la même histoire que pour les femmes hein on va pas calquer exactement l'index égalité femmes-hommes. Pour le faire sur l'index seniors c'est d'autres paramètres et en plus sur l'index égalité femmes-hommes on connaît les billets et les insuffisances de l'index, comment vous allez croiser les deux par exemple. Pour le choc pour les femmes. Seniors. On sait qu'il y a une prévalence du temps partiel. Est ce que le dos partielle des femmes va être considéré comme étant de l'emploi de seniors. Et est-ce qu'on va ainsi renforcer le temps partiel. Il y a toute une série d'interrogations qui aurait mérité. Si nous avions eu un projet de loi normal en fait pas un PLFSS avec un, un raccord ah rapprochement in-extremis de cet article dans. La loi retraites que on puisse travailler finement pour que. L'index égalité femmes-hommes on en tire le pardon président oh excusez-moi j'avais pas vu, je regardais le ministre en espérant qu'ils me regardent et donc j'ai, je, j'ai oublié de regarder le compteur je reviendrai.

Oui merci puisque Laurence Rossignol a pas pu finir. Ben moi je, je vais un petit peu reprendre un petit peu pareil. Un index si vous voulez un index les indicateurs qu'on va choisir dans l'index seront pertinent et donc efficaces que si ils ne commence par. Un diagnostic partagé de ce qu'il fait les discriminations. On prend les femmes effectivement quand vous partez de plus de 20% de discrimination. La part prise par le temps partiel, souvent subi quelques quelques fois je mets entre guillemets choisies effectivement est la première cause de l'écart. La 2ème cause c'est ce sont les secteurs féminin qui pour des raisons diverses, on y reviendra pour la pénibilité. Sont structurellement. Moins rémunéré que les secteurs dits masculins ça recoupe l'industrie, les services

et c'est la par la la plus petite, elle est importante, c'est à peu près 6% si je crois si 7% j'ai pas mis mon truc. Et donc. Effectivement, c'est celle que traque l'index et quand l'index retraité. Tracter à travers quand même des choses comme la promotion l'augmentation individuelle, qui sont il y a pas là par exemple la formation, bref ce. Alors pour terminer pour les seniors c'est pareil les seniors. Si vous commencez par par dire que. Le fait que 11% des retraités étaient au chômage avant si vous traitez pas de travail. L'intensification du travail qui les exclut si vous. Ne traitez pas les contraintes de rythme de travail, donc si vous ne changez pas de travail et tenez compte par exemple qu'ils ont besoin d'anticipation qu'ils ont besoin de transmettre qu'ils ont besoin de se former, vous pouvez mais pourrait mettre n'importe quel index ça changera rien à la réalité de la discrimination. Que je vais soumettre aux voix, y a-t-il des explications. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi avis. De la commission d'abord. Merci, merci Monsieur le Président, vous m'avez. Fait peur j'ai cru qu'après 48 amendements identiques. Sur lesquels nos collègues ont pu s'exprimer, le rapporteur n'aurait pas quelques minutes à leur consacrer. En réponse, donc merci de vous être. Avoir remarqué cela. Alors oui j'ai remarqué qu'il y en avait deux 3 différents mais. Si vous voulez, j'en prends un au hasard et puis je regarde s'il est pas identique. D'accord. Bon. Voilà il y en a un qui est pas identique c'est Monsieur Jacques qui est repris d'ailleurs par quelqu'un d'autre et je l'ai pris en main, pourquoi parce que. Qui parle de quelque chose d'intéressant puisqu'il dit que les salariés de plus de 55 ans. Sont trop souvent une variable d'ajustement. Oui, nous le constatons et quand on va décaler l'âge ça va pas être les salariés de plus de 55 ans, ça va être après. voyez-vous c'est comme ça que ça se passe, c'est dans tous les pays étrangers, ils ont fait partout, ils ont augmenté l'âge partout il y a un emploi des seniors est beaucoup plus important que chez nous, c'est la raison pour laquelle NouvelAn prendre des mesures pour faire en sorte que on accompagne cette dimension autre qui fait qu'on travaille plus longtemps. Et d'ailleurs vous êtes tellement impatient de de d'appréhender les mesures qu'on vous propose à l'article 9 que je vois bien que vous traduisez votre impatience par une répétition des amendements. Il n'empêche que c'est une théorie qui ne vous a pas échappé. Puisque la réforme Touraine c'était bien un allongement de cette durée de travail, un passage de 41 ans et demi à 43 ans un peu différée. Puisque ce sont les générations d'après et que, qui sont celles de maintenant que l'on prend. Et pourquoi vous avez augmenté la durée de travail parce que vous avez constaté qu'en France nous ne produisions. Pas assez. 600. 680 heures de travail quand. À l'habitant, 800 en Allemagne, une balance commerciale complètement négatif. Nous ne produisons. Pas assez. C'est la raison pour laquelle il nous paraît tout à fait important de prendre les mesures nécessaires et d'accompagner accompagner le travail c'est mieux travailler prend en compte effectivement le bien-être et peut-être. Pas forcément faire. En 35 heures ce pour ce qu'on pourrait faire en 39 heures, ne l'oublions pas que mieux prendre en compte le travail c'est aussi peut-être réfléchir à tout ça, ça nous paraît important alors. Qu'est-ce que nous devions faire. Vous parlez d'une. Menace d'inconstitutionnalité. Sur cet article de oui oui oui ça nous a pas échappé. Ça n'avait pas échappé à nos administrateurs, on en a parlé bien avant de lire la note du Conseil constitutionnel qui reprend. Du Conseil d'État, excusez-moi. Merci de suivre du Conseil d'État qui reprend exactement ce que nous nous nous nous pensions. C'est la raison pour laquelle cet avis et est très clair et mais il y a aucun problème. Juste sur ce point.

Les présidents de commission savent bien ce que c'est ces notes confidentielles, moi j'en suis respectueux. Elles sont à la disposition de serre. C'est une personne dont les membres de l'annexe. Voilà et quand je suis interpellé par Cathy. Ah pour se. Elle est membre de l'annexe. Qu'est-ce que j'ai dit il y a je ne sais combien d'heures que j'ai été à disposition pour rencontrer celles et ceux qui, membre de l'Amex parce que la loi est ainsi faite, il y a une confidentialité j'y peux rien. Celles et ceux qui souhaitent. Voir avec moi cette note que je ne peux pas vous confier vous confier, vous pouvez prendre contact avec moi et c'est avec beaucoup. De convivialité que je vous la montrerai, ben vous devez savoir si vous vous êtes membre de la Mecque ou pas quand même. D'accord. Il vous appartiendra ensuite de voir comment vous en parlez à vos collègues s'est ainsi fait c'est ainsi fait de façon à ce que si vous en êtes d'accord, on en parle plus D'accord mais vous serez déçu parce que tout est écrit dans le monde et vous le savez très bien que. Vous verrez que il y a rien de neuf mais. S'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est le le le rapporteur continuer seul et qui ensuite on poursuivra la discussion. reviens j'en reviens à la position de la commission, une fois qu'on a dit ça. Nous avions 2 solutions d'accord soit dire c'est ce sera inconstitutionnelle hop on supprime comme vous le proposez cet article là mes chers collègues. Il y aurait pu rien sur l'emploi des seniors. Vous venez 48 fois. De 48 fois consécutive, nous dire que vous étiez interpellé par rapport à l'emploi des seniors qui ne figurait pas dans cette loi qui auraient dû figurer dans une loi travail ce que nous disons, les choses sont mis à l'envers, effectivement mais nous récupérons. D'accord. Cette dimension de l'employabilité des seniors en le remettant dans la loi. C'est la raison pour laquelle nous avons pas rejeter cet index et puis nous écoutons, nous avons consulté énormément ça fait vous savez, ça fait 4 ans quand même qu'un certain nombre d'entre nous se penche sur l'affaire. Donc les partenaires sociaux on les connaît bien, quand même, qu'est-ce qui nous ont dit les partenaires sociaux, notamment ceux de la CFDT. Nous sommes attachés à l'index ah quelque part on a écouté. Nous avons également des partenaires, il y a Olivier Henno, qui s'est penché Olivier Henno m'a dit ah moi je pense que l'index. C'est pas suffisant mais faudrait. Nous avons écouté nos partenaires pour faire en sorte plutôt que de rejeter d'un revers de main, prendre en compte cet index et trouver une disposition nous permettant d'inscrire une avancée. Dans la prise en compte de l'employabilité des seniors à travers le CDI seniors quand vous proposera tout à l'heure avec justement une exonération de cotisations famille pourquoi. Cotisations famille pourquoi parce que c'était dans la dimension d'un PLFSSR. Qu'une exonération exonération d'une cotisation chômage. Qu'il eut été plus judicieuse et hors PLFSS, vous le savez aussi bien que moi donc on a raccroché cette disposition pour faire en sorte que le gouvernement puisse prendre en compte cette dimension nouvelle qui sera monsieur le ministre. Et on se rejoint dans ce dispositif-là à discuter avec les partenaires sociaux. C'est une avancée, une proposition et ensuite les partenaires sociaux. Ils veulent ils veulent s'inscrire dans ses dimensions, ils nous l'ont demandé. C'est la raison pour laquelle nous avançons dans ce domaine-là et puis un point également particulier c'est que vous l'avez bien dit moi nous trouvons inacceptable inacceptable ces ces seniors qui se retrouvent au chômage ce n'est pas une variable d'ajustement. Si elle le peut, la raison pour laquelle il faut prendre un en compte un certain nombre de difficultés et UC. On sait que certains peuvent être usés par le travail. C'est la raison pour laquelle à travers l'article 9, on a une avancée considérable je ne peux pas entendent, permettez-moi de dire que on a écarté tous les facteurs de risque en dehors du c'est de paix non dans ces deux pays à 4 facteurs de risques ont été retenus, on peut mieux les identifier qui sont bien pris en compte dans le cas de la prévention dans le cadre derrière d'une, d'un travail à temps partiel partiel ou éventuellement aussi de la réparation par un agent anticipé de départ à la retraite mais dans les autres facteurs, notamment les facteurs ergonomique. Il est important de les prendre en compte, il y a une avancée qui a été fait dans le dispositif puisqu'on crée un fonds spécial, donc ils seront pris en compte et nous avons encore à faire avancer le dispositif car certes les âges d'invalidité d'incertitude. D'inaptitude au travail resteront à 62 ans mais par contre je pense que nous pouvons avancer. Et si vous êtes d'accord pour aller jusqu'à l'article 9. En évitant un certain nombre de monologue. Nous pourrons avancer pour faire en sorte que l'incapacité permanente prise en compte, en considération des 60 ans sans attendre 62 ans. Vous voyez ces avancées sociales. On les a annoncé les seniors les attendent, me semble-t-il et nous voulons des garanties me Monsieur le ministre. On espère nous donnera pour que ce soit inscrit dans la prochaine loi sociale, voilà comment nous avons. Envisagé les choses et nous avons même pousser. Encore plus loin puisque il y avait pas de prise en compte sur les l'exposition aux agents chimiques dangereux que nous réinscrivant dans les dispositifs pour qu'il ait à travers ce qui est proposé. La prévention de ces jeunes agents soient mieux prises en compte. Voilà ce que je souhait vous dire. Que notre ambition, c'est clair et ça a été dit par certains d'entre vous. On a besoin de prendre en compte de façon spécifique. L'emploi des jeunes, on a besoin de prendre en compte de façon spécifique. L'emploi des seniors. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans le cadre de cette suppression d'articles pour lequel, vous l'avez compris, je donnerai un avis défavorable. Merci monsieur le rapporteur. Et. Et l'avis de Monsieur le Ministre sur ces mêmes amendements. merci beaucoup monsieur le président, là l'avis du gouvernement évidemment défavorable à ces amendements de suppression j'ai premier bref tout à l'heure je je je vais l'être. De 2 cependant d'abord à écouter. Monsieur Assouline. Je ne vous ai pas interrompu. Quand vous avez partagé avec nous votre connaissance de l'entreprise et de l'économie donc et c'est moi, aller au bout. De de de cette explication. De l'avis du gouvernement. La première chose c'est que j'ai parfois entendu un certain nombre de justification autour de ces amendements. Qui me donner le sentiment qu'on cherchait toutes les bonnes raisons de le supprimer, je prends un seul exemple mais tout à l'heure monsieur Montaugé nous dit. dû vous devriez plutôt. Déplafonner les les points qu'on peut obtenir autour du CDP, ça tombe bien, c'est ce que nous faisons. Donc vous voterez. L'article 9 avec nous. Ne vous avez cité un certain nombre d'actions que nous mettons en oeuvre ou sur lesquels nous nous sommes engagés, comme l'a rappelé monsieur le rapporteur. Donc assumer de vouloir supprimer un outil qui va accompagner l'emploi des seniors sont nécessairement chercher des raisons qui n'en sont pas ou qui sont. Différentes de celles que nous avons mis dans le texte la la 2ème chose c'est vrai que l'Assemblée nationale a fait le choix et, et en particulier parce que un amendement portant le dispositif à trois pardon le seuil de déclenchement du dispositif de 350 salariés avaient été adoptés, a fait le choix de rejeter l'article et c'était pour moi une déception et j'ai vu que c'était c'est toujours été partagée puisque le lendemain de cette suppression votre commission des affaires sociales auditionné les organisations syndicales et monsieur Ricordeau qui est secrétaire national de la CFDT. A dit qu'il regrettait la suppression de l'index, a dit qu'il considérait que l'emploi des seniors ne progressera qu'avec le dialogue social et qu'Supprimons l'index. L'Assemblée nationale, avait pris le chemin inverse et Lise ça notamment parce qu'on renvoie la définition des critères et la possibilité de leur adaptation au dialogue social interprofessionnel pour le décret. Petite question des critères et au dialogue social de branche pour l'adaptation. C'est pour ça que nous avons un index qui renvoie à à ce rôle des partenaires sociaux pour définir les bons indicateurs et la bonne mise en oeuvre. Donc je m'arrête là mais évidemment pour ces 2 raisons complémentaires en plus de ce que j'ai dit, l'avis est défavorable. Bien donc nous avons un double avis défavorable de la Commission et du ministre-sur ces amendements de suppression avant de les soumettre aux voix j'ai des demandes d'explications de vote. Madame Carlotti. Monsieur le Président. Moi je souhaite soutenir les amendements de suppression de cet article de car nous ne devrions même pas en discuter, ça a été très bien dit par ma collègue tout à l'heure. Hé oui d'après la vie. Du Conseil d'État, il s'agirait d'un cavalier social qui pourrait même être inconstitutionnelle. Alors tout à l'heure, la droite n'a pas voulu que cet article soit renvoyé en commission mais c'est vraiment fort dommage surtout quand je viens d'un temps le président de la commission n'aurait pu ensembles remette tout à plat. Faire de vraies propositions pour le maintien en emploi des seniors pour envisager des procédures de reconversion.

que le projet de loi sur le travail en sera l'occasion puis du coup en fait au lieu de ça au lieu d'avoir ce débat complet, finalement on tourne autour de la mesure gadget de de l'index senior. Non c'est pas normal c'est pas sérieux c'est pas suffisant, c'est pas comme ça qu'on devrait répondre à la situation des seniors. On demande donc et je soutiens le retrait de cet article, et même je soutiens Monsieur le Ministre, le, le retrait de votre réforme car vous voyons vous voyez bien qu'au fur à mesure, elle n'est pas abouti. Monsieur Kerrouche. Merci monsieur le président. Juste pour répondre à, à monsieur le le rapporteur, à chaque fois on nous parle des mesures d'âge et notamment des mesures d'âge dans les autres pays européens. Mais vous le savez très bien et plusieurs études l'ont montré d'abord faudrait-il pouvoir comparer exactement les différents systèmes et ce n'est pas aussi simple que ça. Bruno Palier là l'a bien montré. Ensuite vous comparez aussi uniquement des âges. Je vous rappelle par exemple que au Danemark CERC on part à la retraite plus tard mais pendant 6 ans on peut avoir ses études payés pour un étudiant jusqu'à 840 euros par mois et donc il faut avoir l'ensemble des éléments de de comparaison. Par ailleurs. Monsieur le rapporteur, j'ai cru comprendre que vous étiez un peu agacé par la répercuter la répétition des, des arguments qui, qui sont les nôtres mais je ne comprends pas que vous soyez ennuyés. Je ne comprends pas que vous ne puissiez voir la violence que nous sommes que vous êtes en train de vouloir imposer à une partie de la population et vous étonnez que justement vis-à-vis de cette violence. Nous ne soit nous ne soyons pas obligés de répéter les mêmes arguments parce que nous ne discutons pas dans le vide ces mesures, elles vont avoir des effets et des effets dans les vies et dans les chairs. Et bien entendu il faut continuer à marteler ses arguments pour peut être enfin que vous puissiez les accepter les comprendre. Merci, monsieur le Président, je vous ai bien écouté Monsieur le Ministre, mais j'ai aussi écouté toutes les interventions qui vous ont précédés et ce qui remonte, c'est quand même que ce cet index seniors c'est le symptôme du manque d'anticipation, voire d'improvisation de ce texte puisque si cet index et dans ce texte, c'est parce que la question de l'emploi des seniors en réalité clé dans la réforme mais pour ponts vous nous proposez c'est vous nous proposez que ce formulaire, un formulaire qui serait le préalable à une politique ambitieuse que vous nous annoncerez plus tard et dont nous n'avons pour l'instant aucune piste concrète et on devrait commencer par voter cet index et vous faire confiance pour la suite et on va se l'avouer. C'est compliqué de vous faire confiance en ce moment, Monsieur le Ministre, après beaucoup d'enfumage. Mais c'est encore plus compliqué, vous faire confiance quand on connaît votre pudeur lorsqu'il s'agit d'imposer la moindre mesure aux entreprises. On l'a encore vu récemment avec le panier anti-inflation et pourtant il va falloir agir les probabilités de retour à l'emploi, après 50 ans sont très faibles et français considèrent qu'avoir plus de 55 ans est le 1er motif de rejet lors des embauches à compétences égales en 2021. Les testings réalisés par la Darès monte une personne ayant entre 48 et 55 ans à 3 fois moins de chances d'être appelé pour un entretien qu'un qu'd'une personne entre 23 et 30 ans selon la DG trésor, la part des chômeurs à de longue durée, plus d'un an chez les chômeurs de plus de 55 ans en 2018 2 et de 60% le report de l'âge d'ouverture des droits à 65 ans va donc aggraver dramatiquement ce sas de précarité des catégories populaires et le chômage des seniors votre réforme est donc brutale et injuste. Merci monsieur le président. Évidemment je vais voter les articles de suppression de l'article de. Tout d'abord parce que je crois que comme beaucoup d'entre nous dans cette assemblée, je suis attaché au respect de la constitution hein. Je ne vois pas bien l'intérêt de voter une mesure quand nous savons puisque j'ai lu le monde même si je suis très triste de ne pas avoir pu lire la vie mais j'ai lu le monde et il semble que cette, cette disposition de la loi sera censuré. Donc je ne comprends pas bien à quoi ça sert qu'on la vote surtout au Sénat, nous qui sommes attachés au respect de la Constitution. Ensuite parce que je suis aussi attachée au parlementarisme et à respecter le choix de l'Assemblée. Lionel qui a retiré cet article alors même que la droite et la la majorité présidentielle se plaignait que les débats n'aient pas pu avoir lieu et quand ils ont lieu, et bien ça ne les intéresse pas. Sur le fond. On a eu l'occasion de le dire et et j'ai bien conscience qu'on l'a dit qu'on l'a dit de nombreuses fois. Mais néanmoins, c'est vrai. Cet article ne va servir à absolument rien. C'est pour ça qu'il est anticonstitutionnel. S'il était constitutionnelle, ce serait parce qu'il aurait un impact sur les finances publiques cette année et donc il servait à amener des cotisations sociales par exemple. Donc moi ma question c'est aussi à tous mes collègues qui vont voter contre ces amendements et donc ils veulent garder l'index des seniors dans le texte de loi elle ce qui vont aussi voter pour tous nos amendements qui consiste à faire que cet index serve à quelque chose qui soit associée à des sanctions qu'ils permettent de faire quelque chose en réalité qui va permettent d'avoir un impact positif sur les finances publiques parce que sinon, à quoi ça sert de voter en faveur d'un truc qui ne sert absolument à rien et de rejeter toutes les propositions, vous allez voir, parce que nous sommes quand même constructif. Nous en avons beaucoup toutes les propositions qui consiste à faire que cet article 2 est un impact. Merci, monsieur le Président alors. Tout d'abord je voulais vraiment remercier Monsieur Savary. Parce que vraiment pouvoir nous permettre de consulter. Les notes du Conseil constitutionnel. C'est une avancée quand si d'État excusez-moi, c'est une avancée considérable considérable Monsieur Savary. Depuis, on a perdu beaucoup de temps autour de ça depuis jeudi. Nous aurions pu les consulter. Nos nos nos nos nos nos non c'était se créer. Il n'y avait que le président de l'Amex qui pouvait les avoir. Nous ne pouvions pas les avoir. Nous ne nous n'avions pas le droit de les consulter tout à l'heure quand j'ai causé la présidente de la commission, madame Deroche m'a dit qu'elles étaient secrètes ses notes et que je ne pouvais pas en disposer. Si donc bon, en tous les cas il y a une avancée considérable et nous la prenons et nous sommes sommes contents Monsieur Savary et je vais venir, je vais venir, je vais venir Monsieur Savary. On va passer une petite nuit ensemble. On va regarder les choses avec les collègues. Et puis on va consulter ses notes secrètes qui de toute façon ne devrait pas l'être, de toute façon. Elle ne devrait pas être secrète mais bon. On va venir Monsieur Savary ne vous inquiétez pas, on est content. Alors évidemment nous allons aussi voté la suppression de l'article de. Alors si vous préférez évidemment pas une nuit, une journée peut être hein, hein. D'abord parce qu'il est un cavalier social et que nous souhaitons pour notre part, ça a été dit une véritable loi travail la réalité. Monsieur le Ministre, c'est votre gouvernement a une fois de plus répondu favorablement au MEDEF en refusant d'associer l'index senior à des sanctions financières. Aucun pouvoir de contrainte, donc aucun n'est fait. Voilà la réalité est là et donc nous voterons pour la suppression de l'article de. Merci monsieur le président. Mes chers collègues. Reconnaissons que cet article n'est pas le coeur de de cette réforme. Par contre, elle renvoie à ce qui est essentiel. Cette notion de travail travail des seniors et le vrai problème que nous avons en France par rapport aux autres pays, c'est effectivement le taux d'activité des seniors comme des jeunes. Donc la question c'est comment on augmente le taux d'activité en l'occurrence des seniors qui effectivement sont plus touchées par le chômage et souffrent d'une attitude bien française, qu'il faudra changer et dans le temps qu'ils se trouvent les plus souvent hé bien mis à la porte, notamment des grandes entreprises, lorsqu'il y a des plans sociaux. Ça c'est une réalité ça renvoie aux usages aux coutumes et l'État à travers les entreprises dont l'État encore des participations est loin de montrer l'exemple. Donc il y aura des choses à faire donc j'aurais presque pu reprendre, mot pour mot l'intervention du président rénale tout à l'heure. Le problème c'est qu'on a mis encore une fois les choses à l'envers. Et Monsieur le Ministre, monsieur Dussopt tout à l'heure nous disait qu'il y aurait une loi sur le travail sur l'insertion, la formation pas, nous n'avons-nous pas commencer par cela et moi je regrette fortement que cette partie ici de l'hémicycle, n'est pas suffisamment fait pression sur le gouvernement pour que ça passe d'abord sur le travail et qu'après on travaille. Tranquillement, sereinement. Sur les retraites parce que mettez-vous à la place des nombreux. Personnes qui travaillent moins, les plus grandes entreprises que les PME, les PMI et vous voyez tout j'imagine dans les tribunaux de commerce, de vos territoires augmenter. Eh bien les dossiers qui arrivent. Car il ne vous a pas échappé que nous vivons une période d'inflation, une période de de punir une période d'augmentation des prix de l'énergie et que ce Sarko trouve partout et que nous avons des entreprises qui vont faire faillite. Bah, mettez-vous simplement à la place des travailleurs et travailleuses pour reprendre une expression un peu plus âgés au-delà de 55 ans et ben ils peuvent être légitimement inquiets par cette réforme. Donc il faut pas s'étonner qu'il y ait beaucoup de monde dans la rue la semaine prochaine. Donc moi j'aurais vraiment souhaité parce que la fusée de cette réforme si on met les étages à l'envers, elle avait pas près de décoller. Donc moi je voterai cet article et la réforme on verra. Monsieur Breuiller. Merci monsieur le président, effectivement c'est toujours à l'envers. Un petit texte rectificatif pour une grande ambition, c'est quand même assez étonnant ce petit texte qui va quand même permettre à l'administration française de faire des exploits puisque les entreprises d'au moins 1000 salariés devront publier des indicateurs relatifs à l'emploi des salariés âgés dès le 1er novembre 2023 en France, nous allons aller vite et ils seront sanctionnés avant le 31 décembre 2023. C'est à cette condition là qu'il pourrait y avoir des recettes dont les annexes nous rappelle que compte tenu de la compatibilité des régimes de Sécurité sociale est enregistré en droits constatés, le produit d'une sanction juridiquement prononcées notifiées avant le 31 décembre 2023 sera rattaché à l'exercice Vraiment on malmène les entreprises dans ce pays en étant aussi sévère, on publie un index obligatoire au 1er novembre et on les sanctionnera, avant le 31 décembre. Plus sérieusement sur le fond de ce propos. Monsieur le rapporteur. Je voudrais vous dire une chose, moi je souhaite effectivement que nous améliorons les conditions de travail, les conditions de maintien dans l'emploi de tous les salariés pas jusqu'à 64 ans a en allongeant la durée du travail mais jusqu'à l'âge légal du travail et à partir de 55 ans où le taux d'emploi est très faible mais je ne veux pas le faire dans un texte qui est un texte dont l'objectif est de maintenir et de prolonger de 2 années de plus au travail. Je souhaite le faire dans une loi travail débattue et négociée avec les partenaires sociaux sur cet aspect là je sais que nous, nous rejoignons sur la volonté qu'il y ait débat. monsieur le président. Il faut une véritable loi travail votre gouvernement, Monsieur le ministre à supprimer les Chsct, la transparence est donc nécessaire. Une vraie loi travail pourrait nous permettent de mieux échanger dans cet hémicycle. n'aura aucun n'est pas réel dans les territoires d'outre-mer je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le répète, dans ce contexte d'inflation et de vie chère. Il faut de vraies mesures pour combattre le chômage et améliorer la qualité de vie, l'index senior ne peut en aucun cas être une vraie solution. Il faut une loi complète bien réfléchi partager avec les partenaires sociaux une loi-pertinente et bien pensé. Cet article doit être supprimé c'est un cavalier social limité injuste qui ne propose que des maltraitances envers les seniors démunis et déjà précaire. Merci. Merci donc nous en avons terminé avec les explications c'est pas à Madame Poncet Monge excusez-moi je ne vous avez vu. Oui. Oui, je voudrais dire à Alain Milon, que je suis sûr qu'il a tout compris mais que moi en général je réponds au rapporteur et au ministre hein donc c'est forcément après. Donc. Justement, vous avez dit monsieur le Ministre. Que cet index, c'est très bien, vous avez redécouvert le dialogue social, il sera discuté en interpro et par branche tant mieux et que les ouais sont des propositions il y a pas que la CFDT, toutes, elles ont toutes des propositions mais puisque souvent la CFDT. Je vous rappelle qu'elle est contre et qu'vous demande le retrait de cette loi. Moi j'ai. Si vous voulez ce qu'il faut comprendre c'est que cette loi s'applique dès septembre là donc elle va s'appliquer aux gens qui ont entre 58 59 60. 61 ans et de façon brutale et immédiate. C'est là où on va faire des économies qui va vous permettre d'être à 3% en 2027 pour. Pour mes Maestri. Alors aussi à partir de là si vous voulez. Il est bien certain que tout ce qu'on va dire sur l'index n'a pas de d'effet hein c'est. Sur cette population-là, c'est déjà trop tard et c'est pourtant elle elle qui qui sont sollicités. D'ici 2027. Et donc. Ce que je veux dire c'est que ben c'est ce que je disais tout à l'heure qu'en fait il faut changer le travail il y a pas que le taux d'emploi des seniors qui pose un problème, il y a celui des femmes. Il y a celui des jeunes il y a celui des seniors. Il y a celui des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez bien que ça vous nous avez promis une loi cette année ben l'index aurait pu en parler cette année Nancy les là c'est pour vous servir de caution à ce qu'on y compris la CFDT refuse, c'est-à-dire le l'ouverture le le décalage de l'ouverture des droits à la retraite. Monsieur Chantrel. Merci monsieur le le président. Monsieur le le le rapporteur Savary. Vous nous avez dit dans votre propos. Mais écoutez, les syndicats qui sont d'accord pour cet index et d'ailleurs ils ne sont pas unanimes sur le sujet mais vous ne les écoutez pas sur le retrait de la réforme. Alors que là pour le coup, ils sont unanimes, ils se mobilisent constamment depuis des semaines et des semaines et là par contre vous ne les écoutez pas donc c'est vraiment à deux vitesses est et il ne résoudra pas le problème. De l'emploi des seniors s'il est pas sorti de la moindre contrainte. Tous les ces indicateurs ils sont dénuées et vous le savez très bien de la moindre obligation ils sont complètement bidons. Ils permettent seulement aux entreprises qui attribue les labels de faire du profit et impose une couche de bureaucratie supplémentaire à toutes les autres. La vérité c'est que votre réforme va créer un sas de pauvreté pour les seniors. À 62 ans, 40% de ceux qui ne sont pas à la retraite ne travaille pas. parmi eux un tiers vivent sous le seuil de pauvreté votre réforme qui fut l'axe de départ justement à la retraite à 64 ans et violente et cruelle va accentuer cette cette pauvreté. D'après l'Observatoire français de des conjonctures économiques, qui est un observatoire sérieux. Elle se traduira justement par 277.000 chômeurs supplémentaires. 400.000 nouveaux arrêts de travail pour maladie professionnelle et 110.000 personnes de plus aux minima sociaux. Au bout du compte si vous voulez réellement faire quelque chose pour les seniors. Commencez par faire en sorte d'empêcher qu'ils soient licenciés. Et ensuite, lutter contre la discrimination à l'embauche qu'ils subissent. Comment faire, me demanderez-vous, hé bien en leur donnant des droits ainsi qu'aux syndicats afin qu'ils puissent se défendre. Le président rénale. C'est le rapport entre. Ce texte et puis l'année 2023. Du point de vue financier. Et budgétaire. Bon c'est tout ce que c'est faux et si. À la limite on voulait faire un effort, en se disant qu'il on y croit un instant bah il suffirait de se souvenir de ce qui nous a été expliqué, encore une fois récemment sur la réforme de la CVAE ou sur la réforme de la CVAE, un des sujets et de dire que si on veut allouer aux entreprises oh pardon aux collectivités. Ce qu'elle recevait avant. Il faut que les entreprises puissent conserver. Le juste comptage. De leurs salariés et le donner à l'administration. Hé bien on nous a dit à l'époque que c'était infaisable que les entreprises on ne pouvait plus dès l'instant où ont supprimé la CVAE leur demander cet effort de juste comptabiliser leur poste de travail et le donner à l'administration fiscale. C'était infaisable un truc basique ou basique et là on nous explique qu'on va appliquer un texte donc qui va s'appliquer début septembre. Où on va demander aux cons aux entreprises. L'air de rien, de remplir des fichiers pour le mois. De fin octobre et ensuite qu'on va s'ils ne se rendent pas, s'ils ne font pas les choses qu'on va les taxer tout ça dans la même année.

Ce matin encore le JDD nous annonce avec une nouvelle enquête d'opinion que seuls 32% des Français. Sont favorables à cette réforme. Et si l'on regarde les moins de 35 ans, c'est-à-dire ceux qui vont être et plus concerné 74% et ceux qui ne sont pas concernés, à 50%. Je sais pas si. On se rend compte du sujet. Nous sommes ici. En train de discuter d'une réforme dont on sait que 2 tiers des Français la rejettent que pourrait faire le gouvernement et d'ailleurs vous aussi à droite. Ben de discuter avec ceux qui sont opposés à la réforme nous. Qui représentons à peu près l'opinion de 2 tiers des Français pour voir comment on règle. Dans cette enceinte ce ce problème démocratique, c'est-à-dire que le gouvernement devrait être en train de voir comment dans ce débat il va amender regarder, écouter les arguments discuter avec nous. Or ce n'est pas du tout ce qui se passe. Même c'est l'inverse qui est en train de se passer dans cette enceinte. La seule chose qui va être discutée réellement. Entre le gouvernement et la majorité du Sénat. C'est comment la durcir encore plus. C'est-à-dire comment l'éloigner encore plus. Des Français qui la rejette. Comment la rendre encore plus brutale et vous pensez bien que quand on offre ce spectacle aux Français. Hé bien on renforce la crise démocratique et on ne fait le lit que d'une seule force politique, celle qui est contre la République.

Les amendements de suppression identiques que nous venons de débattre avec un double avis défavorable. De la commission et du gouvernement. Donc qui est pour ces amendements de suppression. Qui est contre. Qui s'abstient. Ils ne sont pas adoptés. Donc l'article 2 étant du coup maintenu, nous allons entrer dans le débat des amendements visant à améliorer cet article il y en a 145. Donc le premier et présenté par Madame Poncet mange c'est le 31 65. Oui, merci Monsieur le Président ma puisque nous avons l'index. Nous allons tout comme le rapporteur essayer de lui apporter tout le contenu et puis peut-être qu'à la fin comme ça on révisera notre position, c'est jamais donc. Écoutez bien tout ce qu'on propose nous pour que ça soit un outil réellement ambitieux et opérant. Capable d'avoir un impact sur l'emploi et sur la qualité de l'emploi et le travail de la formation des seniors. nous avons rappelé que 63% des salariés âgés de 44 à 55 ans, vous voyez c'est même avant les seniors en recherche d'emploi n'ont pas été sollicités par des recruteurs au cours des 6 derniers mois, contre 26% chez les 18 24 ans. De plus, la proportion des 55 64 ans, vous l'avez dit qu'. Est pas n'est pas satisfaisante qui occupe un emploi s'élève à 56%, moi j'aimerais bien les statistiques de 60 et 61 et 62 ans donc afin de pallier divers contournement du dispositif. Nous proposons une définition plus claire et plus précise non seulement du contenu des négociations. Vous avez parlé dialogue social, Monsieur le Ministre. Tant en interpro que en branche et que en entreprise en en en suivant la hiérarchie des sources qui est quand même. Très très importante ici. Donc compte tenu de l'urgence pour les seniors d'avoir non seulement un travail décent. Mais aussi une fin de carrière digne et pas finir. Dans le chômage dans dans les minima sociaux ou ou en en maladie dans un contexte de menace de l'âge de, de dépassement de l'âge de départ. Nous proposons que l'application de la Dex débute à partir du 1er mars 2024 a laissé à l'exception des entreprises de plus de 500 salariés, donc vous avez dit qu'ils ont tous dans le dans le GPEC et qui pourront commencer donc l'index en vigueur dès le 1er novembre 2023. Merci. Avis de la commission sur cet amendement. Oui effectivement, cet amendement propose un calendrier différent selon les textes de l'entreprise, puisqu'actuellement, ce sont celles plus de plus de 1000 qui doivent au 1er novembre. Publié le l'index. Sur. Des indicateurs qui ne sont pas encore défini puisqu'il y a pas eu les négociations de branche mais mais qui en attendant pour faire en sorte que le produit des pénalités puissent éventuellement être imputés sur l'exercice 2023. Ces modalités de prise en compte des indicateurs seraient. Proposés par décret en attendant. En attendant, effectivement cela. Alors si on descend à 500 là on, on est sûr. Parce que c'est encore plus compliqué qu'il n'est, n'y avait pas. Effectivement de pénalités qui rentre. En 2023, et puis également vous proposer. Vous proposez quoi. Une augmentation des pénalités. Voilà voilà. Excusez-moi, excusez-moi une augmentation des pénalités. Ah voyez-vous les pénalités qui sont proposées sont quand même significatif, c'est 1% de la masse salariale. Sachant que. Faut véritablement pour. Pour qu'elle soit appliquée vraiment quand même. Avoir fait preuve non seulement une mauvaise volonté mais véritablement en ayant refusé complètement d'entrer dans le dispositif. On voit bien que quand il y a des pénalités par exemple. Sur l'index, une femme. Elles sont pratiquement jamais arrivé à 1% vous voyez c'est un petit 0 5 0 2 0 3. Alors de 5%. Imaginez une entreprise de mauvaise volonté. Il me semble que vous la mettez vraiment situation budgétaire difficile et ça va conduire à licencier des gens, je pense que ce soit pas forcément la bonne méthode, maintenant, il faut fixer de bon niveau hein. Alors le gouvernement nous dit 1%, c'est le en général le taux habituel. Je pense que cela relève de la discussion des partenaires sociaux, si on veut faire en sorte qu'ils s'emparent. De cette dimension. Sur l'emploi des seniors. Il ne faut pas commencer à le remettre un cadre trop contraint en tout cas moi je m'y prendrais pas comme ça, voyez-vous je leur donnerai un peu de souplesse pour voir en sorte qu'elle est réellement leur volonté et là on peut peut-être arriver à quelque chose, il nous définirons effectivement les pénalités, qui s'impose, c'est la raison pour laquelle nous avons donné un avis défavorable. Avis du gouvernement, Monsieur le Ministre. Même avis donc un double avis défavorable. Il y a pas d'explication de vote je peux soumettre l'amendement on voit. Donc il est pour. L'amendement 3165 présentée par Madame Poncet moche. Qui est contre. Qui s'abstient. Il n'est pas adopté. Alors maintenant nous entrons dans la discussion de 139 amendements en discussion commune.

Merci monsieur le président. Donc par cet amendement. Nous voulons insister sur la notion de de senior ou de personnes âgées de plus de 55 ans comme l'a très bien démontré. Le rapport de Monique Lubin et René-Paul Savary. Sur l'emploi des seniors. La première difficulté consiste à définir ce terme. En effet, dans le monde sportif. La catégorie senior regroupe selon les fédérations, les pratiquants âgés de 19 à 40 ans environ plus âgées blessées. Les juniors mais moins que le vétéran dans certaines entreprises un cadre ou un consultant début de sa carrière en tant que junior et devient senior au bout de quelques années d'expérience. La notion de marché des seniors ou de Silver économie renvoie davantage aux retraités, voire aux personnes qui commence à connaître une perte de leur autonomie. Dans certains secteurs professionnels l'âge à partir duquel les salariés sont souvent envoyés alors seniorité et disent ressentir leurs premières difficultés dans les entreprises peut descendre à 45 ans, on le voit bien la définition de la catégorie sa dernière. Ou senior est un enjeu politique en que malheureusement le gouvernement a consciencieusement évacués c'est beaux coins il convient pour la bonne intelligibilité à la clarté de la loi de définir un âge plancher à partir duquel un actif peut être considéré comme senior. C'est l'objet de l'amendement, que notre groupe a déposé en le fixant à 55 ans. Si vous en êtes d'accord monsieur le président. J'évoquerai l'amendement suivant qui est un amendement de L'objet exactement le même on va dire mais qui a fixé le plancher l'âge plancher à 50 ans. Donc vous avez deux amendements hein qui fixe le plancher à 50 ans et l'autre à 55 ans, c'est bien ça. pour être dans l'ordre le le. 2613 ses 50 ans, élu 2614 55. OK. Donc ensuite le 2751. Madame Pumerole. Merci monsieur le président. L'article de tels qu'il est rédigé actuellement mettent en place donc un index seniors sans contrepartie financière et qui n'a nullement été négocié avec les organisations syndicales. Nous vous avons entendu monsieur le rapporteur. Donc nous faisons d'autres propositions et dans cet amendement, nous demandons que ces index actuellement inefficace puisse être remplacé par un index qualitatif qualitatif donc qui porte sur la formation, l'acquisition de nouvelles compétences l'amélioration de la qualité de vie au travail, l'aménagement de poste ou le temps de travail qui sont des facteurs extrêmement importants sur le plan de la santé au travail de nos seniors. Il faudra que cet index qualitatif soit négocié paritairement et il deviendrait alors. Il pourrait être alors mise en place en même temps des sanctions différenciées en fonction de la taille des entreprises. Cela pourrait rendre ainsi ce dispositif efficient.

heure. L'amendement 4126 c'est pour remplacer le terme poursuit par mais en oeuvre. Pour créer une obligation d'atteinte du maintien dans l'emploi des seniors. Je ne peux vous faire l'économie de la lecture de La Linea que nous souhaitons modifier l'employeur poursuit un objectif d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des seniors. Mais sincèrement, est-ce que c'est respecter le travail législatif que de demander aux entreprises un objectif d'amélioration. Est-ce que c'est respecter l'enjeu de l'emploi des seniors que de leur promettre un objectif d'amélioration. C'est le sens de toute la philosophie de cette réforme des retraites et plus largement de votre politique économique et sociale. On va demander aux entreprises de ce serait bien que les employeurs fassent et souvent sans résultat. Dans cette réforme, l'augmentation de cotisations employeurs sera compensé par un transfert des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles par conséquent rien n'est demandé aux employeurs dans cette réforme, c'est du jamais vu dans chacune des réformes que notre pays a connu. Dans votre politique économique et sociale nous demande au total de faire un geste sur les carburants. Total et laissé complètement seul pour fixer la nature et le montant de ce geste debout sur des carburants ou de en deçà de 2 euros a appris ça régulièrement plus élevés que les coûts de production, appris qu'il n'est pas d'actualité. Dans la politique des gestes les distributeurs bouc émissaire du gouvernement peut être trop gourmand. Mais quid des fournisseurs. Dans la politique des gestes, on avait eu les assureurs pendant le Covid. Alors que nos concitoyennes et nos concitoyens ne pouvait sortir de chez eux, il ne pouvait causer d'accident. À partir de ce constat, nous disions qu'il fallait taxer les assureurs ou qui diminue d'autant leur contrat l'année suivante. Le gouvernement leur a demandé de faire un geste. Vous avez créé un outil politique d'un nouveau genre l'aumône gouvernementale la supplique, plutôt que la loi. D'autres il ne Monsieur le Ministre, c'est le principe même de la philosophie libérale du laisser-faire laisser-passer cette doctrine vise à enjoindre au pouvoir politique de laisser les agents économiques les plus libres possible. C'est sûr que vous ne les dérangeait pas cet index ne les dérangera pas. L'amendement 4655 madame Vogel. Merci monsieur le président. Donc c'est un amendement de repli pour également améliorer cet index d'une autre manière. Bon, d'abord pour élargir les informations que qu'se serait publié dans cet index. En n'ayant pas seulement le taux d'emploi mais aussi des informations sur les conditions de travail des seniors sur l'adaptabilité de leur poste, etc. Ensuite. En n'ayant des des notes minimale à atteindre parce que ça sert à rien d'avoir simplement des informations comme ça, si on n'a pas des objectifs donc cet amendement propose d'avoir des objectifs et puis. Des conséquences au fait que les entreprises n'atteignent pas les objectifs avec une demande d'avoir par décret des sanctions financières appliquées aux entreprises qui ne respecteraient pas ces objectifs, ce qui est quand même un peu à priori la raison pour laquelle on met en place un index n'est-ce pas c'est c'est pas simplement pour pouvoir observer de loin le monde des entreprises, c'est quand même pour avoir un impact sur elle. Je crois que c'est pour ça qu'on fait la loi Aussi des propositions pour améliorer l'implication des partenaires sociaux dans la conception de l'index, vous avez dit et répété que certains partenaires sociaux étaient en faveur de certains ex-hé bien j'espère que vous vous accorderez avec nous sur le fait que il serait bien de les associer et puis également ramener la date d'application au 1er janvier 2024 pour les entreprises qui ont plus de 299 salariés et pour celles entre 50 et 299 au 1er juillet 2024. Nous aurons d'autres amendements que nous discuterons dans la suite pour améliorer cet index mais vous voyez que nous avons beaucoup de propositions. Nous essayons de d'aborder la chose de manière constructive. L'idée n'est pas de rejeter l'index en soi c'est de rejeter un index qui ne sert à rien. Donc j'espère que ça. À la fin de la discussion pourra servir à quelque chose et que vous pourrez nous donner des raisons de le voter. Bien merci ensuite deux amendements identiques, le 1er, le 2753 et présenté par monsieur Assouline. Oui, merci monsieur le président. Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à préciser le contenu de l'objectif de d'amélioration de l'embauche et du maintien en activité des salariés âgés qui traitera des thèmes suivants. Hein. Le recrutement des salariés âgés dans l'entreprise de l'anticipation de l'évolution. l'amélioration des conditions de travail et de prévention des situations de pénibilité. IV le développement des compétences et des qualifications et accès à la formation. l'aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite et la transmission des savoirs et des compétences et développement du tutorat. Voilà ce que contient l'amendement concrètement et. Les nouveaux retraités du régime général. Avait validé des trimestres dans le cadre de l'emploi durant les mois précédant la liquidation de leur droit à la retraite selon le corps. Ils étaient. Ils étaient le chiffre exact étant. Excusez-moi. Bon je vous donnerai. Un emploi durant bon hein. Les 25% selon le corps n'avait validé aucun trimestres dans l'année précédente, de leur retraite en 2019, un rapport sénatorial votre rapport Monsieur Savary avec Madame Monique Lubin s'était penché sur le défi des fins de carrière. Vous aviez mis en évidence un marché du travail. Plus. Pour les personnes les plus âgé avec une prévalence de chômage de longue durée plus importante chez les plus de 50 ans que dans la moyenne des demandeurs d'emploi. L'enjeu pour notre système d'Europe. et ben j'arrête. Il y a pas de problème. Il y en a un autre après je continuerai. Oui il y a un 2ème amendements identiques, le 4129 présenté par Monsieur Ouzoulias. Merci monsieur le présent. Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues, j'ai, j'ai du mal qu'on a à comprendre quand même monsieur le rapporteur. Mais je pas revenir sur le débat sur la différence d'appréciation que vous portez sur l'article 1er que vous avez refusé et sur l'article de que vous acceptez. Or, on aurait pu parfaitement mobilisé l'argumentaire de l'article 1er bis qui vous a permis de le refuser. Contre, contre l'article de mais. Puisqu'il faut en venir à à cet article. Ce qui est très gênant, c'est que cet article ne définit pas les index alors. Le. L'article en question renvoie tout ça. Un décret pris en Conseil d'État et pour une loi d'urgence, ça pose quand même problème. On est dans une loi de finances rectificative qui renvoie à un certain nombre de dispositions 10 décret pris en Conseil d'État. Je peux prendre ici le pari que les décrets pris en Conseil d'État, nous les aurons pas avant la loi de finances de de de cette année. par ailleurs. Votre votre gouvernement avait pris une toute autre option quand il s'agissait de définir les critères dans la loi du 5 septembre 2018, c'est l'article 104. Vous n'aviez pas défini précisément les critères mais en revanche que vous aviez fait d'un point de vue législatif s'est donnée par la loi un cadrage qui permettrait la définition de de ces de ces index et je pense que ça aurait été une meilleure solution je vous proposerai dans dans un amendement futur un certain nombre de de cadrage pour permettre la définition de 16 index. Merci monsieur le président. Merci. Ensuite le 3465 Me Poncet Monge. Merci monsieur le président, alors par cet amendement. Le groupe écologiste solidarité et territoires. Propose d'établir. Un barème d'évaluation des indicateurs et d'établir, oui des sanctions pour résultats insuffisants.

un petit peu comme pour les hommes et les femmes où il faut un plan d'action. Il suffira ainsi pour une entreprise mauvaise élève en matière d'emploi des seniors de simplement publié l'index pour échapper à une sanction et nous on a vu que. C'était peu efficace. Donc, il est donc que cet index sera un, un impôt. Un impact nul, c'est un dispositif d'évaluation chiffrée qui inclut un score minimum atteindre forcément sous peine de sanctions n'est pas mis en place ces sanctions financières doivent. Également être adaptés à la taille des entreprises. Je l'ai dit c'est différencier. Qui ne dispose pas des mêmes ressources notamment RH pour mettre en place une telle mesure. Merci. Ensuite le 4656 madame Vogel. Merci monsieur le président. Cet amendement vise à élargir le nombre d'entreprises qui seraient concernés par la l'obligation de publier cet index. En limitant seulement la non publication aux entreprises qui ont moins de 10 salariés. C'est quand même 96,2% des entreprises françaises qui sont des micro-entreprises mais. De, d'obliger les entreprises à publier l'index dès qu'elles ont au moins 11 salariés. En abaissant le seuil de 300 salariés à 50 salariés qui serait déjà un pas dans la bonne direction on rajouterait environ 5000 entreprises à l'obligation de publication. En effet il y a environ. 4520 entreprises qui emploient entre 50 et 249 salariés. Mais c'est pas assez parce que ça exclut toujours toute les micro-entreprises et les et Et. La majeure partie des entreprises françaises comme j'ai dit au début, 96% sont des petites entreprises. La moitié des Françaises et des Français sont employées par des micro-entreprises ou des PME. Il faut donc dans la mesure du possible, élargir le Champ d'application d'index des seniors pour améliorer la transparence en espérant que plus d'entreprise, emploi des seniors s'en effet essentiel pour permettre aux seniors qui devraient travailler plus si cette réforme était mise en oeuvre de trouver un emploi. Nous pensons également qu'un élargissement de l'index, à des entreprises de plus de 11 salariés ne représenterait pas une charge insurmontable pour ces entreprises. Quand on a 11 salariés. On voit vite en fait qu'on Maya de seniors. Voilà si vous voulez c'est un peu plus facile à compter. C'est pourquoi nous proposons d'élargir le Champ d'application de l'index aux entreprises de plus de 11 salariés. Je vous remercie. Merci. Cher collègue, peut être que il peut y avoir un peu moins de conversations à l'intérieur de l'hémicycle. On peut toujours en avoir à l'extérieur. En plus je pense que vous avez souhaité. Adopter cet article donc il est normal qu'il y ait un débat sur les amendements visant à l'enrichir. Donc maintenant l'amendement 1970 qui est présenté par Monsieur Étienne Blanc. l'inverse de ce qui vient d'être indiqué. C'est un amendement qui a pour objet de relever le seuil à 300 salariés. Imposer. À des entreprises de l'ordre de 50 salariés. Ce dispositif. Qui va évidemment évoluer sur le plan réglementaire. Cela va créer des charges sur des entreprises qui souvent n'ont pas les services de ressources humaines. Suffisamment important et on le sait. Un des soucis qui pèse aujourd'hui sur ce type d'entreprise là, c'est la masse des contraintes administratives qui sont excessives. Qui plus est, un grand nombre d'entre elles sont assorties de sanctions, voire même parfois de sanctions pénales. Donc ce dispositif de l'index senior ne devrait s'appliquer qu'à des entreprises de plus de 300 salariés pour éviter, je le redis de pénaliser ces petites entreprises qui font la richesse de la France.

relever le seuil à 300 salariés dans les entreprises. Qui doivent publier un bilan social qui ont des services de ressources humaines mais j'en profite pour faire une remarque. Voilà, mes chers collègues, je vous ai trouvé bien acrimonieux avec ces fameux index senior. J'ai même entendu tout à l'heure que c'était. Une demande du MEDEF. Non. Le MEDEF sur l'index senior, il est sur la même ligne que vous figurez-vous, même si je dois être taquin, il est contre l'index senior le le les partenaires sociaux favorables à l'index senior. C'est la CFDT et donc. Nous proposons cet amendement parce que cet index seniors il doit vivre et il doit pas non plus. Être encadré. Au-delà des contraintes. Parce qu'autrement il n'y aura pas de paritarisme, si on veut faire vivre le paritarisme, il faut laisser les partenaires sociaux travailler sur senior sur cet index. Avant 10 mètres des contraintes et puis je relève aussi le paradoxe, c'est l'incohérence de ceux et celles et ceux qui étaient pour la suppression de l'index senior et qui maintenant veulent l'étendre à toutes les entreprises, pardonnez-moi, mais ça me paraît quand même curieux quand on est contre quelque chose, on ne veut pas le le le le l'étendre à toutes les entreprises me semble-t-il hein. Voilà nous on croit au paritarisme, on croit aussi hein, à la responsabilité sociale. Sociétale et environnementale des entreprises. C'est la raison pour laquelle on est favorable à à cet article est à cet amendement, je vous remercie. Et ensuite donc l'amendement présenté par la Commission, Monsieur Oui merci effectivement on est parti exactement de la même philosophie, à savoir que le seuil de 300, c'est le seul de gestion de discussions au sein de l'entreprise, de la gestion prévisionnelle des emplois et en conséquence véritablement on peut bâtir dans. À partir de 300 salariés. Une véritable. Politique. Ambitieuse d'employabilité des des seniors en dessous, en dessous c'est un peu compliqué, vous voyez-vous. Parce que. Vous êtes dans un bassin d'emploi qui est plutôt dans une population un peu vieillissante. Vous pouvez effectivement. Plus facilement trouver. Des emplois seniors. Vous êtes dans un bassin d'emploi plus jeune là ma foi c'est plus les jeunes qui vont répondre aux appels que vous proposez. Sachant que vous allez pas là aussi dire je veux un homme une femme, je veux un, un jeune je veux un senior. Non il y a pas de discrimination des appels d'offres sans faire des propositions d'offres d'emploi sont ouvertes à toute la population et en conséquence en dessous de 50. C'est difficile il y a pas les ressources humaines qui permettent effectivement de gérer. De façon prévisionnelle notamment les emplois c'est pour. C'est vrai qu'il faut trouver d'autres critères, mais les partenaires sociaux vont nous donner d'autres critères les indicateurs c'est eux qui vont les établir et d'autre part il y a pas que les indicateurs qui compte, c'est bien beau de poser les indicateurs. Encore faut-il qu'il soit évolutif. Parce que 2 ou 3 ans après et correspondent plus forcément aux emplois que vous avez eu il y a véritablement, on le sait, une dynamique nouvelle dans le domaine de l'emploi. Les emplois demain dans, dans 20 ans. Nous ne savons pas quelles ils sont donc il est difficile de former pour les emplois dans 20 ans. Hein. Car il y a une évolution technologique telle que on ne sait pas comment cela va évoluer. C'est la raison pour laquelle il nous semble que il faut limiter ce seuil à 300. Merci monsieur le rapporteur. Ensuite le 2754 enfin il y a 2 amendements identiques, là aussi le 1er présenté par monsieur Assouline. Moments de confusion tout à l'heure dans mon argumentation parce que j'avais des chiffres un peu inverser donc je répète en 2019 55 % des nouveaux retraités du régime général avait validé des trimestres dans le cadre d'un emploi durant les mois précédant la liquidation de leur droit à la retraite selon le corps un quart avait valider leurs trimestres tout en étant soi au chômage en invalidité ou en maladie les 25 restant selon le corps n'avait validé aucun trimestres dans l'année précédente, leur retraite corriger ce moment où j'ai un peu bégayer. Tout à l'heure l'amendement que je défends maintenant au nom du groupe socialiste républicain écologiste et caetera, cet amendement vise à préciser que les indicateurs sur les travailleurs seniors devront être envoyées par l'entreprise au ministre du Travail, ainsi qu'un pôle emploi transmettre. Ces indicateurs est un préalable pour que Pôle emploi puisse oeuvrer au changement de culture des employeurs envers les salariés âgés ou en fin de carrière et déployer des actions spécifiques adaptées d'adressage des candidatures de salariés de plus de 50 ans vers les entreprises. Qui se doivent de développer l'embauche de ses profils et pour conclure, une réponse à notre collègue qui vient de s'exprimer du groupe centriste. Il y a pas de paradoxe à à nous critiquer sur le fait qu'on était pour le rejet. De cet article pour sa suppression et le fait que maintenant on veut l'étendre. Le préciser le renforcer, c'est justement. On a considéré. Que cet article n'apportait rien pas que la question de l'emploi des seniors n'était pas un sujet on pense même que c'est le sujet central qu'on aurait dû traiter avant cette loi. Fait à la va-vite et et nichée comme cela. Sauf que voilà. On vient en parler là où il ne faut pas et de façon. Tellement. Tellement insignifiante. Que ça peut au contraire ça reculer. Cette idée. Que l'on doit traiter y compris par un index pour avoir des données pour avoir une objectif délégation de la de de de la situation. Donc voilà ce que je voulais dire et on va continuer à essayer de faire qu'il ait du contenu à travers les débats qui vont continuer sur cet article.

Pour notre part, nous estimons qu'elles doivent être fournis au ministère du Travail et donc à Pôle Emploi afin de coordonner des politiques nationales et territoriales d'accès à l'emploi des seniors. aussi revenir sur la question des seuils qui a été évoqué. Dans l'amendement numéro 2015. Émanant des bancs de nos collègues centristes et de la commission et je l'ai aussi en j'ai encore une question, pourquoi donc s'opposer à ce que les entreprises de 50 salariés de moins de 300 soient concernés notre amendement lui s'inscrit d'une certaine manière dans l'extension de la base de données économiques sont ce qui a, social et environnemental. Ce document donc transmis par l'employeur aux membres du comité économique et social pour les entreprises dès 50 salariés. Je rappelle que ce document comprend les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, la formation professionnelle, l'organisation du travail, le recours à des contrats temporaires et à des stages des stages je pense pour ma part qu'il suffirait d'intégrer à ce document, les données relatives à l'index des seniors et comme le prévoit cet amendement de le transmettre donc automatiquement au ministère du Travail et un pôle emploi donc je vous pose une question monsieur le rapporteur. Et Monsieur le Ministre, qu'en pensez-vous.

Oui, merci monsieur le Président, je tiens dit en préambule, que nous ne voulons être ni sectaire, ni faire de l'obstruction. Nous sommes là pour débattre ou même si on était contre et moi j'étais fait activement contre mais maintenant que ça a été voté bien je respecte les décisions de notre haute assemblée. il s'agit par cet amendement de mieux encadrer et de fixer les limites et les objectifs prioritaires afin de clarifier les domaines d'application et les étendues, des mesures qui seront prises pour améliorer concrètement les conditions d'accueil et d'ergonomie pour ces seniors. Il s'agit également de mettre en oeuvre des actions de prévention des risques en matière de sécurité mais aussi des risques. Psychosociaux parce que très souvent les personnes déjà fragiles des seniors. Hé bien mérite un encadrement qui serait beaucoup plus pertinent plus précieux Jaziré parce qu'il s'agit à la fois pour l'entreprise de gagner en compétences mais aussi de la personne de gagner en qualité de vie. Donc nous ne devons pas faire n'importe quoi et c'est la raison pour laquelle je souhaite vraiment que cet amendement soit votée, je vous remercie. Merci monsieur le président. Alors l'écart salarial entre les femmes et les hommes est toujours important. Et même si cet écart est moins important qu'il n'était au début du siècle. Rien ne justifie qu'une femme gagne bien moins pour le même travail. Il faut aller beaucoup, C'est dans ce contexte que s'inscrit le projet de réforme dont nous débattons aujourd'hui. D'un côté cette réforme des retraites du gouvernement pénalisera nous en parlerons largement davantage les femmes. Rien que la mesure de repousser l'âge légal de départ à la retraite touche les femmes plus que les hommes car elles travailleront encore plus que ne travailleront les hommes en plus pour avoir droit à la retraite à taux plein. De l'autre côté, cette réforme prévoit que les seniors continuent à travailler, donc de la de leur 62 ans ce qui repose quand même avec toute. Avec beaucoup d'acuité la question de l'égalité des genres. Pour les seniors qui devrait si l'arrêt réforme passe. Ce n'est pas retiré travailler plus longtemps donc il faut à tout prix éviter que les écarts se creusent encore. C'est pourquoi nous proposons de compléter l'index senior par des indicateurs évaluant les écarts entre les hommes et les femmes. Les entreprises de plus de 50 salariés, cela serait alors obligé de publier l'écart des salaires des seniors. Ça n'évitera pas pas tout, il est vrai, mais ça se, c'est un élément important. Porté à notre connaissance et d'autant plus important que les fins de carrière des femmes sont très différentes de celles des hommes. Une étude de la Dares S de 2021 avait montré entre autres que les femmes seniors sont plus souvent en temps partiel dit contraint avec les réductions de salaires que cela entraîne à leur suite au débat à l'Assemblée nationale et aux demandes de la gauche. Le gouvernement a élargi ou plutôt précisé l'index senior pour le ventiler selon les sexes, ce n'est-ce c'est bien mais ce n'est pas suffisant parce que cela n'oblige pas les entreprises à publier les données sur l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Seniors. C'est pourquoi nous proposons cet ajout. Dans, dans Merci le 4136 qui est présenté par Monsieur Savoldelli. Oui, merci Monsieur. Le président, Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues. Cet amendement comme d'autres, pose la question non pas seulement favoriser le maintien dans l'emploi. Des plus de 50 ans mais de le garantir. Et là j'ai retrouvé. Les propos du président Macron en avril 2019, je le cite et et quand les Français, les Françaises se le rappelle, je peux vous dire que ça élargit la mobilisation par rapport à la réforme des retraites. président Macron 2019, je le cite, quand aujourd'hui on est peu qualifiés. Quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielles. Quand on est soi-même en difficulté qu'on a une carrière fracturé. Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. Et alors, on va dire non non faut aller maintenant à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire. Après 55 ans, les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. On doit d'abord gagner ce combat avant d'expliquer aux gens mes bons amis travaillez plus longtemps. Ça c'est les propos du président de la République à son grand débat. Ça vrai. Comprenez ce qui se passe, pourquoi il y a une telle unité syndicale. Une telle mobilisation citoyenne et et politique contre cette réforme parce que qu'est-ce qui a changé et c'est là où la politique ça peut pas être premièrement une valse-hésitation toutes les cinq minutes mais pas non plus du marketing. Quand on prend des engagements il faut les tenir en politique. Et qu'est-ce qui s'est passé 1,5 points supplémentaires pour le ton emploi des seniors en plus pour le porter à 56 en 2021. C'est une augmentation de 2,7%. Qui peut penser qu'à une révolution pour la vie des femmes des des hommes qui ont plus de 50 ans, soit pour leur maintien en activité, soit pour leur embauche il s'est rien passé, le taux d'emploi des seniors et au-dessus de 1980 alors que l'âge de départ était fixé à 65 ans, si bien que là, si on réfléchit, et non pas par un raisonnement par l'absurde. Si bien que dire que l'âge légal et ce qui force au travail plus longtemps. Hé bien, une hérésie sinon dans notre système de retraite actuel à 62 ans, ils devraient travailler moins. Donc le son de l'affaire, le montant des pensions et systématiquement la variable d'ajustement de la réforme des retraites qui nous est proposé. le présent amendement du groupe écologiste solidarité et territoires vise à inclure le temps partiel. Parmi les indicateurs de l'index senior. Il y a plus de temps partiel chez les seniors que dans n'importe quelle autre classe d'âge. Si si une partie du recours au temps partiel s'explique par le cumul. Emploi-retraite. à l'exclusion du cumul emploi-retraite. Il reste encore légèrement supérieure à 10%. Il risque de ça s'accentuer de façon volontaire ou contrainte par l'état de santé. Avec le recul de l'âge de la retraite afin que ces situations qui conduit souvent à une hausse de la précarité des seniors ne soit pas invisibiliser. Groupe écologiste solidarité et territoires demande que l'examen du recours au temps partiel soit systématiquement inclue dans les indicateurs de l'index comme ils auraient dû être dans l'index d'égalité professionnelle hommes- femmes. Si. Le 4145 Madame Cohen. Merci monsieur le le président, effectivement. L'index senior. On l'a dit et inférieur en fait à l'index. Professionnelle entre les femmes et les hommes qui a été vidée d'ailleurs de son contenu et qui a vu se dresser toutes les associations féministes et beaucoup de syndicalistes contre lui parce que les pénalités sont effectivement il faudrait en il faudrait en tirer des des leçons. Je vais vous donner quelques exemples par rapport à cet indicateur professionnelle entre les femmes et et les hommes par exemple, si 10 femmes sont augmentés de 10 euros, tandis que 10 hommes sont augmentés de 100 euros, l'entreprise obtiendra tous les points sur cet indicateur ou encore si tous les salariés sont augmentés à leur retour de congé maternité, ce qui constitue une obligation légale et ce et ceux d'un euro l'entreprise validera également l'indicateur bref un paramétrage qui explique les très bons scores qui sont obtenus par les entreprises depuis le lancement de l'index, alors même que les femmes continuent encore à gagné en moyenne 23% de moins que les hommes et être payé près de 17% de près de 17% de moins à poste égal, donc on voit bien que les index c'est quand même important, mais alors l'index senior. Il est encore inférieur à ses exigences là. d'un des deux d'associer l'index senior à des sanctions, c'est un recul du gouvernement, une fois de plus face au au MEDEF. Pourtant j'ai l'impression monsieur le rapporteur. René-Paul Savary, que vous êtes d'accord avec nous, avec notre groupe et que vous trouvez comme nous inadmissible la situation qui est faite aux seniors face à l'emploi à 60 ans près d'une personne sur 3 n'est ni en emploi, ni à la retraite. La majorité d'entre elles et eux se retrouvent en invalidité ou en situation de RSA ou chômage donc en grande précarité. donc en tirer des leçons et accepter l'enrichissement grâce à notre abonnement. Merci le 4151 madame Gréaume. Merci monsieur le président. Avec cet index vous mettez le doigt sur un problème majeur. Comme disait ma collègue, celui de l'emploi des seniors. Connaissez-vous les réalités de l'emploi que vivent nos concitoyens pour en être certaine. Je vous rappelle quelques chiffres, 61,3 pour des personnes n'existe déjà plus d'activité à 61 ans et cela atteint 73. J'ai On imagine déjà comment cela évoluera jusqu'à 64 ans. Il est difficile d'obtenir un emploi au-delà de 55 ans puisque les employeurs suppose notamment une moindre productivité ainsi qu'une moindre adaptabilité. Cela est encore plus vrai comme comme toujours pour celles et ceux qui ont connu durant leur carrière un certain nombre de discrimination. Je pense aux femmes, aux personnes en situation de handicap, etc. Alors pour votre Addex. Nous proposons de prendre en compte ces critères pour améliorer l'égalité professionnelle et ainsi éviter les manoeuvres pour contourner les dispositions prévues et le sens de cet article, merci. Merci monsieur le président. Donc cet amendement a pour but de rappeler. Donc. De rappeler.

Donc dans certaines de nos localités. La démographie, la démographie est stable dans à d'autres endroits et les croissante et dans d'autres, elle est même décroissante plus la population est grande, plus l'entreprise est grande mais lorsque la population est moindre hein certains endroits certains aux entreprises ne peuvent compter. 300 salariés au sein de leurs effectifs. Il faut donc prendre en compte un plus grand nombre d'entreprises pour que la place des seniors soient réellement une priorité au sein de ces dernières. Cet article ne s'adapte pas assez différences la valorisation du travail des personnes âgées doit s'appliquer à toutes les échelles. Même si l'entreprise ne compte pas 300 salariés. Ce ne sont pas toujours les plus grandes qui doivent être privilégiées afin qu'une telle une qu'une réelle stratégie d'inclusion des personnes âgées dans le milieu du travail soit efficiente. Il faut donc prendre en compte la singularité des territoires. Même si j'aime pas le mot territoire l'exposé de l'article du gouvernement va dans ce sens pour toutes ces raisons, nous proposons d'abaisser le seuil à 150 salariés. Cela permettra plus d'entreprises de prendre en compte la place de nos aînés, au sein de leurs effectifs et de ce fait, de prendre en compte les les territoires que je n'aime toujours pas le mot que je n'aime toujours pas qui n'ont pas la même strate de population. Madame Poncet Monge pour le 3467. Merci monsieur le président. Alors si on veut faire vivre l'index senior. Si on croit au paritarisme. Si on croit à la responsabilité sociale et environnementale. On écoute les organisations syndicales, je viens de citer mon collègue Olivier Henno alors immédiatement presque. J'ai décidé de défendre. Avec conviction. Cet amendement qui est proposée par une des organisations syndicales, l'UNSA. Hein, vous voyez une Il peut pas que la CFDT et donc je pense Monsieur et nous que vous parliez de toutes les organisations. Donc voilà. Cette organisation propose que de la même manière que les entreprises ayant des résultats insuffisants à l'indicateur et d'égalité professionnelle sont sanctionnés financièrement. Le groupe écologiste solidarité et territoires reprend leur proposition de sanctionner les entreprises ayant des résultats insatisfaisants, au regard des critères de l'index senior et pas uniquement celles ne publiant pas simplement l'indicateur sur l'emploi des seniors. cette sanction. Permettrait de créer une incitation financière mais aussi réputationnel c'est pas très joli afin que les entreprises mettent en place des politiques d'emploi réellement efficace en faveur des salariés âgés et du taux d'emploi des seniors. Merci. Ensuite le 3177 toujours vous Madame Poncet mange. Alors toujours dans cette écoute des propositions des organisations syndicales à la, à laquelle on a été invité. Nous proposons d'encadrer l'étendue et les modalités de l'index seniors afin de s'assurer que cet outil, il faut que ça soit vraiment un outil, c'est-à-dire qu'ils soient opérant opérant est réellement un impact sur les entreprises en matière d'emploi des seniors et d'amélioration de leurs conditions de travail. Est ainsi proposé d'entourer la mise en place des critères le composant par décret d'un cadre législatif. C'est important, un cadre législatif ça permet de garantir la prise en compte des politiques d'emplois publics, des conditions de travail et de rémunération des salariés proches de la retraite afin que l'ADEC soit l'outil de mesure le plus efficace possible au service justement ensuite ou en parallèle de la négociation de branche puis en entreprise. Par ailleurs, l'inégalité entre femmes et hommes quant au niveau des pensions de retraite et à l'âge effectif de du départ de l'âge de, à la retraite nécessite une déclinaison des indicateurs dans le Champ de la mise en oeuvre de l'égalité professionnelle. Voilà je vais raccourcir je vous invite à lire le reste puisque c'est dans l'objet et c'est un amendement effectivement proposé par l'UNSA, que le groupe écologiste solidarité et territoires soit. Avec eux, a fini cet index par la clarté, la précision, la transparence dans la définition des indicateurs. Je vous remercie. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes, mes chers collègues, nous nous continuons dans dans le le cadrage que je vous ai présenté le cadrage législatif de la définition des index et vous nous vous en proposons quelques-uns notamment que ces index prennent en compte le recrutement, les fins de contrat le, le taux d'emploi, la prévention des effets d'avis défavorable et les risques inhérents aux carrières longues ensuite la durée des des des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité, la pénibilité, le maintien des niveaux de rémunération, les cumuls d'emploi retraite et et comme nous sommes très sensibles au au dialogue social bien évidemment nous prévoyons par par. Par cet amendement que une convention de branche puisse enrichir la laisse la liste des indicateurs mentionnés au premier Rania telle que je viens de faire et cette liste pourrait se substituer ensuite aux de créer. Merci Monsieur le Président. Merci, ensuite le 2759 présenté par. Madame Monier. Madame Le Houerou pardon. L'index seniors afin de s'assurer de son efficacité. Alors nous proposons. Que soit précisée dans le décret 5 élément à prendre en compte la prévention des effets défavorables et risques inhérents carrières longues ou à la pénibilité des professions, notamment en matière de santé et sécurité des travailleurs. 2ème élément l'organisation des conditions d'emploi et de travail, la durée des contrats de travail, le temps de travail, la mobilité les la pénibilité. 3ème élément le maintien des niveaux de rémunération et les dispositifs d'entreprises de financement des retraites. Le 4ème élément les cumuls emploi retraite la reconversion. Professionnelle des seniors ou les retraites progressives dans l'entreprise. Nous proposons également qu'une convention de branche soit étendu et qu'elle puisse enrichir la liste des indicateurs. Ce cadre permettra de garantir la prise en compte des politiques d'emploi, des conditions de travail et de rémunération des salariés proches de la retraite afin que l'index soit l'outil de mesure le plus Effi efficace possible au service de la négociation en branche et en entreprise. Cet amendement a été travaillé avec l'UNSA, merci.

je pense qu'on l'a bien compris l'index senior. Repêché par le gouvernement après que l'Assemblée nationale ne l'est pas jugé convaincant cet index et peu contraignant puisqu'il ne prévoit qu'une obligation de pour que l'index senior est un réel impact sur les pratiques des entreprises en matière d'emploi des salariés seniors. Il faudrait inclure dans ce dispositif un barème d'évaluation avec une note minimale à atteindre. C'est ce que vous propose cet amendement.

cet amendement. Pour notre part VISA intégrer à l'index senior son évaluation sans quoi il sera, il serait difficile de mesurer la progression restant à accomplir, car l'employeur doit assumer son objectif d'amélioration d'embauche et du maintien en activité des travailleurs seniors après avoir réclamé à cor et à cri que vous lui livre il est encore plus de main d'oeuvre il les voulait ces deux ans de plus que vous arracher au peuple tous ici puisqu'ils devront travailler demain les salariés jusqu'à 64 ans vous voulez-vous vouliez évidemment aussi ses 64 ans. Nous vous avons démontré les économistes l'ont également démontré. Vous ne vous engagez pas pour sauver notre système de retraite, c'est autre chose ici qui vous anime. Et si tel site. Elle n'est pas le cas, pourquoi vous obstiner à à refuser d'établir des seuils satisfaisant pour l'emploi. Des travailleurs les plus vulnérables, vous promettez des grandes négociations qui laisserait la part belle à l'expression de toutes et tous et et qui permettent d'entretenir évidemment le flou. Nous ne voulons pas d'un flou sur ce type de mesure un barème d'évaluation comprenant une note minimale à atteindre doit constituer un cadre d'objectifs, nous souhaitons qu'au-delà du fétiche ou plutôt de cet épouvantail qui ne prend auprès de personnes nous soyons un peu sérieux. La construction de cet index et son évaluation permettra de situer précisément les marges de progression de chaque entreprise un tel seront 200 en matière de formation qui, nous le savons, est un très grand chantier. Un hôtel sur l'aménagement des fins de carrière. porteuse de sens, nous introduisons d'ailleurs un délai afin d'atteindre un seuil minimal acceptable. Merci. De notre groupe socialiste, écologiste et républicain vise à confier à un accord national interprofessionnel le soin de construire les indicateurs de l'index. Senior alors un accord national interprofessionnel est un accord négocié et signé par les partenaires sociaux et donc nous donnera des gages d'efficacité dans la mise en oeuvre le dialogue social important primordial, même dans ce domaine précis de la définition des index la place des partenaires sociaux doit être respecté. La discussion avec avec ses partenaires doit permettent de trouver le bon équilibre et les indicateurs les plus pertinents pour assurer l'efficacité de cet index

et non pas de manière discrétionnaire mais par un accord national interprofessionnel. La. Avec notre amendement nous redonnons donc toute sa place. Vous nous dites, Monsieur le Ministre, je pense que vous la voulez aussi. C'est la place que doit avoir la négociation collective dans la mise en place de l'index senior. Donc j'ai pu retrouver avec mon groupe les les dires de l'ancien membre du Conseil constitutionnel, Olivier. La Motte qui résumait dans sa contribution à la revue semaine sociale les 4 atouts possibles une norme négociée collectivement. Et vraiment. Son diagnostic est utile. D'abord elle vient des acteurs même de l'entreprise. Deuxièmement les mains des partenaires sociaux et elle est le plus souvent novatrices la troisième elle est souvent impliqués car. Et enfin elle est au souvent plus stable au vu de l'enjeu. Le seul cas collectif qui convient reste celui de de l'année, donc l'index senior ne peut se passer de négociation nationale visant à couvrir une majorité des travailleuses et des travailleurs. Seniors. Voilà le sens de cet amendement. Je pense que le caractère massif et nationale des discriminations faites aux salariés âgés rend légitime de laisse au dialogue social, le temps nécessaire aux revendications et à la discussion. Merci et ensuite le 2756 Madame Rossignol. Merci monsieur le président. Alors l'alinéa 6 de l'article 2 prévoit que la liste des indicateurs et leurs méthodes de calcul sont fixées par décret, nous proposons avec cet amendement de préciser qu'il s'agit d'un décret en Conseil d'État. Alors pourquoi un décret en Conseil d'État parce que le décret en Conseil d'État est une procédure différente et suppose par ailleurs de passer par le Conseil des ministres. Or ce décret nous paraît important dans la mise en oeuvre de l'index senior. Nous sommes beaucoup ici ont cité. L'index égalité femmes-hommes, or, il faut tirer les leçons de ce qu'on constate sur l'index égalité femmes-hommes nombreux biais. Et des billets qui tiennent à la fois sur la question des des comparaisons sur les augmentations des femmes des augmentations sur les nombres de femmes promues comparer bien entendu aux aux augmentations accordées aux hommes aux augmentations au nombre d'hommes promus Laurence Cohen tout à l'heure à fait référence à un certain nombre de de d'exemples qui montrent que ces biais en fait permettent à des entreprises qui ne respectent que la moitié. des prescriptions de l'index égalité d'obtenir le nombre de points suffisants les 75 points qui leur permettent d'échapper. Aux sanctions d'abord et ensuite au rattrapage de leur politique. Donc instruit de tout cela il nous faut nous prévoir le meilleur indicateur et on pense que lundi que le Conseil d'État est est une est une garantie d'un meilleur indicateur et surtout de plus d'interministérialité et puis enfin dernière élément. Un indicateur au Conseil d'État, un décret en Conseil d'État a un gros avantage, c'est que peut-être il y aura un avis.

je défends l'amendement qui a été présentée par mon collègue Thomas Dossus mais qui a dû. Rentrer à, à Lyon, c'est aussi d'ailleurs un amendement proposé par le groupe écologiste solidarité et territoires. Il vise à prendre le décret qui définira la liste des indicateurs à l'index senior après consultation de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail l'Anact. L'index senior qui est proposé dans le texte et la principale. Et avouons-le, nous l'avons d'ailleurs tous reconnus ensemble bien maigres mesures prévues par le gouvernement pour. Mettre fin au chômage des seniors ou en tous les cas pour réduire le chômage des des seniors. Cette mesure se base sur l'idée qu'un index. Que les entreprises de plus de 50 salariés devrait publier tous les ans suffirait à résoudre les difficultés auxquelles font face les seniors en recherche d'emploi. Olivier Mériaux. L'ancien directeur technique et scientifique de l'Anact a jugé hypocrite et dangereuse. La proposition du report de l'âge légal de départ à la retraite. Dans une tribune parue dans Le Monde fin janvier. Il précise qu'aucune mesure ne pourra contrebalancer les impacts d'un recul de la borne d'âge pour une large partie du corps social déjà fragilisé. Selon lui, l'index senior n'échappe pas à ce constat, l'index senior est une mesure plus qu'insuffisante qui ne comporte de surcroît aucune garantie renvoyant à un décret le soin de fixer la liste des indicateurs de cet index ainsi que leurs méthodes de calculs établir de tels indicateurs ne peut se faire sans la consultation des acteurs concernés par la thématique du travail et de l'emploi et notamment l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et d'emploi l'Anact à plusieurs domaines de compétences notamment. Je m'arrête puisque excusez-moi j'ai dépassé le temps. Et pour rattraper un peu de ce temps. Si vous m'y autorisez. Monsieur le Président, j'enchaîne avec l'amendement suivant. Absolument, il y a trois amendements identiques, c'est vous qui présentez, le premier, allez-y. le présent amendement porté par le groupe écologiste solidarité et territoires vise à prendre le décret qui définira la liste des indicateurs de l'index senior après consultation cette fois-ci du Conseil économique, social et environnemental de ces Si l'on en croit l'étude d'impact fournies par le gouvernement, l'index senior prévu à l'article de de ce texte a notamment pour objectif d'objectiver la place des seniors en entreprise d'assurer la transparence en matière de gestion des âges et de mettre en oeuvre une logique d'amélioration continue des pratiques des entreprises, en mobilisant le dialogue social dans l'entreprise. L'emploi des seniors est un sujet qui mérite d'être traité avec sérieux. D'après l'OCDE, le taux d'emploi des 55 64 ans atteint 56 8 % en France contre 62 6 % dans la zone euro. Les salariés de plus 50 ans sont souvent victimes de pratiques délétères de la part d'un d'un certain nombre d'entreprises qui préfèrent les placardisés ou les licenciés les discriminations ont la vie dure. Ces salariés en fin de carrière sont nombreux à être jugé trop coûteux ou encore trop susceptibles de tomber malade. Ils subissent une double peine une fois licenciés. Il leur est très difficile de retrouver du travail. Si le gouvernement veut prendre à bras le corps le problème du chômage, comme il l'affirme, l'index senior est une solution bien maigre et ce ne sont pas les résultats de l'index de l'égalité professionnelle hommes-femmes comme vient de le démontrer. Ma collègue qui contredisent ce constat. C'est pourquoi face à la détermination de tels indicateurs comme la détermination de ces indicateurs ne peut se faire à la légère. Nous proposons par cet amendement de repli d'obliger le gouvernement à consulter le 16 pour établir par décret l'A10 des indicateurs de l'index senior. Merci. Ensuite donc 2 amendements identiques à celui-là le premier la présidente Rossignol. Merci monsieur le président. Qu'on se fasse bien comprendre d'abord moi je l'ai dit tout à l'heure je suis pas hostile à la technique des index. Je pense qu'elle a une utilité dès lors qu'il s'agit d'identifier des discriminations. De mieux en comprendre les mécanismes et les raisons et aussi les vices et à Sidi remédier et nos amendements ne

La meilleure performance de l'index dans un 1er temps et peut être j'aurai une toute petite nuance avec mon collègue Daniel Breuiller, s'il s'agit pas d'obliger le gouvernement à sur les 16 il s'agit de mobiliser le 16h pour qu'ils soient consultés pour apporter au gouvernement son expérience. Voyez-vous ce n'est pas une contrainte, c'est un apport qui est à qui que que nous proposons pour le gouvernement il y a au CESE beaucoup de ressources beaucoup de richesses et en particulier lorsqu'il s'agit de comprendre à la fois la manière dont les salariés vivent leur éviction du monde du travail, la manière dont les entreprises. Et vite rejette les salariés les plus âgés et puis aussi le CESE un autre Avantage c'est qu'on y trouve l'ensemble des des des types d'activités. Vous avez tout aussi bien des grandes entreprises, l'agriculture, l'artisanat et ceux-là ont des questions différentes de de de d'emploi des seniors. C'est pas simplement qu'une affaire de texte, c'est une affaire de mobilisation de toute la société de toute entreprise bien sûr les artisans bien sûr les PME ne seront pas incluses dans le Champ parce que je ne doute pas que l'amendement sur les 300 va très probablement trouver une majorité. Pour autant, les petites entreprises peuvent avoir envie de contribuer à cet effort national pour l'emploi des seniors et consulter le CESE l'associé à la création de l'index et se garantir la plus le le la plus grande communauté autour de cette ambition est de cet objectif commun. Et le 4179. Laurence Cohen. Oui effectivement hein. Monsieur le président. Un amendement de repli qui est identique qui a été très bien présenté par mes deux collègues mais je pense que c'est important, Monsieur le Ministre, que effectivement. Vous puissiez vous nourrir de l'expérience du Conseil économique, social et environnemental. Ce sont des représentants de salariés le secteur associatif et même le le le patronat qui sont présents au CESE s'élèvent tous contre cette réforme des retraites et pour des raisons différentes, donc ça c'est intéressant d'avoir leur point de vue leur expérience, leur, leur analyse et je vais m'attacher à présenter des faits objectifs que nous pouvons partager, me semble-t-il, sur tous les bancs de notre hémicycle le taux d'emploi des plus de 60 ans. En France est beaucoup plus faible que la moyenne de l'Union européenne, ça a été souligné mais je le redis, c'est extrêmement important de l'avoir en tête le taux d'emploi des personnes de 60 à 64 ans discriminent particulièrement les moins diplômés 25% des sans diplômes sont sans emploi. À cet âge, contre 53% des diplômés de l'enseignement supérieur. Plus on avance en âge, moins on a de chance d'avoir un emploi prétendent faire travailler 2 ans de plus, celles et ceux qui ne travaillent déjà plus n'aura qu'un effet renforcer la trappe à précarité en 2019 ne 939.000 personnes âgées de 50 à 64 ans, déjà en dessous du seuil de pauvreté, un seuil de pauvreté fixé à 50% du revenu médian. Concrètement, 939.000 personnes vivent en France avec moins de 919 euros par mois. En réponse à cette réalité sociale qui doit toutes et tous nous préoccuper franchement se contenter de la publication d'un index telle que prévu sans obligation de résultat et quelque chose de totalement dérisoire. D'où le sens de notre amendement. Merci. Ensuite le 46 rectifié madame Guillotin. Voilà. Oui monsieur le le président donc l'index senior doit effectivement être un outil au service de l'amélioration et de l'employabilité et le maintien. Dans l'emploi des seniors. Il doit être en fait plus qu'un simple Index quantitatif et doit prendre en contre le bien-être et la qualité de vie au travail car on le sait tous ici, au-delà du salaire et des avantages que peut conférer un emploi les salariés aujourd'hui sont en quête à la fois de sens et d'une qualité de vie qui leur permet effect de sentir bien et de poursuivre l'emploi auquel ils sont où peut être rentré dans un nouvel emploi. Je vais juste prendre un exemple le Danemark. Qui a une prévention de l'usure professionnelle et le développement d'une culture d'entreprise qui est importante, qui mise sur un management bienveillant à l'écoute et qui sont et, dans ce pays en fait dans les entreprises s'est imposé cette bien est-ce ce bien-être au travail avec un véritable enjeu réputationnel qui fait que l'entreprise. Entre met en avant cette qualité de vie au travail. Est-ce bien être au travail. C'est pourquoi nous proposons donc dans cet index au travers de cet amendement que l'index senior soit mise en place et prennent en compte ces indicateurs relatifs à la fois au bien-être et à la qualité de vie.

Merci monsieur le président. Alors ce projet de loi se caractérise par un silence absolu sur la question des licenciements pour inaptitude des salariés vieillissants. vieillissants. Ou. Pourtant à plusieurs dizaines de milliers par an. C'est une véritable épidémie silencieuse, monsieur le ministre, il n'y a pas que des ruptures conventionnelles. Il y a beaucoup de rupture pour inaptitude. Cet amendement a donc pour objet qui a minima l'index senior permettent de disposer d'une information fiable et transparente sur ce fait social majeur. Par ailleurs, il faut absolument différencier les PME et les grandes entreprises vous voyez nous sommes aussi très sensible à ça, à ce que ces dernières disposent des moyens conséquents pour mettre en oeuvre l'index senior. C'est pourquoi la sanction doit être. Différencier notamment plus dissuasif pour les entreprises, 300 salariés au moins. À défaut, rien ne sera installée par des temps dans des temps raisonnables. Alors je je reprécise que nous avons souvent dans les statistiques. Les licenciements économiques. D'un côté et les licenciements non économiques de l'autre et dans les licenciements non économiques, il y a effectivement les licenciements pour inaptitude et il y a aussi les licenciements pour rupture conventionnelle dont dont on va beaucoup parler là effectivement prochainement pour leur taxation donc il est vraiment indispensable de pas simplement dans cette catégorie qu'on fusionnant tu des licenciements non économiques des licenciements qui ont vraiment. Des natures très différentes qui a le licenciement pour inaptitude lui est vraiment subi et à a quelques fois des conséquences on en reparlera dramatique pour le salarié.

Donc moi je maintiens simplement l'année A6 en disant que celui-ci doit être complété par cette phrase parmi ces indicateurs figurent le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour inaptitude des salariés de plus de 45. Merci et. Un amendement identique Madame Monnier. Oui. Merci monsieur le président, Monsieur le Ministre, les nombreuses limites que présente l'index senior instauré par cette réforme ont été précédemment pointé par mes collègues. Le présent amendement vise à renforcer sa portée en précisant dès à présent sans entendre l'élaboration du décret sur lequel n'auront plus de prise que cet index seniors doit prendre en compte le nombre de licenciements pour inaptitude et le nombre de reclassement pour une attitude des salariés de plus de 45 ans. La Première ministre Élisabeth Borne a elle-même admis lors de la présentation du projet de réforme. Le 10 janvier dernier que de nombreuses entreprises avaient recours à une pratique abusive voire discriminatoires qui consiste à faire partir les salariés quelques années avant la retraite. Il est essentiel de tout mettre en oeuvre pour disposer d'une information fiable et transparente sur ce phénomène d'ampleur qui concernerait plusieurs disiez de milliers de personnes par an et serait probablement amenée à s'accélérer. Avec le recul de l'âge légal de départ à la retraite.

Mais effectivement. Il s'agit de ne pas passer sous silence ce licenciement pour inaptitude mais tout à l'heure c'était juste qu'on ait les licenciements pour inaptitude et là je souhaite qu'il y ait aussi les reclassement pour inaptitude. Je crois que Alain Minau c'est aussi. Cela, moi je voulais quand même re-insister pour avoir été consultante en entreprise quand même sur le fait que vous avez des salariés qui redoutent plus que tout. La visite médicale. Il redoute plus que tout l'avis d'inaptitude pour eux c'est une catastrophe. Ils savent très bien les les les possibilités de de de reclassement. Alors vous allez me dire avant on avait une visite médicale tous les 2 ans. Ben ils sont au moins maintenant c'est tous les 5 ans donc ça leur donne un répit pour leur préjudice dans d'anxiété ceci cette plaisanterie mise à part, je voudrais quand même rappeler quand même qu'à ces âges-là ils avaient dit. Si tu dis vous avez des branches. Que se connaît bien du soin de l'aide et du soin à domicile qui ne sortent plus par retraite c'est fini plus personne au fait plus les départs en retraite dans cette branche, on a que des sorties par inaptitude et les courbes entre la sortie par retraites et la sortie par une aptitude se sont croisés après la loi 2010 hein il faut bien le savoir. Donc voilà c'est une inquiétude justifiée, ils ne sont pas anxieux pour rien. 95% des. Salarié déclaré inapte sont licenciés. Donc est-ce c'est un, un rapport de 2019 de la Haute Autorité de santé sur la désinsertion professionnelle qui le signal et ce malgré mais c'est pas toujours possible, l'obligation de reclassement, à la charge de l'employeur. Il s'ensuit alors pour le salarié, une perte durable d'emploi qui est d'autant plus grande pour les seniors. Le 3732. Monsieur Fernique. Oui, merci Monsieur le Président. Les femmes sont particulièrement victimes on l'a dit, des inégalités salariales qui se creuse au fil du temps, les inégalités liées au genre s'ajoutant aux problèmes liés à l'âge. Le montant moyen des pensions de retraite en est d'ailleurs le reflet. Donc l'introduction d'un indicateur sur le genre dans l'index senior permettrait ainsi de contribuer à ce que les entreprises publiques de manière distincte les chiffres relatifs à l'emploi des femmes ce senior de ceux des hommes seniors afin de constater plus nettement les inégalités de genre en fin de carrière constater plus nettement pour permettre dit mieux remédier, telle est l'objet de cet amendement. Oui Monsieur le Président, toujours au nom de de mon collègue Thomas dessus. Cet amendement vise en fait à garantir le fait que dans l'index senior. Il y a bien des indicateurs spécifiques aux travailleuses et aux travailleurs seniors qui occupent des emplois d'employer. Si la situation des seniors sur le marché du travail est déplorable, ce n'est peut-être pas la peine de le répéter puisque ça beaucoup a été dit qu'à 60 ans près d'une personne sur 3 n'était ni en emploi, ni à la retraite. La majorité d'entre elles en situation d'invalidité de RSA au chômage et donc de précarité mais il y a des difficultés particulières qui concerne les les personnes qui sont dans la situation d'employer et notamment les conditions de travail qui peuvent aussi être désastreux. Ce à quoi on pense moins souvent que pour d'autres métiers durée dans l'emploi est plus difficile pour les personnes les plus précaires qui exercent des emplois à forte pénibilité à titre d'exemple, 20% des infirmières finissent en invalidité. À la fin de leur carrière à cause de la pression psychologique notamment et surtout du rythme imposé par le travail qui les empêchent d'avoir une carrière complète l'index senior telle qu'il est présenté dans ce texte ne peut évidemment pas résoudre les problèmes inhérents à l'emploi des seniors et à leurs conditions de travail. C'est il pourrait rester un pansement sur une jambe de bois. Si nous ne nous ne le nourrisson pas à défaut d'un dispositif ambitieux, nous proposons de l'améliorer, notamment en ce qui concerne concerne ces indicateurs et de préciser dans le texte que la liste des indicateurs de l'index senior ainsi que leur m'étude de leur méthode de calcul seront fixées par décret, ce qui offre peu de garanties, mais qu'il est fondamental que ça examine les conditions de travail des seniors avec des indicateurs spécifiques pour les seniors occupant un emploi d'employer. et républicain vise à garantir que ces index seniors quand il y a néanmoins des indicateurs spécifiques aux travailleurs occupant un emploi d'ouvrier. Mais sur ce sont des indicateurs portant essentiellement sur la qualité de vie au travail, les aménagements de poste les aménagements d'horaires. Tout cela pour éviter les maladies professionnelles ou les accidents du travail qui sont plus importants bien sûr au delà de 60 ans et les ouvriers sont aussi ceux qui ont les facteurs de pénibilité les plus importants et dont il faut tenir compte.

Alors nous souhaitons alors on a parlé des. Voyez, mais que la liste effectivement contiennent des indicateurs spécifiques aux travailleurs seniors. Occupant un emploi d'ouvrier. Je voudrais dire en préalable que tous les travailleurs sont touchés de façon brutale par cette. Par cette réforme effectivement de façon différenciée plus pour les femmes plus pour les ouvriers, plus pour les employés. Donc. Il est important effectivement de contenu d'avoir cet indicateur spécifique aux travailleurs seniors occupant Les ouvriers seront les premiers touchés par cette réforme brutale inégalitaire. Il est nécessaire de rappeler que, selon l'Insee. 10 à 11 ans, selon les statistiques d'écart d'espérance de vie sans incapacité dite en bonne santé c'est pas pour les hommes, les ouvriers et que les hommes, comme dans une moindre mesure effectivement pour les femmes. Alors selon la dernière dernière étude de la Dares s le service statistique du travail, tout le monde connaît le taux d'emploi des seniors. Après 60 ans s'effondre, seulement 35% bon ça a été dit, je peux sauter. Mais les ouvriers. Quand même par rapport. À ça 61 ans ce n'est pas par hasard si il n'y a plus que 28% en emploi, alors que pour les cadres. À 61 ans il y a 61% des cadres mais je tiens à dire quand même que les cadres. 13% sont aussi touchés par le phénomène. À ces âges-là. 61 ans des personnes ni en emploi, ni en retraite donc 13% des cas sont dans ce sas de précarité, c'est pour ça que vous avez toutes les organisations syndicales y compris celles qui représente les catégories cadres. Si ce n'est plus le temps donc je vais m'arrêter là et je vous invite à à lire les autres points qui sont dans l'objet. Ou bien, merci. Le 3109 présenté par le Marie-. Pierre de La Gontrie. qui le défend là monsieur Assouline.

de toute façon ça va ça va pas être. Une défense très longue. Comme j'en ai l'habitude, cet amendement vise à garantir que l'index senior contiennent au moins des indicateurs spécifiques aux travailleurs en situation de handicap. Je vais y revenir à travers plusieurs amendements mais cet indicateur spécifique et est très important si l'on veut parler. De ces personnes en situation particulière, y compris par rapport à la retraite. Merci le 4183 qu'il présente dans le groupe communiste, madame Gréaume. merci Monsieur le Président, les seniors ne sont pas égaux devant la précarité selon le rapport du corps à l'âge de 62 ans près de 16 7 % des personnes se sont ainsi ni en emploi, ni à la retraite entre la cessation définitive d'activité et la retraite, l'écart est en moyenne de 2 années. Parmi ces grands oubliés, 3% sont au chômage et 13 7 % l'inactivité. Si bien qu'il ne dépendent que du RSA ou d'une pension d'invalidité ou du revenu d'accrocs l'un des grands arguments de notre Harper rapporteur doit nous dans son rapport, c'est que le taux d'emploi connaît une hausse rapide autour des années 2010 en passant de 40 sac % fin 2010 à 47,1% fin 2013. Les réformes de retraites successives ou contribué à augmenter le taux d'emploi des ça comme sac. 64 ans oui, nous vous accordons que le taux d'emploi a augmenté de 2 voix va point pour les 60 et 61 ans. Mais je cite au prix social élevé d'un allongement du sas de précarité et on en revient précisément notre amendement sur les conséquences d'une réforme des retraites, sur l'emploi des seniors. Les ouvriers ont payé un lourd tribut. Si bien que le taux de ce ni en emploi, ni en retraite a augmenté de 16. Par conséquent, en 2019, les ouvriers à 61 ans sont plus souvent ni en emploi, ni en retraite. Cette situation concerne 35% d'entre eux, les conséquences sont lourdes. Selon l'adresse, le taux de pauvreté de ces personnes et de 32% contre 7 7 % pour ceux en emploi ou à la retraite. Toutes les données statistiques le démontrent vos arguments ne sont pas recevables. Je vous dis tranquillement. Nous vous appelons solennellement retirer ce projet de loi en posant en préalable, la question du travail plutôt que de vous acharner sur les droits à la retraite. Merci. Merci ensuite. Madame Poncet mange le 3123 et ensuite, vous en avez plusieurs d'ailleurs, donc vous pouvez peut-être les présenter. En prenant le temps nécessaire. Oui merci. Alors il s'agit, là, on revient un petit peu au licenciement pour inaptitude mais de les préciser pour les les salariés de plus de 50 ans. Et sur les 5 dernières années. En effet, on y reviendra beaucoup hein les contraintes et les risques physiques se sont fortement accrues depuis 30 ans. L'adresse à mesurer ainsi. L'évolution sur 30 ans. En partant de 1984 et les dernières statistiques, c'est 2016. L'adresse, dit que l'Exposition à au moins 3 contrainte physique ou éventuellement je pourrais vous dire qu'elle. Concerne 34% des salariés

qui sont concernés par cette exposition à trois risque pour les ouvriers qualifiés ou un peu moins mais guère hein. 813 % des employés étaient exposés à au moins 3 contrainte. Ils sont 46 9 ça a été multiplié par presque quatre l'intensification du travail touche donc particulièrement les salariés les plus âgés. Et d'ailleurs. L'Observatoire Everest avait posé une question, à savoir demander aux ouvriers à 60 ans. Comment ils envisageaient. La possibilité de travailler 2 ans supplémentaires. Hé bien la moitié des ouvriers, des employés doutent que leur état de santé leur permettent à l'horizon de 2 ans de poursuivent leur travail actuel. Alors, on nous parle de reconversion à 60 ans on va arrêter peut-être le cynisme et je propose qu'on refasse cette évaluation et qu'on leur demande maintenant à 60 ans s'il se voit travailler 4 ans de plus. Ah ouais c'est pas la moitié que vous allez avoir bon j'en ai fini pour le premier amendement je passe au second. Monsieur le président, si vous permettez. peu un peu la, la même chose mais il y a, il n'y a pas que les contraintes. Physiques hein qui effectivement touche massivement. Je l'ai dit les ouvriers, les employés hein il y a aussi les contraintes de rythme et dans les contraintes de rythme. Vous allez trouver la flambée en France mais aussi en Europe. Il est vrai des risques psychosociaux. Et là. Être exposé à trois contraintes de rythme, ça concerne désormais un tiers des salariés ils étaient quasi inexistants. 30 ans avant ils étaient à 6%, et ça concerne pas seulement les cadres, là encore ça concerne massivement les par rapport à l'évolution mais aussi 53% des ouvriers qualifiés, soit 6 fois plus que 30 ans auparavant. Qu'est-ce que c'est c'est c'est rythmes c'est effectivement ces contraintes temporelles où ces contraintes de rite c'est de ne pas pouvoir quitter son emploi des yeux. Aujourd'hui 43% des salariés sont sous cette contrainte. Avoir un rythme de travail imposé par un contrôle est un contrôle humain ou un suivi informatisé concerne un tiers des des personnes. Et tous ces indicateurs d'intensité soit physique soit de contrainte par le rythme. effectivement explose et il y en a une autre qui est intéressante, c'est l'imposition de normes de production à satisfaire en une journée là et là les cadres aussi sont touchés. 21% des salariés effectivement on une contrainte temporaire sur la journée et plus grave quand même, vous en avez quand même. Non maintenant c'est 48%. Excusez-moi, c'était 21%, donc ils ont été multipliés. Et ce qui a été multiplié aussi c'est l'imposition de normes de production à satisfaire en une heure. Qui est passé de 5% à 29%. Voilà toute cette intensification du travail des contraintes de rythme, ce qui nous a. Conduit à dire qu'avant de prolonger de 60 à 62 et A64. Il faut changer le travail bien évidemment

Ainsi que les actions mises en oeuvre pour favoriser l'emploi au sein des entreprises. Parce que quand même vous voyez ça fait le lien avec les régimes spéciaux hein quand on nous dit hein mais ils vont passer dans le c'est de paix c'est pas gênant, je le répète le CDP ces deux ans maximum de départ anticipé et qu'on passe à 64 ans c'est 62, donc les femmes ouvrier les 50% qui disait à 60 ans qui pourront pas aller à 62, vous voyez. Là si on leur donne deux ans ben ce sera 62 hein. En tout état de cause, dans le meilleur des cas. Et Madame Poncet. Je vous en avez encore hein ensuite. Parce qu'il y a 2 amendements identiques qui suivent.

il supprimait la possibilité laissée un accord de branche de déroger aux indicateurs et méthodes de calcul déterminés par décret est relatif à l'emploi des seniors. oui moi je suis assez pour la hiérarchie des sources, donc effectivement je pense qu'il faut les branches c'est bien mais elles doivent être plus favorable hein je rappelle plus favorable que le niveau supérieur qui est le cadre légal qui lui-même doit respecter des règles européennes, donc des indicateurs des. Définie, claire comme des méthodes de Calais. Tu permettent des analyses. Intéressantes et y compris de façon. Comparative Je pense qu'il n'est pas normal de risquer de les faire disparaître lors de discussions de de branche parce que ces données sont précieuses. Elles sont comme elles doivent être commune à toutes les branches qui permettent une analyse globale pour les politiques publiques et pour changer le travail pour la prochaine loi ça éclairera le gouvernement, il faut des critères communs à l'échelle d'une société tout entière. Par contre bien sûr la branche peut ajouter des indicateurs pour tenir compte de sa spécificité mais. Je pense qu'il ne faut pas qu'elle en retire. merci madame mange donc maintenant amendements identiques au dernier que vous avez présenté le 4186. Le groupe communiste. 4100. Non non on va les exposer tranquillement. Allez-y Madame hein pour. Merci monsieur le président. Cet amendement de bon sens a reçu un avis défavorable de la commission alors qu'il souhaite simplement assurer une clause de non-régression sur les indicateurs mesurés par l'emploi des seniors. Cet amendement est l'occasion de revenir sur l'anthologie de cet article qui prévoyait comme pour faire croire que les marges de négociation était possible que l'index senior ne s'applique qu'aux entreprises de plus de 1000 salariés. Cette obligation de publication n'aurait concerné que 0,15 des entreprises, 6040 au total seulement un peu plus de la moitié des salariés du pays auraient été couverts par cette disposition. Les autres leur sort n'intéressait pas a priori le gouvernement, l'Assemblée nationale avait justement avant de rejeter l'article abaisser le seuil de publication à 50 salariés. Je vous remercie. merci monsieur le Président, cet amendement donc concerne la un set où nous proposons de remplacer le mot déterminé par le mot enrichir dans la phrase une convention, un accord de branche étendu peut déterminer la liste des indicateurs cet amendement vise effectivement à ne pas laisser la possibilité à la branche d'établir des indicateurs sur l'emploi des seniors moins disant que le décret qui sera pris à cet effet. Merci. Ensuite le 4189. Madame un ponceau. Merci monsieur le président. Cet amendement de repli du groupe CRCE entend s'assurer que par convention ou lors d'un accord de branche étendu. Les indicateurs retenus ne puisse être inférieure inférieure à ceux de la norme nationale le cas échéant et même si nous le regrettons défini par la loi réglementaire, je vous remercie. Merci. Ensuite le 2483, Monsieur. Merci Monsieur le Président, c'est toujours moi, pour mon, mon collègue Thomas Dossus. La réforme proposée par le gouvernement va grandement affecté les seniors. C'est la raison pour laquelle. Ils seront avec les salariés des millions dans la rue le 7 mars prochain. Le gouvernement fait un pari qu'un recul de l'âge légal augmentera mécaniquement le taux d'emploi des seniors ce fait était avéré dans les réformes précédentes mais si ce fait est partiellement avérée. Ce qui est également avéré, c'est que les seniors, les plus éloignés de l'emploi ne sont pas miraculeusement embaucher après la réforme et à chaque réforme de décalage de l'âge légal du départ en retraite. Nous avons constaté un pic de rupture de contrat de travailleuses et de travailleurs seniors des seniors sont ainsi licenciés ou placardisés sans raison basculant, le plus souvent dans la précarité. On a évoqué 100.000 pour la réforme de 2010. le texte de l'article 2 renvoie à un décret le soin de fixer la liste des indicateurs de cet index ainsi que leur méthode de calcul. Or cet article laisse également la possibilité à la négociation collective. Ce qui est une bonne chose mais de branches d'adapter ces indicateurs. Si l'adaptation de l'index peut permettre une meilleure prise en compte de chaque milieu professionnel la rédaction actuelle de l'Arctique pourrait être dommageable. Il y a un risque de dégradation. Des mesures de l'emploi des seniors qu'il convient d'encadrer. C'est pourquoi par cet. Amendement, nous demandons à ce que toute nouvelle modification des indicateurs par accord de branche ou conventions n'entraîne pas une dévalorisation des indicateurs déterminés par décret.

3734. Donc l'index senior en l'état, risque fort de ne pas permettent de réels changements de comportement des entreprises faisant preuve d'une discrimination dans l'emploi des seniors. Pour le rendre plus ambitieux le présent amendement. Propose que pour les entreprises qui ont conclu un accord de branche ou une convention relatifs à la définition des indicateurs mentionnés le bénéfice des dispositifs généraux de réduction ou d'exonération de cotisations sociales soit conditionné à une mise en place effective et au respect des indicateurs de l'index senior. Le suivant. Alors le tableau ne montre pas, c'est le 3735. C'est un amendement de repli par rapport au précédent puisque il s'agit d'un amendement presque identique, sauf qu'il ne concernerait que les entreprises de plus de 300 salariés. Et je passe au suivant, si vous le permettez. Donc c'est le 736 c'est le 3736 mais le tableau est en panne. C'est pas grave c'est 3736 donc l'amélioration de l'emploi des seniors ne passe pas seulement par la mise en place d'un index seniors ambitieux en parallèle des procédures devraient être instauré dans les entreprises pour permettre de garantir les bonnes conditions d'emploi des seniors. Nous proposons donc de conditionner les exonérations fiscales des entreprises à la réalisation d'entretien avec les salariés de plus de 55 ans qui travaille dans l'entreprise depuis plus de 3 ans. Ces entretiens. Pourraient aborder la question de la pénibilité du travail de la formation de la qualité de vie au travail et de l'aménagement du poste de travail. C'était le 3736. Est le suivant, c'est le 3737. Voilà. Donc pour faciliter la mise en place de l'index senior et le rendre effectif. Il est important et nécessaire qu'il y a une échéance clair et réalisable qui soit fixé. Nous proposons donc la fixation d'un délai précis de publication et de transmission pour les entreprises concernées, à savoir le 1er février pour l'année civile précédente et donc par dérogation présentes dispositions les indicateurs portant sur l'année 2022

par une phrase ainsi rédigée, l'inspection du travail se voit immédiatement communiqué sur sa demande. Les données ayant permis la construction des indicateurs lors de ses contrôles sur pièces et sur place. C'est pas que nous pensons que l'inspection du travail a des moyens démesurés pour aussi suivre avec vigilance ce futur index seniors mais ça nous semble absolument nécessaire. de prévoir un accès aux indicateurs de l'index senior à l'inspection du travail lors des contrôles sur pièces et sur place parce qu'à défaut d'une mesure réellement ambitieuse, nous proposons, pour notre part de revaloriser aussi les outils de contrôle de l'index senior nous proposons bien sûr de revaloriser l'implication des partenaires sociaux et c'est je voudrais le redire la mesure essentielle qui il a sur ce sujet de l'index senior mais il nous semble nécessaire que l'inspection du travail puisse également jouer un rôle de contrôle dès lors que l'index senior telle qu'il est prévu actuelle ment n'est en rien contraignant ou en presque rien contraignant excusez-moi de. Dénaturer un peu la réalité de l'index. Merci l'amendement suivant identique présentée par Madame Ferré. Par les entreprises qui sont soumises à publication d'un texte dit senior. Merci et l'amendement 4198 présenté par Madame Cohen. Oui effectivement, c'est le même amendement avec l'index telle qu'il est conçu, les entreprises d'au moins 1000 salariés seront eux tenus de faire état. D'en faire état pardon à partir de novembre 2023. Les entreprises d'au moins 300 salariés auront jusqu'en juillet 2024 et celles qui en compte moins de 50 en juillet 2025. Vous l'aurez compris, en écoutant toutes nos interventions, nous souhaitons cet index plus contraignant qu'il ne soit pas un gadget ou un badge de bonne conduite pour les entreprises mais une mesure permettant aux salariés, aux syndicats, aux représentants du personnel d'objectiver. Ce qui se passe réellement derrière les portes closes des entreprises aussi. Nous avons à coeur que sa publication soit un impératif l'index montrera en creux en réalité les pratiques des sociétés envers leurs salaires, leurs et finalement leur bien-être au travail. Sa non-publication de la, de contrevenir aux dispositions légales peut révéler en effet une politique d'emploi et de gestion des seniors problématique plus exposés aux maltraitances dans l'emploi, je pense au chantage placardisation pression au départ Exposition à des contraintes physiques ou harcèlement sont autant de pratiques que peuvent subir un certain nombre de travailleurs et de travailleuses seniors aussi le non respect de la publication de l'index constitue pour nous une voie d'entrée pour l'inspection du travail dans les entreprises, nous visons donc à permettre un ciblage des contrôles par celle-ci et la transmission des données ayant servi à la construction des indicateurs à sa demande-t-elle et le sens de notre amendement et monsieur le ministre du Travail, j'en profite pour vous dire que ça serait bien que vous donniez des moyens supplémentaires à la médecine du travail. Merci, chers collègues. Chers collègues, je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h 30 pour la suite de l'examen de ce texte. La séance est suspendue.